La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casino présenté par. Par Madame Catherine Deroche. Messieurs, Stéphane Piednoir et Claude nous hein et plusieurs de leurs collègues à la demande du groupe les républicains. Dans la discussion générale. La parole est donc à Madame, Catherine Deroche, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. La proposition de loi, il nous vous présentons cet après-midi avec mes collègues, Stéphane Piednoir et Claude Nogent reprend en partie un texte déposé en avril par les 4 sénateur de Maine-et-Loire sollicité alors par le maire de la ville de Saumur le texte étendait la possibilité d'installation d'un casino aux communes comptant dans leur périmètre un ou plusieurs éléments du Patrimoine matériel ou immatériel, propriété de l'institut français du cheval et de l'équitation Les FCE. Le texte déposé cette année a été avec les députés de Maine-et-Loire et de Corrèze des circonscriptions des communes de Saumur arnaque Pompadour que je salue Laetitia Saint-Paul, député du Maine-et-Loire qui en tribune et j'associe le premiers cosignataires nos collègues Emmanuel Capus Daniel Chassain. L'ouverture d'un casino, une source importante d'emplois et contribue de façon déterminante au développement touristique et culturel ce qui rejaillit nécessairement sur l'ensemble des autres activités de la commune où il est implanté. Participant ainsi à son animation et à l'attractivité du territoire concerné. sont sous les casinos sont souvent parmi les premiers contributeurs du budget des communes qui accueillent. Les jeux d'argent et de hasard dans les casinos font partie sont régies par un principe de prohibition qui connaît toutefois des dérogations limitative et encadré. En effet les textes en vigueur voté avant l'existence des jeux en ligne limite l'ouverture des casinos seules stations thermales, balnéaires ou climatiques ainsi qu'aux villes principales agglomérations de plus 500.000 habitants ayant des activités touristiques et culturelles particulières participant pour plus de 40% fonctionnement par exemple d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra. Ainsi que les communes dans laquelle un casino était régulièrement exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et enfin les communes ou stations classées de tourisme de plus de 15.000 habitants du département de la Guyane. Ceci a l'Avantage de poser des limites à une activité qui se doit en effet et nous partageons cet objectif qui se doit d'être strictement encadrée. Ce faisant, ceci a aussi pour effet de concentrer les casinos dans certaines zones géographiques et notamment les bords de mer ou les départements les plus urbanisés en privant d'autres zones moins dynamique de cette activité pourtant susceptibles de les aider à développer une économie locale. La législation actuelle sur l'implantation des casinos, et donc à l'origine d'inégalités territoriales peut justifier les départements ruraux du centre de la France ont notamment pour certains pour très touristique, les activités équestres qui de par leur lien avec le monde du jeu de Paris pourrait constituer le support au développement d'infrastructures touristiques telles que des casinos. Ainsi, en autorisant les villes ayant développé une activité importante en lien l'équipe avec l'équitation à ouvrir des casinos. Il serait possible de pallier l'inégale répartition de ces établissements sur le territoire. Pour cette raison, notre proposition de loi propose d'autoriser la création de casinos dans les communes, site historique du Cadre Noir et d'nationaux qui ont organisé pendant au moins 5 années avant le 1er janvier 2023 10 événement hippique de rayonnement national ou international. À ce jour, seules 2 communes arnaque Pompadour et Saumur rentre dans ce cadre, l'institut français du cheval et de l'équitation à l'opérateur public au servir au service de la filière et qui une française qui assure notamment la gestion du Cadre Noir à Saumur. Moi aussi. Une vingtaine de haras nationaux, partout en France, il est dépositaire d'un Patrimoine matériel et immatériel équestre unique. Il lui appartient de porter de valoriser, seul ou en partenariat. Ces actions se déploie sur tout le territoire sous les marques patrimonial haras nationaux et Cadre Noir dans Saumur et arnaques Pompadour sont les sièges sociaux et administratifs. Il a noté qu'il ne reste que 2 sites haras nationaux en France avec participation de l'État. Pas eau et Saumur. De plus, il faut savoir que les missions régaliennes ayant évolué, l'État se désengage sera progressivement de ses 2 sites les autres haras nationaux, une vingtaine ont été cédées ou données res Uzès encore haras national mais qui ne reçoit plus de compétition et qui n'est plus utilisé que pour des formations et de plus ce site n'est pas historique puisque construit en 1962. Conditionner l'ouverture d'un casino à l'existence d'un Patrimoine et. Participera ainsi au développement de cette filière touristique importante et assurera également un soutien à la relance de l'ensemble de la filière cheval. La Commission partageant l'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi souhaitait améliorer le dispositif en propose proposé en s'assurant que les communes visées satisfont aux critères pertinents justifiant l'ouverture d'un casino sur le territoire d'une part et d'autre part en permettant communes doté des infrastructures équestre similaire à celle de Saumur et d'arnaques Pompadour de pouvoir le cas échéant à accueillir un casino. Mes collègues coauteur Stéphane Piednoir et Claude nous hein s'exprimeront un discussion générale mais je vous remercie d'ores et déjà du soutien apporté à ce texte. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à monsieur François Bonhomme, rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre. Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Ce texte proposé par la présidente Catherine Deroche et ses collègues une ambition simple son article unique vise à répondre aux atteintes ancienne. Hé bien compréhensible des maires des territoires ruraux qui souhaitent accueillir un casino. Il s'agit plus précisément. De Saumur et d'arnaques Pompadour qui dispose dans leur commune d'équipements équestres ancestraux. Nécessitant trouver rapidement eu des financements pour assurer leur pérennité. En effet, il faut rappeler que depuis plus de 10 ans, l'État se désengage progressivement de la filière équestre laissant bien souvent. Les collectivités territoriales, bien esseulé pour entretenir et financer des activités ainsi que les infrastructures de cette filière. Or ces équipements et les événements un font partie intégrante du Patrimoine de ces territoires et. Sont de véritables atouts et levier pour attirer les touristes comme les visiteurs. Or vous le savez. L'ouverture d'un casino municipal par principe prohibés. Et depuis plus de 2 siècles l'État encadre soigneusement et de manière très stricte les jeux d'argent et les jeux de hasard. Cette interdiction est justifiée pour des motifs d'intérêt. Général qui sont la prévention des risques d'atteinte à l'ordre public et aussi à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. Néanmoins, l'exploitation des casinos fait partie des exceptions bien ancienne au principe de prohibition. Mais son étendue a peu évolué au cours des dernières années. Actuellement, seuls les seules catégories des communes qui peuvent accueillir un casino de manière dérogatoire sans les de manière limitative à l'article L. 321 tiré. Du code de la sécurité intérieure. Il s'agit principalement des communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques de tourisme ou de villes principales d'agglomérations de plus de 500.000 habitants doté d'établissements culturels spécifiques. Par ailleurs, une singularité existe depuis plus d'un siècle pour la ville de Paris. Puisqu'il est interdit d'exploiter un casino à moins de 5 kilomètres. Exception faite pour la commune d'Enghien-les-Bains. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2018 la capitale expérimente l'exploitation de 7 clubs de jeu. Et cette expérimentation de prendre faire au 31 décembre 2024. En fait l'ouverture du casino municipal nécessite une double autorisation à la fois municipales et ministérielle. L'autorisation du ministère de l'Intérieur fait notamment suite à une enquête administrative. Les services de ce ministère contrôlent et régulent alors de manière très rigoureuse. Cette branche de jeux d'argent et de hasard. Au point qu'à ce jour, il existe 203 Casino et leur nombre n'a que peu évolué au cours des dernières années. À l'issue de cette courte présentation je souhaite. Du cadre juridique, je souhaite vous exposer la position notre commission. Ses membres se sont prononcés favorablement à la proposition de loi qui vise donc à introduire une 6ème hypothèse de dérogations à l'interdiction d'exploitation des casinos. Car la commission a été notamment sensible au fait. Que les territoires ruraux ne dispose pas des mêmes atouts que les communes du littoral, c'est une évidence et qui pourrait donc être utilement Elle pourrait ainsi utilement bénéficier de l'ouverture de casino pour accroître leur attrait touristique ainsi bien évidemment que leurs ressources financières. En outre, les communes qui ont une activité équestre importantes sont déjà en lien avec l'univers du jeu. Et des paris, de sorte que l'ouverture d'un casino viendrait compléter. Une offre touristique liée aux jeux d'argent et de hasard qui est déjà existantes. En fait, les maires de Saumur et d'arnaques Pompadour ont mis en avant l'importance de l'arrivée d'un casino dans leur commune. Et ce afin de financer l'activité équestre très présente sur leur territoire ou à proximité. C'est pourquoi l'intention qui anime la proposition de loi de nos collègues de la présidente de Roche. A emporté la complète adhésion de notre commission qui a néanmoins souhaité. Améliorer le caractère opérationnel du fait. Du dispositif qui ciblent mieux. Les communes susceptibles d'en bénéficier en 1er lieu la commission des lois. A jugé pertinent de permettre aux communes disposant d'une infrastructure équestre plus réticulaire d'accueillir un casino dans leur territoire. Elle a décidé d'étendre. Mais de manière très restrictive néanmoins. Le Champ de la proposition de loi aux communes qui accueillent soit le site historique du Cadre Noir soit un haras national. Cette extension demeure donc très limité dans la mesure où, selon les informations transmises par l'institut français du cheval et de l'équitation. Seulement 8 communes pourraient éventuellement justifier de la présence d'un art dit nationale. En second lieu, la, la commission a maintenu l'exigence d'activités équestres régulière ou anciennes au sein de la commune, en effet, la commune doit pouvoir justifier l'organisation d'au moins 10 événements équestres par an. Entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023. Et en fait un 3ème lieu. Afin de conserver un lien étroit entre la commune. Les activités hippiques ou les paris sportifs qui sont associés. La commission a introduit une 3ème condition à savoir la présence du siège d'une société de courses hippiques de la commune. Au total. Le texte voté en commission de permet aux communes d'accueillir un casino si elles répondent aux 3 conditions cumulatives. Qui sont disposés de un haras national ou du site historique du Cadre Noir. Deuxièmement avoir organisé au moins 10 événements équestres donc à caractère national ou international par an au cours des 5 dernières années. Et enfin être le siège d'une société de courses hippiques au 1er janvier 2023. À l'aune de ces trois critères, le texte qui est soumis à votre appréciation offrent la possibilité d'ouvrir de nouveaux casinos mais de manière extrêmement réduite en effet. Notre commission a souhaité s'inscrit dans la philosophie de législateur qui est celle de restreindre au maximum la création d'établissements de jeux et de hasard. En fait, la commission a pris en compte l'urgence de répondre aux difficultés actuelles de financement des activités infrastructures terrestres équestre des communes Saumur et d'arnaques Pompadour. Il s'agit en effet d'une initiation particulière que la proposition de loi entend régler. Le texte issu. Du vote de la commission veille également assurer une égalité de traitement avec les communes disposant d'infrastructures similaires sans pour autant déséquilibrer la filière des casinos sur l'ensemble du territoire. souhaite, je souhaite insister sur le fait qu'il apparaît nécessaire d'envisager à l'avenir une réflexion plus globale sur les critères permettant l'installation d'un casino dans une commune un effet. Je rappelle que la flemme de l'exploitation de l'expérimentation relatives au club de jeux parisien est prévue le 31 décembre 2024 et devrait permettre à l'initiative du gouvernement d'opérer une clarification ainsi qu'une remise à plat générale des règles qui gouvernent l'installation des casinos en France dans le cadre d'un véhicule législatif plus adapté. Enfin pour conclure, mes propos. Mes chers collègues, je tiens à souligner que j'ai régulièrement échanger avec les auteurs de la proposition de loi. Et je les remercie chaleureusement pour leur concours à leur disponibilité ainsi que la qualité de nos échanges pour formuler des pistes de solutions équilibrées et consensuelle dans l'intérêt de tout cela bien évidemment de nos territoires ruraux et de nos communes. Je vous remercie de votre attention. Merci monsieur le rapporteur. La parole est à madame Sonia Backès s'secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Merci monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur François Bonhomme madame la la sénatrice. Catherine Deroche. Monsieur le sénateur Stéphane Piednoir mesdames et messieurs les sénateurs. Avec plus de 200 établissements sur son territoire. La France concentre 40% des casinos de l'Union européenne elle jouait ainsi d'une offre ludique considérables qui est un véritable atout pour l'attractivité de nos territoires. Pour les 196 communes acquis accueillant un casino. Au-delà des revenus fiscaux Directs perçu cette exploitation participe au développement d'une économie locale et d'une attractivité du territoire en créant des emplois en son sein mais aussi dans son environnement Direct. Toutefois, compte tenu de leurs critères d'implantation l'offre de Casino est inégalement répartis sur le territoire national. Elle se concentrent majoritairement sur les bords de mers ou dans les départements les plus urbanisés. D'autres zones moins dynamiques sont quant à elles non couvertes. C'est le cas de 38 départements français. Ces critères d'implantation sont le fruit de près de 2 siècles d'encadrement strict mais nécessaire des jeux d'argent et de hasard par l'État. Actuellement et conformément au code de sécurité intérieur les communes pouvant accueillir un casino de manière dérogatoire sur les communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques de tourisme ou des villes principales d'agglomérations de plus de 500.000 habitants doté d'établissements culturels spécifiques. La multiplication de démarches émanant aussi bien d'élus locaux que de parlementaires témoigne d'une volonté sur le terrain de faire évoluer les conditions d'un plan d'implantation de ces établissements. Pour autant, il est essentiel de penser cette évolution avec prudence et sagesse. Il est fondamental qu'une réforme du cadre juridique d'implantation des casinos assurent une évolution maîtrisable du nombre de casino. Compte tenu des enjeux de sécurité et de santé publique liés à leurs activités les casinos font l'objet d'une grande vigilance et attention des services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. C'est dans cet objectif que la direction des libertés publiques et des affaires juridiques procède aux interdictions administratives de jeu ou bien agrée les employés de casino. De même, le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire réalisent des audits périodiques des établissements pour veiller au respect de la réglementation réalisent des enquêtes administratives sur les employées et mobilise un réseau de correspondants territoriaux préserver la capacité du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer à moyens constants d'assurer ses missions est fondamental pour la sécurité de tous. Nous devons également penser cette évolution avec précaution et discernement pour ne pas fragiliser le réseau de casinos existants et garantir une aire de chalandise suffisante pour ces établissements. Si une remise à plat des critères d'implantation des casinos devait avoir lieu, elle mériterait également une large concertation avec les acteurs de ce secteur économique singulier afin d'étendre le maillage actuel de l'implantation des casinos en France et permettre à des communes rurales d'en bénéficier. Cette proposition de loi étend la possibilité d'installation des casinos à un nouveau cas de figure. Il est en effet proposé d'autoriser l'implantation d'un casino communes sur le territoire desquelles sont implantés au 1er janvier 2023, le siège d'une société de courses hippiques hippique pardon ainsi que le site historique du Cadre Noir ou un haras national ou ont été organisées au moins 10 événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023. 3 nouvelles communes non dotés de Casino, à l'heure actuelle, serait à l'origine éligibles arnaque Pompadour Saumur et Segré. La rédaction proposée à l'issue de l'examen en commission conduit ainsi à étendre l'autorisation d'implantation d'un casino à un nombre limité de communes si elle n'est pas une fin en soi, cette proposition de loi permet de faire évoluer les conditions d'implantation de nos casinos et d'aller vers des zones blanches. Cette évolution permet de répondre à une attente forte des territoires concernés. pour ces raisons pardon le gouvernement donnera un avis de sagesse pour ce texte. Néanmoins, nous souhaitons que la rédaction de ce texte de la de lois pardon soit retravaillé à l'occasion de la navette parlementaire afin de prévoir le cumul d'un critère tirés de l'activité hippique et d'un critère lié au classement touristique de la commune. Cette nouvelle rédaction permettra de s'inscrire dans la logique de l'article actuel du code de la sécurité intérieure, ce dernier exige toujours la vérification d'un critère d'attractivité touristique constaté par un Label nous attire également l'attention sur le risque que des ajouts dans la loi au gré de la promotion d'intérêts particuliers aboutissent à un inventaire à la Prévert de critères dépourvue de cohérence entre. Un casino est certes un atout pour l'attractivité d'un territoire, un atout pour le développement local toutefois son implantation ne peut guère faire l'économie des moyens de vigilance accrue que ces établissements mobilise face aux enjeux de sécurité et de santé publique intrinsèquement liées à leurs activités. Je vous remercie. Les parlementaires qui se sont saisis de cet enjeu qui touchent au coeur de nos territoires et aux loisirs de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci madame la ministre, hein. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union centriste pour huit minutes. Monsieur le président, madame la ministre. Madame la présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, la manne représentée par les casinos et d'un peu plus d'un milliard d'euros au 31 octobre 2021, ce chiffre d'affaires est un peu en diminution par rapport aux années précédentes. Plus de 11 milliards de flux financiers générés par les activités de la filière équine, comme l'estime l'Observatoire économique et sociale du cheval l'idée d'utiliser ces filières pour soutenir les collectivités locales et le Patrimoine n'est pas nouvelle. L'expérience la plus récente est sans doute le Loto du Patrimoine du célèbre Stéphane Bern. Les collectivités locales souffrent d'un manque de budget pour financer les infrastructures existantes, on vient de le dire, l'idée qui a donc séduit nos collègues rédacteur qui ont opéré un rapprochement entre ces 2 activités pour combler un désert ludique et profiter du revenu des Jeux est parfaitement logique et cohérente. Le texte qui nous est proposé, comme l'ont rappelé les orateurs précédents peut sembler simple et inspiré d'une certaine logique. Il s'agit d'aider au financement de l'entretien des infrastructures du Cadre Noir de Saumur. Pour ce faire, la proposition de loi comprend un article unique, qui vise à introduire une 6ème hypothèse de dérogation au principe d'interdiction générale des jeux d'argent et de hasard qui serait fondée sur l'existence d'une infrastructure et d'une activité équestre au sein de la commune. Le critère proposé par le texte est double. La commission est revenue sur la condition cumulative. Tendant à l'existence du site historique du Cadre Noir et d'un haras national sur le territoire d'une même commune. La commission a donc choisi d'étendre le Champ de la proposition de loi aux communes qui accueillent un site historique du Cadre Noir ou un haras national. En second lieu si ces 2 communes organise annuellement un nombre d'événements équestres, les événements dit hippiques ont lieu dans les hippodromes se trouvant sur le territoire de la commune voisine. La condition, la commission a donc retenu le terme équestre qui renvoie à l'ensemble des activités relatives au monde du cheval et à l'équitation. La commission a souhaité maintenir un lien étroit entre la commune et les activités et Ipik équestre et les paris sportifs en retenant comme critère d'implantation là. Présence dans la commune du siège d'une société de courses hippiques. Sur ce texte. Je suis saisi d'une double sincérité. Dès mon département l'Orne comprend à la fois un haras national le haras national du pain. Propriété du département depuis la loi trois S et le casino de Bagnoles de l'Orne donc me voilà absolument comblée par ce texte

un casino, unique dans le cadre de Saumur l'extension fragilise le texte en cela qu'il manque de négociations avec les. Les autorités compétentes comme je l'indiquerai tout à l'heure, lors des auditions non publié le rapporteur indique. Il ressort des auditions des syndicats de Casino, de l'association nationale des élus des territoires touristiques et des services du ministère de l'Intérieur, mené par le rapporteur qu'il apparaît nécessaire d'envisager aujourd'hui une réflexion plus globale sur les critères permettant l'installation d'un casino dans une commune c'est exactement ce qu'a indiqué Madame la Ministre à cet égard, la fin de l'expérimentation relatives au jeu. Parisien Parisien devra aussi être évaluée par ailleurs la facilité qui consiste à fusionner l'hippisme et l'équestre, c'est-à-dire ce qui relève des courses et ce qui relève du sport et des concours hippiques n'est pas forcément évidente pour les spécialistes, la complexité de la situation appelle une réflexion plus globale. La proposition qui nous est proposé. Malgré ses mérites, est un texte de circonstance. Qui devra être travaillée elle lance clairement le débat sur le sujet qui mérite d'être approfondie avec l'ensemble des acteurs de la filière. Les voies de financement provenant des paris en ligne et des courses hippiques sont déjà bien identifiés et serve à financer la filière l'extension dans la version de la commission complexifie le sujet et appelle d'autres réflexions d'ailleurs engagée par les autorités de tutelle et les syndicats d'opérateur parce que c'est en fait à ça qu'il faut arriver c'est qu'il y ait un débat global sur le sujet pour arriver à un bon équilibre Un texte de circonstance. Peut déséquilibrer l'ensemble de la filière. C'est ce qui s'est passé. Avec l'ouverture mains dicton du casino de Saint-Gervais les bains qui affaiblit dans le même temps, celui de Megève et celui de Chamonix donc il est vrai que les, les territoires ruraux peuvent avoir des casinos. C'est vrai qu'il faut rééquilibrer les territoires et. Je pense que la proposition a ce mérite d'évoquer ce sujet je pense néanmoins que c'est un sujet qu'il faut. Retravailler. C'est la raison pour laquelle le groupe centriste s'abstiendra sur ce texte. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion là par l'État la la présidente Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour cinq minutes. Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, l'implantation des casinos pourrait donner le sentiment d'être un sujet anecdotique ou du moins à faire l'impression qu'il est secondaire, voire marginal au regard des préoccupations. Quotidienne de nos concitoyens. Je crois que chacun conviendra dans cet hémicycle qu'effectivement l'actualité appelle peut-être à d'autres Cependant j'ai la conviction que nous aurions tort de nous désintéresser de cette proposition de loi car pour parler de mon département, la Gironde, il compte six casinos, soit autant d'expériences qui me permettent de mesurer l'impact positif de la présence de ces établissements sur notre territoire pour prendre l'exemple particulier du casino de Bordeaux. Ouvert depuis maintenant une vingtaine d'années, il représente un gain significatif pour la ville puisque celle-ci perçoit directement un prélèvement sur le produit des jeux de l'établissement qui viennent alimenter notamment des lignes budgétaires consacrés au social. Aussi sans encore évoquer les aspects juridiques, la question de l'implantation des casinos je présente donc des intérêts économiques certains pour les communes concernées. Notre pays compte un peu plus de 200, Casino, soit plusieurs dizaines de milliers d'emplois il y a un développement économique certain pour les espaces touristiques qui les accueille. De ce point de vue chacun s'accordera donc autour de l'opportunité de cette proposition de loi. Cela étant je rejoindrai certaines remarques que j'ai pu entendre déjà à ce sujet sur ce texte, l'implantation d'un casino ne saurait être une solution pérenne pour répondre aux difficultés financières que rencontrent nos collectivités dans leur ensemble. C'est un problème plus globale qui mérite une réponse généralisé à l'ensemble des collectivités no tamment lorsque nous examinons le budget mais aussi lorsque nous recherchons des solutions pour dynamiser les politiques économiques de nos collectivités sur sa dimension juridique en revanche, je suis plus circonspecte notamment lorsque je lis la rédaction de l'article L 321 1 du code de la sécurité intérieure, qui fixe une liste de dérogations permettant l'ouverture de nouveaux casinos actuellement les villes déclarées ville station thermale ou balnéaire ainsi que les villes principales d'agglomérations de plus de 5 500.000 habitants ayant des activités touristiques et culturelles particulières peuvent accueillir de tels établissements. Cette proposition de loi vise à ajouter une nouvelle catégorie. Très singulièrement liée aux événements hippiques. Je veux bien admettre le lien qui peut exister entre le monde des paris, et celui des jeux. Nous comprenons surtout que cela permettrait d'inclure les communes d'arnaque Pompadour et Saumur et dans la continuité. La commission. A assoupli davantage les critères afin d'y inclure une dizaine de communes supplémentaires, et j'en aurai si vous le souhaitez, d'autres, notamment en Gironde, si besoin. Seulement à vouloir élargir le dispositif d'autorisation, avec des critères si spécifique, ils ne viserait qu'une ou deux communes déjà bien identifiés. Autant peut être le repensée dans sa globalité pour qu'il soit moins contraignant du point de vue législatif. Enfin j'entends qu'il ne fallait pas tomber dans une forme de moralisme excessif mais je refuse aussi de faire comme si le phénomène de la dépendance aux jeunes avait rien de préoccupant. Une proposition de loi qui élargit les possibilités d'implantation des casinos ne peut s'affranchir de toute réflexion sur la promotion et le développement d'établissements de jeux de hasard et d'argent à une époque où les paris sportifs en ligne pose de grandes difficultés, notamment chez les jeunes générations le législateur se doit de faire preuve de vigilance pour ne pas donner le sentiment qui l'accompagne favorablement ce développement inquiétant au moment même où les casinos français ont connu des baisses de fréquentation significative depuis le début de l'année par rapport à 2019 à l'instar du casino de de Bordeaux prennent en charge les addictions. Mais il est toujours bon de pouvoir. Le répéter et en faire une ligne de de conduite importante même si le situation semble s'arranger en 2023, la pandémie de Covid a bouleversé les habitudes de plus en plus de joueurs préfèrent désormais les jeux d'argent en ligne malgré l'interdiction des jeux de hasard sur Internet. Cela mériterait une étude des pactes un profond dit ce que ne permet pas la présente, proposition de loi. Ce qui est fort dommage. Cela dit, le groupe RDSE reste pour l'ensemble favorable à cette proposition de loi, je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Claude nous hein pour les groupes Les républicains pour cinq minutes.

Monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues. Notre et Édouard ruraux sont trop souvent abandonnés. Alors qu'ils sont pourtant si dynamique et si innovant. Aujourd'hui plus que jamais notre espace rural mérite une véritable ambition est de plus en plus perçu par les Français comme une richesse comme un facteur d'équilibre social et comme un lieu d'épanouissement. Mais malgré cette image positive la vérité du monde rural reste mal connue et mal comprise. On ignore souvent ses besoins d'infrastructures un service public. Les dernières lois récentes comme Lausanne pour accentuer la désertification rurale et le désengagement de l'État. Un désengagement qui sonne aujourd'hui comme une alerte dans les esprits des élus qui défendent leur territoire. La filière cheval et parfois une composante importante du développement des territoires ruraux créatrice d'emplois et génératrice d'activités sportives, sociales et culturelles. La filière cheval, mes chers collègues et créatrice de lien social. Un appui au développement rural est un allié du développement durable. Le cheval. C'est aussi un acteur majeur de la culture française. L'équitation de tradition française est inscrit depuis 2011 par l'UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En Corrèze, par exemple, nous avons la chance d'avoir incité historique de la filière équestre avec le haras national d'arnaque Pompadour véritable emblème d'un territoire mais dans la filière se délite au fil du temps. La commune dans la Pompadour abrite encore aujourd'hui le siège administratif de l'Institut français du cheval et d'équitation. FCE. Cependant, devant la gestion toujours plus complexes. L'État souhaite sortir de cette filière se concentrant bien sûr sur ses missions régaliennes et c'est peut-être très normal. Alors comment compenser ce désengagement. Comment sauver cette filière équestre connu et reconnu. Bien sûr, les territoires ruraux, on l'innovation c'est lié au corps, bien sûr. Les élus ruraux font toujours preuve d'imagination et d'innovation pour faire livrent leurs territoires. Les départements ruraux du centre de la France ont notamment pour attrait touristique les activités équestres. Qui de par leur lien avec le monde du jeu et des paris Point constituer le support au développement d'infrastructures touristiques telles que des casinos. Ainsi, en autorisant les villes ayant développé une activité importante en lien avec l'équitation et à ouvrir des casinos un double objectif pourrait être réalisé, il serait possible de pallier l'inégale répartition de cet établissement, que les orateurs précédents ont parfaitement décrit et aussi sauver la filière cheval. La législation en vigueur. Bénéficie aujourd'hui essentiellement à des communes du littoral, il y a des stations thermales qui dispose déjà de nombreux atouts touristiques. Donnant à ses casinos d'ailleurs un certain monopole. À l'inverse de nos territoires ruraux bien plus enclavés. De plus, l'ouverture d'un casino là une commune est une source importante d'emplois comme il a été déjà dit il contribue ainsi de façon déterminante au développement touristique et culturel ce qui rejaillit nécessairement sur l'ensemble des autres activités de la commune où il est implanté notre participant ainsi à son animation et à l'attractivité du territoire concerné. Ils sont aussi souvent parmi les premiers contributeurs du budget des communes avec la redistribution fiscale. Alors, mes chers collègues, cette proposition de loi va au-delà de la simple autorisation d'ouverture de casino dans Casino. Il s'agit de maintenir en vie toute une filière d'une économie locale dans les communes comportant. Je le répète hein ça les caisses et un établissement de l'institut français du cheval et l'équitation et ayant développé une attractivité particulière et récurrentes liées à l'organisation d'événements équestres de rayonnement national ou international. Par exemple sur la commune d'Arnas compas d'où c'est plus de 160 journée équestre qui seront maintenus. Ce n'est pas rien, c'est la vie de ce territoire à ce dispositif. Seules quelques communes. Pour pas lourd et mur bien sûr rentre dans ce cadre, des communes qui sont des sites historiques du Cadre Noir ou daaras nationaux. De plus il n'y a pas de casinos dans ces territoires et il n'y a pas de casino au alentours. Moins de 100 kilomètres il y a pas de casinos Pompadour et je pense que son mur je connais moins bien mais ça doit être je crois pareil. Ce serait des petits établissements certes mais viable et qui paierait des taxes permettant de sauver cette filière équestre. C'est l'économie locale et l'attractivité de tout un territoire qui en dépendent. Ces ouvertures de casino assure aurait des retombées économiques aux communes dotées d'une activité équestre pluri-séculaires et permettrait d'accroître leur attrait touristique et leurs ressources financières. Chers collègues, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de défendre la multiplication de Casino. Aujourd'hui, ils savent. Il s'agit de défendre la survie de la filière équestre dans ces villes historiques du cheval et donc notre groupe les Républicains se prononcera en faveur de cette proposition de loi Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Les corps Munn d'arnaque Pompadour et de Saumur. Dans mon département de Maine-et-Loire sont de au lieu de l'équitation. Leur nom est associé à une longue tradition d'élevage et des activités équestres. Leur réputation dépasse largement nos frontières. Saumur et le site historique du célèbre Cadre Noir il participe avec ses écuyer et ses chevaux au rayonnement international de l'art équestre à la française. Son Patrimoine ces compétitions et ses infrastructures équestre constitue l'une des clés de voûte de l'attractivité de la commune. Ils irriguent l'ensemble des secteurs d'activité locaux. Le désengagement progressif du ministère de l'agriculture risque de compromettre la poursuite des activités équestres sportive à Saumur comme arnaque Pompadour et dans les territoires ruraux avoisinants. Ce texte vise donc tout simplement à introduire une dérogation à la loi afin de permettre l'ouverture d'un casino à Saumur et arnaque Pompadour. Et il s'agit d'une demande de longue date des élus locaux, des parlementaires locaux et dont je salue la mobilisation. Je salue la présence aujourd'hui du maire d'arnaque Pompadour et de sa de la députée de Saumur les notre collègue Laetitia Saint-Paul qui est dans la tribune. Ces 2 communes. Sont historiquement est intimement liés au monde équestre par cette proposition de loi de la présidente de Roche de Stéphane Piednoir. De Claude Mougin de Daniel enfin et que co-signé par l'ensemble des sénateurs de ces, de, de nos 2 départements enfin pas soutenu par l'ensemble des sénateurs et co-signé par Daniel Chassain et par moi-même. Cette proposition de loi amendé par le rapporteur. Il s'agit. Tout simplement de palier là par cette proposition de loi l'implantation également déséquilibrer des casinos sur le territoire national. Mes chers collègues. En France les casinos, vous le savez sont concentrés principalement sur le littoral, les territoires ruraux du centre du pays sont totalement à à de rares exceptions près, laissés de côté quand on sait à quel point ces établissements sont un atout pour leur territoire. Nous ne pouvons que le regretter l'implantation d'un casino. Cela a été dit. Par notre collègue. Claude Mougin contribue de manière déterminante au développement touristique et culturel local, son exploitation est une source importante d'emplois à l'année et Madame la Ministre vous l'avez dit cette vraiment une source d'activité économiques pour le territoire dans lequel il est implanté l'implantation d'un casino dans ces 2 communes seraient donc une chose excellente et ce d'autant plus pour répondre à la question de Claude Mougin que pour ce qui concerne Saumur le casino le plus proche est à 106 kilomètres puisque c'est le Petit Casino de La Roche posait donc il n'y aura pas de concurrence pour répondre à notre collègue Nathalie Goulet, il n'y aura pas de grosse concurrence avec le, les autres casinos. C'est la raison pour laquelle la majorité du groupe les indépendants votera comme de des cosignataires Daniel Chassain et moi-même pour ce texte et je voudrais rajouter. Si vous m'y autorisez, monsieur le président. Rajouter un argument qui est que c'est peut être, mes chers collègues, la dernière proposition de loi qui sera déposé par notre collègue Catherine Deroche et cela fait une raison supplémentaire pour manifester par notre vote positif notre reconnaissance pour son travail. Sur cette proposition de loi évidemment, elle ne m'écoute pas mais vous lui direz. Sur ce, sur cette proposition de loi et sur ces 3 derniers enfin sur ces trois. Mandat. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Monique de Marco pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre madame l'auteur. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Notre retrait du nôtre être du jour à l'approche des élections sénatoriales nous réserve parfois des surprises parfois non. Cette proposition de loi comprend un article unique, qui vise à être conduire une 6ème dérogation. Son possible au principe une interdiction générale des jeux d'argent et de hasard. Dérogation qui reposerait sur l'existence une infrastructure et d'une activité équestre au sein d'une commune. Cette dérogation bénéficierait principalement à de communes en France, dont l'une située dans le département d'élection des auteurs de la proposition. Outre l'opportunité d'inscrire une telle loi. 6 mois avant les élections sénatoriales qui concerneront ce département cette proposition de loi nous semble problématique sur plusieurs points. Tout d'abord la loi à travers l'addiction de de nouvelles conditions a donc pour finalité de permettre à Deville, de pouvoir implanter des casinos sur leur territoire. Nous le savons tous, et ses auteurs le défendent avec justesse en raison des critères, l'installation d'implantation des casinos est très inégal sur notre territoire. Cette inégalité d'implantation pèsent clairement en termes d'opportunités liées aux emplois Directs ou indirects générés de retombées touristiques induite par la présence des casinos. Au-delà de l'argument de la création d'emplois. Les communes qui ont des casinos sur leur territoire bénéficie d'une manne financière certaines. Pour, c'est presque 200 communes, c'est en moyenne 1,4 millions d'euros chaque année au travers d'une taxe sur les produits de jeu. En Gironde. Comme l'a expliqué ma collègue Nathalie Delattre. Nous avons six Casino et représente donc une manne financière non négligeable. Ces ressources représentent environ 30% du budget des villes. Nous entendons les besoins de la filière équestre et bien entendu les difficultés actuelles de financement des activités et d'infrastructures et Caisse des communes de Saumur et une arnaque Pompadour. Nous entendons aussi cette petite musique issue des travaux de la commission qui trouve nécessaire d'envisager aujourd'hui une réflexion plus globale sur les critères permettant l'installation des casinos sur une commune. Toutefois, nous ne pensons c'est même pas simplement pas que la solution envisagée au travers de nouveau casino pourrait remédier soit la bonne solution. Cet objectif de création d'emplois. Ce revenu espéré supplémentaire pour les communes et pour. Favoriser la filière équine ne saurait cacher les problématiques liées au casino. Notre groupe considère que la restriction d'implantation des casinos se justifie par des considérations de santé publique. Les jeux d'argent et de hasard en général et dans les casinos sont régies par un principe de prohibition rappelé le rapporteur. Leur interdiction est justifiée par des moyens motif d'intérêt général que sont la prévention des risques d'atteinte à l'ordre public à l'autre social notamment en matière de protection de la santé des mineurs. L'addiction aux jeux d'en faisant peut avoir des conséquences financières psychologiques et familiales dramatiques pour les victimes. En France, 48.000 personnes sont tentative de jeu. Selon le sociologue spécialisé Jean-Pierre Martignoni sans tenir compte du nombre de personnes insérées dans des dispositifs de régulation de jeu. Selon SOS Joueurs. 79% de ses victimes d'addictions sont endettés. Évitons d'ouvrir une brèche pour la multiplication d'installation de ses installations de jeux d'argent. Ce texte, à nos yeux ne présente qu'une des solutions envisageables peu respiration financière. Des communes. Nous le répétons souvent les baisse de la DGF, la mainmise du préfet sur de trop nombreux financements les restrictions du levier fiscal propre la suppression de la CVAE asphyxie des collectivités locales. C'est bien là le coeur du problème de nos territoires. Problème qui limitent leur capacité d'action et qui ne peut et ne doit pas être résolu qu'au travers de mesures structurelles pérenne adaptées à chaque territoire. Nous soutenons l'ambition de retrouver pour les collectivités territoriales, les moyens d'une plus grande autonomie financière. ton financière mise à mal depuis plusieurs années et plusieurs groupes très au Sénat il travaille en ce moment. Le véritable enjeu est là et pas dans l'ouverture de nouvelles portes du casino de jeu. Ce texte facilitant ces ouvertures n'est en rien une solution nous ne le voterons pas. Merci, cher collègue, la parole est à madame Nicole Duranton pour le groupe RDPI pour six minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues nous débattons aujourd'hui d'une proposition de loi importante pour réduire les inégalités territoriales. En ce qui concerne l'ouverture de casino. Cette proposition de loi vise à permettre leur installation dans les Terres de cheval qui draine chaque année. Un public nombreux pour des événements équestres et courses hippiques. Or, ces dernières sont déjà une forme de jeu d'argent et dès lors l'arrivée du casino ne fait pas de différence morale majeure et puis passion du jeu et cheval sont liées l'une offre la chance d'un instant l'autre incarne la force et la beauté du mouvement. Permettez-moi de souligner l'importance économique du secteur des casinos en France actuellement. Notre pays compte 196 casinos qui joue un rôle majeur pour notre économie dans 190 communes d'implantation privilégiée. Dans ces communes les la contribution financière du casino représente en moyenne près de 10% du budget communal et jusqu'à 80% pour certaines. De plus, la filière française des casinos représente 50.000 emplois dont 18.200 emplois Directs. Ces établissements sont des acteurs essentiels de l'animation locale et contribue au dynamisme des régions où ils opèrent. Ma région, la Normandie, Pays du cheval est un exemple concret de la richesse que peuvent apporter des activités équestres, les centres équestres normand comme par exemple comme la Cité ma collègue de l'Orne, le célèbre haras national du pain. Donc il a, lui, un casino donc proche Bagnoles de l'Orne. Attire donc ces centres attire des passionnés de chevaux du monde entier. Il offre une multitude d'activités allant des compétitions équestres à la vente de chevaux en passant par les concours de dressage et saut d'obstacle. La législation actuelle limite l'ouverture des casinos aux stations balnéaires, thermales et climatiques, ainsi qu'aux grandes agglomérations de plus de 500.000 habitants, avec des activités activités touristiques et culturels spécifiques cette concentration des casinos. Dans certaines régions a pour conséquence de créer des inégalités territoriales, sur le plan économique, lors de son examen en commission des lois, la proposition de loi a été modifiée pour garantir son opérationnalité un amendement a été adopté pour permettre aux communes de Saumur et de arnaque Pompadour d'accueillir un casino sur leur territoire. Ces villes se distinguent par leur activité équestre prestigieuses telles que le concours national d'arnaque Pompadour et la compétition Saumur complet qui attire des milliers de spectateurs chaque année. Bien sûr les jeux d'argent sont aussi un enjeu de santé publique qu'il faut considérer avec prudence l'ordonnance d'octobre 2019 sur la régulation des jeux du hasard démontre l'engagement du gouvernement envers la protection des citoyens. La transparence, Laurence et l'intégralité dans le domaine de jeux d'argent et de hasard en effet elle a créé l'Autorité nationale des jeux, doté de pouvoirs renforcés encadrer la privatisation de la FDJ et préserver le contrôle rigoureux sur ses activités. Le titre de du livre III du code de la sécurité intérieure prévoit des je vois le dispositif pour par lequel les communes peuvent demander l'ouverture d'un casino. Ce dispositif comporte une possibilité d'appel de la décision préfectorale et celle d'octroyer des dérogations tout en étant d'accord sur le principe on peut donc interroger le véhicule législatif choisi ouvrir des casinos seulement dans les stations thermales. C'est la double peine pour les autres départements touristiques qui méritent aussi leur part de frissons et de jackpot ces territoires méritent leur tour de roulette ouvrons-leur les portes de la chance. Cette ouverture permettrait de développer davantage ses infrastructures touristiques et contribuerait à l'épanouissement économique local. De plus, ce texte n'est pas dépourvue de garantie les communes éligibles devront avoir organisé au moins 10 événement hippique de rayonnement national ou international, pendant une période d'au moins 5 années avant le 1er janvier 2023. L'amendement adopté en commission précise que les communes doivent disposer soit du site historique du Cadre Noir soit d'un haras national et doivent être le siège d'une société de courses hippiques au 1er janvier 2023. De plus, elles doivent avoir organisé annuellement au moins 10 événements équestres en en cours des cinq dernières. Années cette PPE le PPL pardon offre une opportunité unique de dynamiser ces deux villes Saumur et arnaques Pompadour en leur permettant d'ouvrir de casinos, cela aurait un impact positif sur l'emploi en créant de nouvelles opportunités pour les habitants de ces régions, les casinos sont connus pour offrir une variété de postes allant des croupiers au serveur en passant par les agents de sécurité et les responsables marketing ainsi l'ouverture de casinos permettra à ces villes de stimuler l'économie locale, l'emploi et d'offrir aux habitants de ces territoires des événements culturels Hatem dîners spectacles et animations au sein des lieux uniques bien souvent des offres financières spécifiques sont négociés pour les locaux. Cela aura également un impact positif sur les commerces locaux tels que les hôtels, les restaurants, les magasins, les attractions touristiques. Les retombées économiques seront significatives, créant ainsi un cercle vertueux de développement de prospérité et d'attractivité. Les autres pistes d'extension des dérogations pour ouverture de casino explorée par les amendements de mes collègues Franck Menonville pour les plans d'eau et elle Joseph pour les départements frontaliers mérite également d'être discutées ici en conclusion cette proposition de loi oeuf l'occasion de réduire les inégalités territoriales et d'envoyer un message fort sur notre engagement en faveur de l'équité des territoires. elle peut être perçu comme un effort trop sectorielles trop spécifique à peu de villes et n'a peu n'appelle pas la nécessité d'en faire une loi. Les membres du groupe RDPI voteront chacun en toute liberté sur ce sujet. En ce qui me concerne je voterais pour, La parole est à monsieur Joël Bigot pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour cinq minutes.

Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi très spécifique. Pour permettre à deux communes d'ouvrir un casino dans les communes de Saumur en Maine-et-Loire. Et ça ne s'invente pas. Arnaque Pardo Pompadour en Corrèze. Ce texte vient répondre utilement une demande ancienne des élus locaux et notamment du son roi. En 2019. Lors de l'examen de la loi pacte je partais avec mes collègues de Maine-et-Loire Catherine Deroche, Stéphane Piednoir. Un amendement visant le même objectif. Permettre l'ouverture de casino dans les villes accueillant l'Institut français du cheval et de l'équitation. Nous voulions ainsi préserver le Patrimoine équestre et la très touristique de ces communes. En leur apportant des moyens financiers apte à garantir la pérennité d'une filière initialement. D'une filière cheval en France. Cet amendement n'avait malheureusement pas pu être discutée, pour des raisons d'irrecevabilité. Cette proposition de loi s'inscrit dans la continuité de ce travail transpartisan et est conforme à l'objectif d'attractivité du territoire. Nous espérons donc l'adoption de ce texte consensuel qui au regard des déclarations du président de la République devrait recueillir l'assentiment du gouvernement en effet. Interpellé sur le sujet par le maire de Saumur en 2019 lors du grand débat national Post gilets jaune. Le président de la République, il avait promis. Comme à son habitude, que la commune recevrai l'autorisation avant la fin de son premier quinquennat, est-il indiqué même ne pas confondre ne pas comprendre les freins juridiques à la réalisation d'un tel projet. Depuis, certains élus disposent même d'un engagement écrit de la présidence de la République favorable à cette implantation. Les modifications actées par la commission la semaine dernière précise et améliore la proposition de loi initialement déposé. La nouvelle rédaction permettent en l'occurrence de lever les difficultés posées par les conditions cumulatives d'existence du Cadre Noir et d'art national sur le territoire d'une même commune alors que c'est là, cela n'est pas le cas tant pour Saumur que pour arnaque Pompadour. L'ajout d'un critère pour la commune, bénéficiaire d'être le siège d'une société de courses hippiques au 1er janvier 2023 mais également d'avoir organisé annuellement au moins 10 événements équestres au cours des 5 dernières années. Me paraît suffisamment restrictif pour encadrer le dispositif proposé. Ainsi la version actuelle permet de clarifier et rend opérationnels la volonté des auteurs de la proposition de loi à laquelle je souscris. Elle devrait néanmoins également inspiré nos députés impliqué sur ce sujet pour qu'ils concourent à l'adoption finale de ce texte au plus tôt. Les retombées attendues en termes d'attractivité. Sont très importantes pour la Maine et Loire et notamment vous l'avez compris pour la ville de Saumur. De l'aveu même du maire il escompte entre 200.000 et 300.000 visiteurs supplémentaires par an. L'activité pourrait ainsi générer entre 60 et 100 emplois selon la taille de l'établissement. Et les recettes fiscales sont non négligeables de un à 2 millions d'euros par an, auxquels s'ajoutera un soutien à l'activité équestre. Ce texte permettra de toute évidence d'apporter des solutions à nos territoires qui n'entrait pas dans les critères actuels de la loi. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je salue cette initiative de notre assemblée qui arrive à point nommé. Les élus de Maine-et-Loire et d'ailleurs peut se rendent compte en acte que la chambre des territoires demeure toujours attentive à leurs usages locaux. Le Sénat est dans son rôle lorsqu'il rappelle l'exécutif à ses promesses. Je souhaite enfin utiliser cette tribune pour enjoindre nos députés à se saisir de ce travail pour aboutir rapidement sur ce dossier qui n'a que trop duré. Tous les feux sont au Vert tâcher d'en assurer un dénouement heureux. Je voterai donc pour cette proposition de loi, ainsi qu'un certain nombre de mes collègues, même si la majorité de ceux de mon groupe ne s'y opposera pas je vous remercie. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Cécile Cukierman. Pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Merci monsieur. Le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi sur laquelle nous nous apprêtons à débattre, se présente comme un outil pour réduire les inégalités territoriales, via l'ouverture des casinos. Je crois et je vous l'avoue, nous n'avons pas la même définition de lutte contre les inégalités, puisque votre proposition de loi ne concerne à l'origine que de communes dans un pays qui en compte plus de 35.000, en changeant un seul mot monsieur le rapporteur, je le reconnais, vous avez élargi à 13 communes. Cette proposition de loi. Vous pourrez en convenir, cela reste encore très faible et je parle bien évidemment de ces communes qui peuvent accueillir les différents événements et caisses mais nous pourrions y compris, et de façon très sérieuse, s'interroger sur les communes qui accueillent des gros événements et qui ne peuvent privilégié d'une autorisation pour ouvrir un casino. Il faudrait donc mais je l'avais dit en commission mener une réflexion d'ensemble sur les règles d'implantation des casinos et finalement arrêté de parler d'inégalités territoriales entre des communes alors que la ville de Saumur reçoit une dotation globale de fonctionnement à hauteur de plus de 7 millions d'euros pour 26.000 habitants. Ensuite, on ne peut utiliser je crois l'ouverture d'un casino pour simplement pallier à la perte des moyens financiers des collectivités qui sont une réalité d'ailleurs nous avions lors du projet de loi de finances au Sénat. Voter l'injection de cette DGF pour l'année 2023 sur l'inflation sur a été retiré dans le cadre du 49.3 c'est fort regrettable. Chaque année il y a donc moins de ressources directes pour les collectivités. Il faut donc que l'état qui se désengage depuis des années, soit responsable face aux besoins de toutes nos communes et ce n'est pas une délégation de service public via les casinos qui permettra toujours assez Budgets de pouvoir résister. Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne certaines collectivités dépendent essentiellement de cette ressource. Le rapport de la Cour des comptes souligne les limites de cela et nous ne pouvons avancer ni prendre de décision sans prendre en compte la crise sanitaire par exemple que nous avons traversé la crise énergétique que nous vivons actuellement. Dans le rapport de la Cour des comptes, on note la dépendance forte de certaines collectivités à cette ressource, surtout en période de crise, elle s'oppose au retournement de la conjoncture économique en faisant reposer le financement de charges récurrentes et pérenne sur les recettes en provenance du casino local ce risque a été visible à deux reprises je disais pendant le confinement et après le confinement avec les restrictions sanitaires certaines recettes ont ainsi chuté de 20, 30 voire 50% le prélèvement sur le produit des jeux représentent près de 30% des recettes réelles de fonctionnement je laisserai donc au plus mathématiques d'entre nous faire les ratios vous défendez le fait que l'ouverture de casino permettra de répondre à des enjeux liés à l'emploi à l'économie locale au tourisme. Mais certaines communes d'ailleurs en témoigner de l'effet limité de son installation et pour autant, certaines communes qui ne bénéficient pas de Casino ont ont également de l'emploi de l'économie locale et un développement touristique important. Nous pourrions également regretté dans une. En l'absence d'une loi d'envergure qui viserait je disais à repenser réellement l'installation et les règles d'ouverture de casino pour l'ensemble des communes de notre pays, qu'il prendrait également en compte. Cette difficulté liée notamment à l'addiction aux jeux à ses conséquences sur la vie des gens et comment en partenariat, y compris avec une politique publique avec les responsables et les gérants de casinos et d'ailleurs je sais. Qu'un certain nombre y sont très attentifs, nous pourrions avoir une politique de prévention en la matière. Sans réelle réflexion change sur l'implantation des casinos, vous l'aurez compris. Sans surprise, nous ne pouvons être favorable à cette proposition de loi simplement et je le souhaite oeuvrons pour pouvoir être utile à nos collectivités dans le cadre du prochain débat budgétaire et donner les moyens nécessaires et indispensables à nos communes pour pouvoir bâtir sereinement leur budget dès l'an prochain. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. C'est le président, madame la Ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. La France compte actuellement 200 casinos répartis dans 63 départements, nous 38 départements français sont dépourvus. Rappelons que que ces établissements sont également des complexes de loisirs intégrant des spectacles, des animations culturelles et artistiques de la restauration et Initiée par Napoléon en 1804 afin de lutter contre la clandestinité des jeux d'argent. L'implantation de casinos dans notre pays est régie par une vieille loi, une loi de 1906 qui souhaitait la réserver aux villes thermales ou balnéaire par conséquent l'implantation des casinos est très hétérogène sur notre territoire avec une très forte présence le long du littoral dans les grandes stations touristiques et dans les villes d'eau en lien étroit avec le tourisme, donc, mais sous une forme restrictive. Partant de ce constat avec mes collègues du groupe Les Républicains ma collègue Catherine Deroche du Maine et Loire Claude Mougin de Corrèze. Nous avons d'abord souhaité grâce à cette proposition de loi que nous vous proposons aujourd'hui élargir le Champ des possibles en la matière et rectifier ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme une inégalité territoriale tout en restant fidèle à cette. Caractéristique touristique et tous ceux qui connaissent ce beau département de Maine-et-Loire savent que la ville de Saumur remplit parfaitement ce 1er critère. Au coeur du Parc régional Anjou Touraine est posée sur ce fleuve royal qu'est la Loire. Citons parmi ses nombreux atouts, son château ses troglodyte ces caves, bien sûr et même son marathon qui s'est tenu dimanche dernier. Avec les coauteurs de cette proposition de loi. Nous sommes convaincus qu'il faut renforcer l'attractivité de cette belle ville qu'on dit souvent endormi et il ne fait aucun doute que l'implantation d'un d'un casino contribuerait à la fois au renforcement de son rayonnement touristique et à son développement économique. Il ne faut pas oublier que les casinos sont des établissements créateur d'emplois souvent le principal employeur d'ailleurs de la localité dans laquelle ils sont implantés. Cela représente environ 15.000 emplois Directs, que ce soit pour l'activité de jeux pour la restauration hôtellerie l'animation, l'accueil, la sécurité auxquels on peut ajouter 30.000 emplois indirects supplémentaires. Une centaine d'emplois, ça a été dit serait ainsi générer avec l'implantation d'un casino à Saumur, sujet très régulièrement mis sur la table depuis plusieurs décennies. Enfin les retombées financières potentielles se mesure aussi sur le budget des collectivités locales concernées à hauteur de 30% par exemple à Deauville soutenir ce projet donnerait donc incontestablement des marges de manoeuvre intéressante aux élus pour porter des initiatives créatrices de valeur. Mais il y a évidemment et ça a été évoqué plusieurs fois une autre dimension tout aussi essentiel, la filière équine. L'École de cavalerie et ses nombreux manèges font partie des véritables fierté et de l'histoire de cette sous-préfecture de Maine-et-Loire Saumur ville du cheval s'il en est accueille le siège social de l'institut français du cheval et de l'équitation FCE institut public au service de la filière équine qui assure la gestion du Cadre Noir de Saumur et des haras nationaux. Il est dépositaire d'un Patrimoine matériel et immatériel unique en France qui lui appartient d'entretenir et de valoriser. Or celui-ci souffrent depuis quelques années d'un désengagement fort de l'État, fragilisant l'ensemble de la filière. Particulièrement sensible au soutien qu'il convient de lui apporter ces temps n'étroite collaboration avec l'FCE eux. Que nous avons souhaité écrire cette modification de l'article L 321 1 du code de la sécurité intérieure qui régit l'implantation des casinos dans notre pays. Toutefois, comme toute modification dérogatoire d'un texte de loi existant, il convient d'être mesuré. C'est donc dans cet esprit d'équilibre que nous avons limité, cette nouvelle dérogation aux communes accueillant des sites historiques de haras nationaux ou du Cadre Noir clairement. Cela ne concernerait concrètement que quelques villes et tout particulièrement Saumur et arnaques Pompadour. Y compris avec d'ailleurs la nouvelle rédaction de la commission sous la conduite du rapporteur François Bonhomme dont je salue l'excellent travail. Je termine par la question de l'accès aux jeux d'argent. Dans l'absolu, on peut considérer que. Toutes mesures de facilitation pourrait inciter un public plus nombreux à à céder à la tentation, voire à tomber dans les travers d'addiction dont on connaît les dangers potentiels. Mais ce serait pour moi à tenir un discours d'un autre temps. En faisant abstraction des changements radicaux de pratiques que l'on observe depuis une dizaine d'années. Rien de plus facile en effet aujourd'hui. Pour des foyers y compris pour des foyers aux revenus modestes que d'acheter un jeu à gratter ou de s'inscrire tout simplement sur une plateforme de jeux en ligne. Le buraliste connaît bien ses clients et c'est les mettre en garde contre les dépenses excessives de même le croupier la Casino a l'expérience nécessaire pour repérer le joueur qui s'enflamme et dont la banqueroute pourrait finalement nuire à l'établissement lui-même pour toutes ces raisons, mes chers collègues, vous l'avez compris, je vous demande le plus entier soutien à ce texte à cette proposition de loi, je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Daniel Chassain. Pour le groupe les indépendants pour 2 minutes. Monsieur

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Saumur et Pompadour ont des activités équestres mondialement connu Pompadour bénéficie de la réputation de son haras et de l'ancienneté de ses activités équestres, on les doit, notamment, la famille de Pompadour. À l'origine de la construction du château de Style flamboyant et de ses écuries cette dynastie s'arrête en 1728, Louis XV achète le château et l'offre à sa célèbres favorite qui va devenir ainsi la marquise de Pompadour. Il décide. À Arras, inspiré par la qualité des pâturages Limousin. À la révolution, le haras devient bien national il est vendu puis réquisitionné par Napoléon Bonaparte, pour être un bien public. Sous Napoléon III le sénateur Brunet empêche la privatisation du château, puis la République. Conserve le arabes pour la guerre et aussi l'activité équestre. Par la suite le domaine accueil progressivement le siège de plusieurs grandes organisations équestre le. Les pas des haras nationaux puis les FCE depuis 2010, mes chers collègues. Voici un très bref résumé de l'histoire prestigieuse de Pompadour et de son art. L'activité d'élevage est très importante sélection reproduction mais aussi des activités sportives Jumping hippodrome qui ont des retombées économiques très importantes sur la commune et ce territoire rural. Le vote de ce texte. Donnerait la possibilité aux communes de Saumur et bien sûr Pompadour d'avoir un casino pour Pompadour le nom l'histoire de ce lieu de son haras national mais aussi l'absence d'un casino dans un rayon de 100 kilomètres, sont des données en faveur de ce projet. De plus les retombées financières permettront de maintenir les 160 journée parent d'activité sportive équestre nationales et internationales à Pompadour si importante pour l'activité. de l'économie et du tourisme suisse territoire comme cela a été dit par mes collègues. Je vous invite donc à voter cette proposition de loi. Si cher collègue. La parole est à monsieur. C'est une Bourget pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur, chers collègues. La France compte plus de 200, Casino, cela a été rappelé l'objectif initial de cette proposition de loi qui est d'offrir la possibilité à deux communes arnaque Pompadour en Corrèze et Saumur en Maine-et-Loire de se doter chacune d'un casino objectif légitime et recevable au regard du droit positif en vigueur cette faculté écarté malheureusement ces deux communes en effet des conditions permettant l'ouverture de tels établissements et réglementer strictement par l'article 321 tirer 1 du code de la sécurité intérieure sont pour l'heure autorisée à se doter d'un casino, des communes qui ont un statut de communes balnéaires, thermales, climatiques ou les communes Centre des grandes métropoles dotées d'équipements culturels particulier. le choix de ces communes est un choix arbitraire qui comprennent une surconcentration de ces établissements sur les littoraux et dans une moindre mesure dans les communes thermales laissant de nombreux territoires français écarté de la possibilité de se doter de ce type d'établissement. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui avait donc l'objectif d'élargir ce champ dans sa rédaction initiale. Elle permettait en effet de d'ouvrir cette possibilité aux seules communes dotées de sites historiques du Cadre Noir et des haras nationaux ont organisé pendant au moins 5 années a minima 10 événement hippiques par an au rayonnement national ou international. Jugeant que ces critères cumulatifs rendez la présente, proposition de loi difficilement opérationnel. Monsieur le rapporteur a préféré modifier la rédaction de son article unique, cette modification de la législation en vigueur, devait permettre l'ouverture à terme d'une douzaine de nouveaux casinos supplémentaire en France. Le texte originel pouvait faire sens dans la mesure où les activité hippique et équestre alimente grandement le monde des paris, et donc des jeux d'argent dont les casinos tirent leurs recettes cependant la nouvelle rédaction nous interroge et nous inquiète si de nouveau casino n'étaient pas de nature à bouleverser les équilibres territoriaux en la matière. Qu'en est-il de l'ouverture potentielle d'une douzaine de nouveau casino. nous il dit-on aucunement que ces nouveaux établissements constitueraient des sources nouvelles d'attractivité économique et touristique pour les communes qui les accueille. Pour autant, nous ne pouvons adhérer à cette libéralisation excessive pour au moins 2 motif que je vais vous exposer. Le 1er motif et qu'il est à craindre que l'ouverture d'une douzaine de nouveau casino ne viennent bouleverser cette activité et mettre encore plus en difficulté. Cette filière qui est déjà fragilisée par l'essor des jeux de hasard et des jeux de paris en ligne. La 2ème. Raison pour laquelle cette libéralisation nous inquiète c'est la fréquentation des casinos à la pratique des jeux de hasard et les paris en ligne qui sont source d'excès de dépendance et d'endettement pour certains de nos concitoyens aussi au cours de ces 5 dernières années, les dépenses de jeu des Français ont augmenté de 12,5%. Par ailleurs, 1,6% de nos concitoyens, ça donnerait à une pratique excessive en la matière, soit plusieurs centaines de milliers de personnes et particulièrement au sein des milieux sociaux défavorisés populaire et paupérisé nous partageons donc les réserves et la prudence qui ont été exprimées tout à l'heure lors de leurs interventions, aussi bien par notre collègue Nathalie Goulet que par la ministre lorsqu'elle a pris la parole ces réserves étant exprimé une fois n'est pas coutume, les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain Bénéficieront d'une liberté de vote sur ce texte lié à la fois aux enjeux locaux tels que nous l'a précisé tout à l'heure notre collègue Joël Bigot nous comme je le disais à Pompadour, Saumur, oui mais l'ouverture à une dizaine de nouvelles communes, ça n'est pas nécessairement raisonnable nous partageons donc ses réserves, nous partageons cette prudence et nous laissons une liberté de vote aux membres de notre groupe dans sa majorité, le groupe socialiste, écologiste et républicain s'abstiendra sur cette proposition de loi. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Édouard Courtial. Pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le président de la commission des lois. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Faire plus avec moins, c'est ce que casse-tête récurrent que les élus locaux doivent résoudre au quotidien. C'est donc naturellement que les communes cherchent de nouvelles sources de revenus. Les casinos en tant que jeu d'argent et de hasard sont régies par un principe de prohibition ce principe salutaire que cette PPL ne remet nullement en cause vise à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. Et si l'on peut comprendre que les dérogations à la prohibition de principe d'implantation des casinos concernent des villes ayant une culture du tourisme on peut néanmoins s'interroger sur les inégalités territoriales résultant de cette logique en effet cette logique a finalement contribué à rendre encore plus attractif des communes ayant déjà de forts atouts touristiques. L'objectif de la PPL et donc de lutter contres les inégalités territoriales sans pour autant supprimer l'interdiction de principe des casinos et transformer les villes françaises ont autant de mini-Las Végas. L'extension prévue se limite aux communes ayant un lien particulier important avec l'activité hippique en effet ces communes partagent déjà une relation étroite avec l'industrie du jeu et des paris, du fait des paris hippiques qui prennent place. Un casino dans la commune ne ferait que compléter une Oeuvres déjà présentes et permettrait à la commune de dégager une nouvelle manne financière. Cependant, je m'interroge sur le caractère trop restrictif de cette définition en effet, cette nouvelle opportunité ne semble concerner que de communes en France. Arnaque Pompadour et Saumur. Ainsi, elle exclut des communes de 1er plan en matière hippique qui méritent tout autant de se voir accorder l'ouverture d'un casino sur leur territoire. Et je pense évidemment en particulier au sud de l'Oise caractérisée par ses nombreux haras ou à des communes hippique de 1er plan comme la cité impériale de Compiègne ou encore Chantilly capitale du cheval, n'en déplaise à Fontainebleau plus grand centre d'entraînement de chevaux de course d'Europe un musée vivant du cheval attirant chaque année 200.000 visiteurs. 197 courses hippiques par an dont les prestigieux, je le rappelle. Prix du Jockey Club et de Diam 2000 personnes vivant de la filière hippique. Pourquoi alors chantilly aurait telle une activité pluri-séculaire autour du cheval moins importante que ce mur et arnaques Pompadour cette PPL, je le redis à de bonnes intentions et des effets positifs mais je regrette son caractère trop restreint. J'ai envisagé d'amender le texte mais j'aurais sans doute remis en cause l'équilibre fragile ainsi trouver je lance donc cet appel Madame la Ministre, chers collègues, en faveur d'une ouverture plus large qui bénéficierait également à cette terre de chevaux quel was et je vous remercie. Et nous avons 2 amendements. Le 1er monsieur Menonville. Offrir la possibilité aux communes riveraines d'un étang salé ou d'un lac supérieur à 1000 hectares d'implanter un casino donc supérieure à 1000 hectares donc soumis à la loi littoral actuellement donc seules. Certaines villes communes stations balnéaires, thermales et climatiques peuvent qu'y souscrire. En effet, donc l'ouverture d'un tel établissement contribuer complète le développement économique d'un territoire et son animation touristique. Les lacs soumis à la loi littoral accueillent des bases de loisirs. Qui proposent donc des activités nautiques de plein air des hébergements de la restauration, l'ouverture d'un casino donc permettrait de compléter l'offre touristique.

Donc c'est quand même un élément important. Deuxièmement, je rappelle que la proposition de loi vise à bien sûr à trouver de de nouveaux sources de financement mais. S'inscrit quand même et s'appuie sur le fait qu'il y a un lien entre les jeux d'argent et de hasard avec les courses hippiques ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est une raison pour laquelle. je suis défavorable à cet amendement. Je demande son retrait à défaut et également. Ça a été dit dans les propos de de plusieurs intervenants, on considère que, on atteint le rendez-vous de 2024.

Merci, monsieur le Président effectivement donc votre amendement propose d'ouvrir la possibilité aux communes riveraines d'un étang salé ou d'un lac. D'une superficie super supérieures à 1000 hectares d'implanter un casino en fait de nombreuses communes sont riveraines de ces étant et l'adoption de votre amendement conduirait à ouvrir la possibilité d'ouvrir un casino à l'ensemble de ces communes. Aucun mécanisme de régulation de l'implantation des casinos qui relèveraient de ce nouveau critère. N'est par ailleurs prévue. Dès lors, l'ensemble des communes riveraines d'un lac ou d'un étant donné pourraient être être pourraient toutes se doter d'un casino. Ce qui n'apparaît pas opportun. Ce que nous vous proposons d'une manière générale sur cet amendement mais globalement. Sur les demandes de faites par par le sénateur Courtial tout à l'heure et sur un certain nombre de demandes qui ont été faites, c'est que dans le cas de la navette parlementaire, nous travaillons. Avec les services de l'État pour voir quels sont les critères qui permettent. Le cas échéant d'élargir mais avec un cadre. Correct. Donc pendant la navette parlementaire. En attendant, nous vous proposons le retrait de cet amendement. À défaut, nous serons défavorable. Merci. Il est battu. Il est pas. Donc je le mais voix avec 2 avis défavorables l'amendement numéro inquiet pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté la l'amendement numéro 2. Qui le présente. Madame Joseph. la mise en place de casino peut contribuer au développement de nos territoires dans le respect de la législation et et selon des critères objectifs qui souligne le caractère exceptionnel de cette activité. Donc cet amendement propose. D'éteindre l'autorisation de casinos dans les territoires qui en sont encore privés et envisage donc la possibilité d'une ouverture de. De casino pour chaque département frontalier, qui en seraient dépourvus, mais dans une ville classée commune touristique. Membre d'une intercommunalité à fiscalité propre et plus de 100.000 habitants. Donc cet amendement. Indique un rééquilibrage salutaire dans l'implantation des des casinos en inscrivant donc dans la législation spécifique. Ce souci d'aménagement de nos territoires, qui reste absent des dispositifs actuels. Donc cet amendement présente pour moi et mon collègue Marc Laménie des Ardennes un intérêt pour tous nos territoires frontaliers en évitant en particulier des fuites fiscales importantes vers la Belgique ou le Luxembourg récupérer donc cette assiette fiscale et il y aurait d'ailleurs un rapport de l'administration centrale sur ce sujet un refus serait incompréhensible, d'autant que le gouvernement s'était engagé dans ce sens dans le cadre du pacte Ardennes le 15 mars 2019 lors de sa signature. Donc ici. Pas de dépenses publiques, bien au contraire un atout touristique certains est un enjeu stratégique pour inciter à la consommation en France, en Belgique et non au Luxembourg, notamment pour tous les départements frontaliers du Nord-Est. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, je comprends parfaitement l'intention de de notre collègue. Donc qui oppose deux 3 3 conditions cumulatives, à savoir être cité dans un département limitrophe un département frontalier

Alors si j'ai bien compris. Parfaitement l'l'intention de de de notre collègue. Je crois qu'il est important quand même de dire que dans le même cadre de de de veiller à ne pas bouleverser l'implantation actuelle des des des casinos aujourd'hui en France et de prévoir de s'inscrire dans la clause de revoyure de 2024 est prévu par. La révision des des des statuts de Paris en 2017 qui prévoit ce rendez-vous en 2024 après l'expérimentation pour remettre en doute, sans doute à plat cette question. Des zones transfrontalières et de l'implantation plus équilibrée des casinos sur notre territoire. Merci. Donc c'est un avis défavorable, madame la Ministre. Merci Monsieur le Président effectivement votre amendement vise à répondre à la situation particulière. Des départements frontaliers dont les habitants en l'absence d'offre de jeux en France vont jouer dans les casinos étrangers. J'observe qu'en plus il tend à limiter le nombre de casino qui pourraient être ouvert avec un triple mécanisme de de contrôle. Un seul cas des un seul casino par département frontalier. Le casino de peut être ouvert que dans une commune, classée et la commune en question doit être membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100.000 habitants. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'en remet à la sagesse de cette assemblée. Oui, monsieur le président, madame la ministre. Globalement. Comme je me suis exprimé lors de la discussion générale le notre groupe était assez hostile momentanément à l'extension en attendant une une étude plus poussée mais alors mettre un casino à la frontière luxembourgeoise. Quand on travaille sur la fraude fiscale, ça c'est vraiment un amendement contre lequel je je je je, sur lequel je vais voter évidemment contre. On a déjà tellement de problèmes de blanchiment. On va pas mettre en plus une lessiveuse, à la frontière. Merci madame Joseph. Je remercie le gouvernement pour son avis de sagesse. Bon courage évidemment mes collègues à voter cet amendement. Je rappelle que. Il y a eu il y a une il y a une réflexion à l'heure actuelle, je l'ai entendu sur une possibilité d'évolution donc des critères relatifs à à l'implantation donc des qui a été demandé en 2019 par le ministre de l'Intérieur. Ce travail me dit on. A abouti donc qui permettrait de donner une une base législative à ses demandes d'ouverture de casino. Et dans ce rapport. La ville de Sedan comme celle de Saumur seraient cités. Donc pour moi c'est une occasion de revenir sur cette carte relativement ancienne donc hein c'est clair des casinos en France qui résulte de de de de texte assez ancien et qui privilégiait à l'époque des communes touristiques et thermales.

mais je crois que l'argument. Et bon je je respecte l'intervention de notre collègue Madame le goulet mais les Ardennes c'est le le le Luxembourg n'est pas très loin mais ne notre plus proche frontière c'est la Belgique Historiquement. Les les casinos sont implantés dans les stations thermales et dans les Ardennes, on a aussi beaucoup de stations thermales et il se trouve que il y a réellement et. Il y a un volet turban. Pas pact Ardennes qui a été fait il y a quelques années par notre collègue notamment notre collègue député Jean-Luc Warsmann et puis aussi un certain nombre de, de représentants des collectivités territoriales en liaison avec. Le gouvernement bien entendu pour justement avec une fiche pour l'implantation de de casino en secteur frontalier et la Belgique et à deux pas et c'est quand même dommage, ça serait dommage que je dirais, on a eu une fuite ma ma malheureusement vers

a aussi vraiment des arguments forts et je crois que ça concours réellement à l'attractivité des territoires et dans le volet pacte urbain notamment, donc je soutiens et merci aux collègues qui nous soutiendrons et puis merci aussi à Madame la Ministre pour son avis de sagesse. Merci. Merci cher collègue. Donc je me mettre aux voix cet amendement de avec un avis défavorable de la commission un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour.

Merci. Qui est contre. Qui est contre bien la main à ceux qui sont contre ce.

Qui s'abstient. Il est adopté. Donc. Mes chers collègues, je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi. Le vote sortie qui voudra bien sûr vote sur l'ensemble de la proposition de loi.

Une seconde, Monsieur le Président. Même la ministre et chers collègues, je voulais juste dire à Catherine Deroche et aux auteurs que notre position n'est absolument pas dirigé contre la proposition initiale mais qu'au plus tôt dans son extension que les amendements qui ont été déposés en séance et le débat qui a eu lieu montres qu'il y a besoin d'un vrai débat. Il y a déjà au sein du ministère de l'Intérieur. Des négociations avec les, les opérateurs, je pense qu'il est extrêmement important qu'on puisse les poursuivent madame le ministre a parlé d'une navette Swat, mais j'espère qu'au moins ce sera ce texte ne sera pas frappée de l'urgence du fait de façon à ce qu'on puisse en débattre tranquillement avec toutes les études d'impact et les évolutions qui sont probablement nécessaires. C'est la raison pour laquelle nous nous abstenons favorablement. Merci donc je mais au voilà cet article unique. visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casino. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. La proposition de loi être adopté. Je vais suspendre la séance. Quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point lors du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure. Après 6 ans d'un travail scrupuleux et objectif dans la pure tradition du Sénat. Oui je peux l'affirmer la France agricole décline. Au-delà du risque de perdre notre souveraineté alimentaire, je pense que nous pourrions dans un avenir proche. Si nous continuons comme cela connaître leur risque de la sécurité alimentaire. D'ailleurs les événements Covid et la guerre en Ukraine nous on fait toucher du doigt cette réalité pourtant improbable il y a si peu de temps. La proposition de loi que nous avons écrit avec mes 2 collègues Pierre et Serge que je remercie a pour but de mettre fin à ce déclin. De mettre fin à cette naïveté coupable bien française qui consiste à empêcher de plus en plus la production chez nous tout en fermant les yeux sur l'ouverture de plus en plus grande des portes de nos importations. Nous ne pouvons plus continuer à nier les évidences. À force d'interdire à force de stigmatiser à force de ne pas regarder la réalité en face. Notre pays achètent ils l'achètent de plus en plus. Et la France devient de fait de plus en plus dépendante des autres. 60 et 11% des fruits sont importées 85% du coulis de tomate est importé 56% de la viande de mouton est importé. La débâcle de notre agriculture s'explique par les mêmes raisons que celles qui ont ruiné notre industrie ou le secteur de l'électricité et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le choix de l'État, conditionnée par une minorité qui terrorise la majorité nous conduit dans une stratégie malthusienne fondée sur le tout monter en gamme. Mais au moment où la pression du pouvoir d'achat est maximale. Cette stratégie s'avère une erreur fatale. Obligeant à déclasser. Plus de 40% du lait bio tandis que les produits d'entrée de gamme et de moyenne gamme sont importées. Alors notre pays doit se repositionner rapidement comme une grande puissance agricole en donnant la priorité à la souveraineté alimentaire. Ce qui implique d'augmenter la production de répondre aux besoins du marché de masse, de s'opposer frontalement à la logique décroissante du projet farm to Forks qui planifie la dépendance et la famine. Notre prose position de loin pour un choc de compétitivité de la ferme France peut y contribuer à travers ses 26 articles. Je remercie les 174 sénateurs, qui ont cosigné cette proposition de loi et je leur dis de cette tribune, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car vous êtes élus de toutes les campagnes de France vous là les, vous la connaissez cette lente agonie qui s'accélère. N'ayez pas peur de redonner de l'espoir à nos paysans car vous les connaissez mieux que quiconque. Et vous connaissez leur désarroi face à toutes ces injonctions contradictoires. N'ayez pas peur enfin de ces messages de chantage et d'intimidation sous couvert d'écologisme car nous sommes largement majoritaires à penser qu'il vaut mieux produire en France plutôt que d'importer de l'autre bout du monde. Alors, mes chers collègues. Comme l'a dit Clémenceau. Nous avons eu le courage de le dire maintenant il nous faut avoir le courage de le faire. Alors soyons fiers de notre agriculture et votant cette loi. Merci à tous. La parole est à monsieur Pierre lourd. Auteur de la proposition de loi pour 3 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous sommes devant une réalité. L'agriculture française et de moins en moins compétitives. Les jeunes ne veulent plus devenir agriculteur. Un certain nombre de branches professionnelles travaille 70 heures par semaine pour gagner la moitié du SMIC. Il y a urgence à réparer un certain nombre de moyens pour que l'agriculture française redevienne compétitive. Nous avons laissé s'effondrer de notre industrie. Nous avons laissé s'effondrer notre production nucléaire. Les conséquences sur notre souveraineté sont graves. Allons-nous maintenant regardez notre agriculture disparaître. Notre souveraineté industrielle et alimentaire se dégrader ça chaque jour sans réagir. C'est pour cette raison que nous avons décidé de proposer cette loi d'urgence agricole qui a été enrichi par les travaux de notre rapporteur Sophie Primas. À l'occasion de l'examen en commission. Les mesures ils font forte mais lorsqu'un fruit et légumes sur 2 consommée en France est importé lorsque la moitié des poulets consommés en France sont importés. Lorsque les éleveurs laitiers doivent travailler 70 heures par semaine pour gagner la moitié d'un SMIC. Nous avons besoin de mesures fortes. Les mesures sont fortes mais n'en font pas moins empreinte de bon sens. Réduction d'énormes baisse des charges, sécurisation de l'accès à l'eau le 20 des frères à l'innovation, voilà ce dont nos agriculteurs ont besoin. Ces mesures ne sont pas non plus anti-écologique. On peut parfois l'entente dans ces très midi. Elle fait une régression que de permettre l'épandage de perte de pesticides très ponctuellement sur des zones ultra ciblés plutôt que d'arroser tout le Champ. Je conclus en mentionnant une disposition qui me tient à coeur, celle relative au Livret A gris. Cette idée n'est pas nouvelle, au Sénat et comme bien souvent, il fait son chemin. Elle va permettre aux Français de se rapprocher de son agriculture de placer leur argent disponible sur un livret qui permettra aux agriculteurs et à toute la production agricole d'investir de manière urgente. C'est à l'heure où les taux d'intérêt remontent et donc où l'investissement pour l'adaptation et de résilience face au changement climatique. Du côté de nos concitoyens ce nouveau livré leur permettra de témoigner tout leur attachement à l'agriculture. Le gouvernement annonce un plan de relance pour l'industrie. Qui met en avant la réduction des délais administratifs de moitié. Il faut étendre cette mesure à l'ensemble de l'agriculture qui n'en peut plus. Face à une sur-réglementation. Le moral des agriculteurs est au plus bas. Les jeunes ne veulent plus être agriculteur et on ne forme pas un agriculteur en quelques mois. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi va permettre de résoudre d'accompagner les agriculteurs dans ce changement.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Répondre à l'urgence, répondre à la crise. Donner aux agriculteurs français. Les moyens de nous nourrir, voilà l'objectif 1er de ce texte, un texte qui fait parler un texte critiqué et pour cause, ils traitent de sujets majeurs, il n'est pas seulement un focus sur l'agriculture. Mais il interroge notre relation à l'alimentation à notre souveraineté alimentaire à nos différents modèles agricoles à son adaptation au changement climatique ou encore à notre modèle de société et notamment notre relation entre urbain et rural. Difficile, voire impossible de trouver un consensus quand on aborde ces questions. D'ailleurs, le texte que nous examinons aujourd'hui est un texte de compromis qui se bat sur des constats eux sans appel du rapport que mes collègues Laurent Duplomb et Pierre Louÿs au avant et moi-même avons publié en septembre dernier. Pour reprendre une expression la ferme freins se brûle notre modèle agricole décline notre marché est submergée par des importations de denrées qui ne respectent pas nos exigences environnementales, sanitaires et sociales. Notre agriculture aucune nos. Agriculteurs ne parviennent plus à écouler leur production. Tout simplement à gagner leur vie, ce texte j'en conviens, est loin d'être parfait. Et j'ai d'ailleurs toujours fait part à mes collègues de mes réticences sur le volet pesticides et notamment l'article 13. met ce texte vise à stopper l'hémorragie contenir l'incendie chercher des solutions concrètes pour sortir la ferme France d'une crise dans laquelle elle s'est engouffrée depuis plus de 20 ans. La détresse des agriculteurs, leurs difficultés, je les connais pour y avoir consacré une grande partie de ma vie professionnelle, mon département, la Dordogne, est un département rural et ce rapport tout comme cette PPL, ils y ont été bien reçu. Les agriculteurs et nos concitoyens, notamment les plus modestes compte sur nous. Ces derniers n'achète pas tous bio ou moins qu'avant, non pas par dogmatisme mais tout simplement car ils n'en ont pas les moyens. Difficile de consommer 100% bio ou sous signe officiel de qualité. Cantona SMIC pour trois enfants, alors on se contente de produits importés moins chers mais de bien moindre qualité. Être de gauche, c'est combattre les inégalités. Or, la première d'entre elles c'est le contenu de l'assiette. J'en suis convaincu, donner à nos agriculteurs de moyen de nourrir tous les Français avec nos normes de qualité supérieure à celle de nos voisins est un moyen pour concrets pour lutter contre ces inégalités et aller vers une agriculture durable, une agriculture. Relocaliser que j'appelle sincèrement de mes voeux. Poursuivons cette stratégie d'importations massives actuelles c'est contribuer à l'érosion progressive de notre souveraineté alimentaire. Enfin parce que cette loi ne se limite pas aux questions de pesticides, ce texte parle de compétitivité ainsi que d'innovation et d'adaptation au changement climatique. Nous souhaitons donner aux exploitations des moyens d'investir dans ce tas d'appellations changement et dans l'évolution de ces pratiques. Je me réjouis donc qu'un diagnostic carbone figure dans cette loi, il s'agira d'une première Pierre vers le développement de ce dispositif outils. Essentiels tels transition des exploitations agricoles et point de départ, utile à la démarche de l'eau de labellisation de pour conclure ce texte il issu d'une initiative transpartisane. Il a le mérite de mettre les questions d'agriculture et notamment de souveraineté alimentaire au coeur de nos débats, à l'aube de la grande loi agricole annoncé par le gouvernement. La parole est à madame Sophie Primas présidente et rapporteur de la commission des affaires économiques pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la compétitivité agricole et pour les auteurs de cette proposition. Un sujet majeur c'est d'abord un impératif pour protéger notre modèle agricole français si singulier et si éloignée des modèles industriels décrié pour lui permettre de faire perdurer cette agriculture en faisant émerger des générations de jeunes agriculteurs motivé à la double perspective d'une juste reconnaissance de leur importance et d'une juste rémunération. La compétitivité. C'est ensuite de corollaire de l'investissement et donc de la modernisation continue de notre agriculture hier de sa mécanisation pour sortir les agriculteurs de la pénibilité aujourd'hui pour permettre l'adaptation aux conséquences du changement climatique et aux attentes sanitaires, environnementales et alimentaires de la société. Enfin la compétitivité est une obligation ardente si nous Français souhaitons restons rester durablement maître de notre alimentation en quantité et en qualité. Par conséquent je tiens une fois encore à le dire et à le répéter la compétitivité n'est pas l'ennemi d'une agriculture durable. Pas plus que la durabilité ne peut s'opposer à la compétitivité, le temps de ses oppositions doit cesser et je sais, Monsieur le Ministre, que sur ce point nous nous rejoignons. Alors pourquoi faire un texte aujourd'hui sur la compétitivité, depuis les états généraux de l'alimentation et les loi Egalim la politique du gouvernement repose sur 2 pieds d'une part une exigence environnementale à nul autre pays européen pareil se traduisant par une explosion en chaîne des normes et donc des charges pesant sur les agriculteurs. D'autre part un encouragement à la montée en gamme pour bonifier les revenus encouragements qui se traduit en réalité par une fuite en avant, comme l'a parfaitement décrit le rapport sur la compétitivité de la ferme France cependant à l'heure où les Français font face à une grave crise du pouvoir d'achat et à une forte inflation. inflation. Uniquement à toujours plus de monter en gamme et donc toujours plus de normes et de charges liées c'est pousser les Français les plus modestes à acheter des produits étrangers qui pour certains ne sont produits ni dans les normes françaises, ni même dans les normes européennes. Nous observons aujourd'hui dans les faits, ce que nous redoutions ici au Sénat depuis toujours une alimentation à 2 vitesses, une alimentation française normer labellisés la pluie à la part la plus aisée de la population et une alimentation d'entrée de gamme d'importation pour ceux qui ont des fins de mois difficiles. En définitive, mes chers collègues. À force de ne plus jamais parler de compétitivité, on ne s'occupe ni de la fin du mois des Français ni de la fin du monde ni de la faim dans le monde. Aujourd'hui, cette proposition de loi transpartisane de nos collègues fait suite à leur rapport de la sur la compétitivité de la ferme France elle entend poser les jalons essentiels de l'agriculture de demain compétitive durable sobre en intrants attractive pour les jeunes arrivant stockage et partage de l'eau, incitation à l'innovation, baisse des charges, lutte contre les surtranspositions, formation continue des agriculteurs adaptation au changement climatique. Les 26 articles de cette proposition de loi enrichies en commission aborde des sujets fondamentaux pour l'avenir de notre agriculture. L'enjeu de ce texte, c'est la place de notes agriculture en Europe et dans le monde sa résilience et son rôle face au changement climatique, sa capacité à renouveler ses exploitants. Mes chers collègues, je vous présente aujourd'hui un texte cosigné par plus de la moto. C'est de cet hémicycle améliorer en commission et qui je l'espère saura susciter un débat sans caricature ni opposition stérile entre 2 types d'agricultures supposées irréconciliables les auditions d'ailleurs souligné à quel point dans sa très grande majorité le monde agricole, ces filières comme ces organisations représentatives souhaité voir assumer la thématique de la compétitivité. Ce thème nous le déclinons en 3 axes, le premier axe porte sur la lutte contre les distorsions de concurrence, véritable fléau de la compétitivité de notre agriculture face à nos concurrents. Les surtranspositions sont vécu douloureusement par nos agriculteurs quand ils doivent se plier à des exigences toujours plus grandes qui n'existent pas ailleurs et notamment chez nos principaux concurrents européens. La commission a ainsi enrichi les prérogatives du haut commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires créée dans ce texte, véritable guichet unique des problématiques des filières, il pourra être saisi rendre ses avis publics au sujet des normes et des surtranspositions. Loin de se substituer à vous Monsieur le Ministre. Il sera votre meilleur allié sur ces sur-surtransposition je souhaiterais m'attarder sur le très commentée article 13

non plus nous donnons simplement Ministre de l'Agriculture ce qui semble avoir réclamé dans les derniers temps, la possibilité de faire réaliser sur des cas particuliers une balance bénéfice-risque de la décision et ainsi d'éventuellement suspendre temporairement prend une décision d'interdiction de la. Lorsque celle-ci n'est pas synchronisée avec les autres États membres qui n'existe pas de solution de substitution ou qu'il existe des et des risques avérés pour la pérennité des productions agricoles ou des outils agroalimentaire qui mettrait ainsi en risque notre souveraineté alimentaire, c'est pour vous Monsieur le Ministre, le meilleur le moyen à la fois de pousser parallèlement la recherche fondamentale et appliquée sur les productions en péril. Et également de pousser l'Europe à prendre des décisions communes à tous les agriculteurs européens en même temps et ainsi d'assurer l'équité concurrentielle de notre agriculture, mais aussi la sécurité sanitaire de l'ensemble de l'Union européenne en même temps également je pense là qu'il s'agit d'un juste équilibre trouvé en commission le 2ème grand axe de la proposition de loi de notre collègue entend modéré les charges de nos agriculteurs pour que leur revenu ne soient plus la variable d'ajustement de la compétitivité. Déduction pour épargne de précaution pérennisation du TO-DE. Exclusion des entreprises. Ah ah ah production saisonnière du bonus-malus, ce sont des sujets que nous aborderons lors des discussions mais qui sont très importants, les. La commission d'ailleurs les a rendus budgétairement budgétairement abordable enfin le 3ème et dernier grand axe de cette proposition de loi vise à encourager le renouvellement des pratiques, l'innovation et ainsi accompagner l'agriculture dans sa nécessaire adaptation de dispositifs encourage et accompagne l'investissement un crédit d'impôt d'une durée de 3 ans qui vise à soutenir les investissements dans les secteurs les plus intensifs en main-d'oeuvre et la création d'un livret A gris qui aura la double vertu de resserrer les Liens entre les agriculteurs et les actes et les Français et celle d'orienter l'épargne vers les investissements agricoles y compris d'ailleurs l'acquisition du foncier pour les jeunes agriculteurs. Par ailleurs, 3 dispositions concernant l'usage de l'eau ont été adoptés et améliorer par la commission, nous aurons sans doute l'occasion d'aborder cette problématique d'actualité et facteur majeur de compétitivité et enfin s'il me reste un petit peu de temps je voudrais ici mentionné l'autorisation de l'usage des drone pour la pulvérisation aérienne de précision. Il ne s'agit évidemment pas d'autoriser la pulvérisation tous azimuts par des avions et des hélicoptères. Il s'agit d'une mesure nécessaire si l'on veut encourager et accompagner l'innovation faire de réels progrès dans la baisse des intrants et susciter des vocations parmi les plus jeunes. Cet article 8 ressort de son passage en commission sous la forme d'une expérimentation limitée aux terrains agricoles en pente et à l'agriculture de précision. Nous sommes bien loin de la caricature, encore une fois c'est davantage par la recherche par l'investissement et l'accès à l'innovation que tous les agriculteurs pour tous les agriculteurs que nous assurerons la résilience de notre agriculture et l'attractivité de de ces métiers. Je n'ai pas pu être exhaustif tant les 26 articles ouvrent des champs diversifiée. Je suis certaine que notre discussion sera riche en séance si elle sait éviter les effets de manche pour conclure je tiens ici à le redire avec force notre agriculture n'attirera pas les jeunes arrivant si elle demeure enserrées dans un carcan de normes toujours plus nombreuses et complexes les unes que les autres si l'on étouffe la production et l'innovation, par l'application irraisonnée d'un principe de précaution devenu principe d'inaction. Si l'on continue à pointer du doigt une profession qui pourtant change. Évolue innove et dont les pratiques répétons-le sont déjà parmi les plus vertueuses du monde et enfin si l'on ne permet pas et c'est peut-être le plus important une juste rémunération des agriculteurs, les agriculteurs ont une noble mission, celle de nourrir nos concitoyens et de nourrir une partie de la planète afin d'assurer les grands équilibres géopolitiques, celle d'être totalement acteur et aussi bénéficiaire de la lutte contre le changement climatique. Il est nécessaire et vital pour la nation, de les soutenir de considérer toutes leurs missions et de les rémunérer dignement pour cela, Monsieur le Ministre, soyez assurés que ces thématiques continueront d'être portés par le Sénat, à l'occasion, à l'occasion des prochaines échéances agricole. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Marc Fesneau Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. monsieur le président, madame la présidente de la commission que je salue également en sa qualité de rapporteur. Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, du plomb, monsieur le sénateur Murillo, Monsieur le Sénateur relou. Une lente et inquiétante érosion de notre souveraineté agricole et alimentaire. C'est en substance le constat du rapport de la mission d'information sur la compétitivité de la ferme France. 2 septembre 2022 au Sénat qui a inspiré la proposition de loi dont nous allons débattre. Il serait sans doute plus juste de parler de rapport au pluriel, car en réalité, cette proposition de loi, elle aussi, est aussi l'aboutissement d'un travail initié en 2019 avec un 1er rapport d'information de Laurent Duplomb. Je voudrais aussi avant d'en venir aux constats et aux mesures proposées saluer la qualité du travail mené par le Sénat depuis le constat éclairant posée par le travail de la mission d'information, jusqu'à cette proposition de loi cosignée comme vous l'avez rapporté. Pour plusieurs par plus de 170 parlementaires issus de cinq groupes politiques différents. Et je voudrais naturellement salué le travail de votre rapporteur ainsi que de la commission et de ses services et la qualité des échanges que nous avons toujours eu en vue de l'examen de ce texte. C'est un débat utile que nous allons avoir alors que la concertation sur le pacte et le projet de loi d'orientation et d'avenir agricole que j'ai lancé en décembre dernier qui a eu lieu dans tous les territoires dont vous êtes les élus s'achèvera prochainement. Je souhaiterais tout d'abord. Évoqué les constats qui ont nourri cette proposition de loi pour vous dire ce que je peux naturellement en partager une partie, pas tous mais une partie sans doute n'aurons-nous pas tout à fait en effet la même appréciation sur ce que le président de la République et le gouvernement ont fait. Essayé de mettre en oeuvre depuis 2017 pour répondre aux difficultés notre agriculture, notamment en terme de compétitivité et donner de nouvelles perspectives à l'agriculture, je pense notamment aux allégements de cotisations pour a tourné à l'à la création d'un fonds de portage du foncier dont le prix en France est un élément d'attractivité au soutien à la modernisation de notre outil de production avec France relance ou France 2030 ou à des réformes plus structurelles comme les loi Egalim le variant de l'eau et de l'adaptation au changement climatique ou la réforme de l'assurance-récolte. Je pense aussi à la question des clauses miroirs et la la réciprocité des normes qui pour la première fois été mis à l'agenda européen, même si nous devons aller plus loin et faire en sorte que ça se généralise. Elles sont au coeur de la bataille que nous avons et que nous devons mener pour garantir à nos producteurs français l'équité, la loyauté par rapport à nos concurrents étrangers. De la même manière je ne présenterai pas la stratégie du gouvernement comme celle du monde tout monter en gamme à vrai dire d'ailleurs sur la stratégie du monter en gamme, c'est une stratégie ancienne je ne vous ferai pas l'offense de dire la date à laquelle on a créé les IGP les AOC, il y a une volonté continue en France de la montée en gamme reconnaissons aussi d'ailleurs que, y compris dans les échanges internationaux, les produits qui sont les plus grands rendu sont ces produits-là et donc c'est une oeuvre continue ça n'empêche pas d'ailleurs qu'on puisse se poser d'autres questions comme l'a souligné le rapport je pense que la question est plutôt de savoir ce qui le rapport de la montée en gamme et ce qui est la nécessité de de conforter toutes les gammes pour répondre à l'ensemble des des demandes des consommateurs. C'est plutôt cet équilibre-là qu'il faut trouver, je n'ai pas entendu d'ailleurs autre chose dans vos propos plutôt qui nous position entre d'une part la montée en gamme et de la satisfaire les besoins de tous les consommateurs. Ça fait donc je disais 60 ans que nous développons des signes officiels. De qualité, combien ont été créés. D'ailleurs ces 5 ou 6 dernières années. ce soit beaucoup moins que ces 60 dernières années dans le discours que le président de la République a prononcé à Rungis, il me semble que la qualité plutôt était plutôt présenté comme un élément qui permettait également de créer une rémunération supplémentaire. Assumons collectivement, c'est plutôt une fierté d'avoir porté ses signes de qualité, quand vous regardez d'ailleurs y compris en installations agricoles. Je pense à certains types de fromages, les endroits où on installe plus c'est souvent les endroits où il y a des labels de qualité, je pense aux par exemple. Pour ceux qui sont de cette région et ceux qui ne sont pas d'ailleurs aussi, donc le signe de qualité peut aussi un puissant levier pour installer des jeunes et donc assumons c'est plutôt une fierté, me semble-t-il c'est signe de qualité dans notre pays à l'extérieur de nos frontières. C'est un atout pour nos exportations, ça n'empêche pas de travailler sur les autres sujets au-delà de ces divergences, bien sûr, il me semble comme vous que la perte de souveraineté alimentaire que les auteurs du rapport font d'ailleurs remonter à la fin des années 90 est un élément absolument majeur. Il me semble que nous pouvons collectivement tiré quelques enseignements pour relever les défis auxquels notre agriculture fait face. D'abord se dire que ce qui a été défait pendant des années ne pourra se reconstruire. Du jour au lendemain. Et il faut donc poser les enjeux et avancer des solutions avec humilité. En assumant aussi la complexité des sujets en refusant de tomber dans les caricatures et je sais que cette proposition de loi, on a pu être l'objet. La présidente là la rapporte votre rapporteur l'a évoqué, de grâce, essayons sur ces sujets. En tout cas j'essaierai d'y veiller. Pour ma part dans ces débats ne pas caricaturer les positions et c'est quand même assez regrettable que sur le sujet agricole on soit obligés en permanence de tomber dans les caricatures ou de vous faire tomber dans les caricatures quand nous défendons au fond la même chose, c'est-à-dire la volonté de compétitivité, la volonté de de défend les agriculteurs et la volonté de défendre les différents modèles d'agriculture et donc je sais que c'est des préoccupations. Vous avez et je suis de ceux qui regrettent que parfois on ait pu qu'arrêter raturer ce texte au-delà des désaccords que nous pouvons avoir le 2ème élément c'est naturellement celui du changement climatique qui se pose aujourd'hui avec une urgence inédite, c'est qui va forcément constituer un impératif pour penser ce que nous devrons mettre en oeuvre pour bâtir notre souveraineté alimentaire la souveraineté alimentaire sera durable et résilientes ou ne sera pas qu'un autre agriculture ne pourra pas produire en quantité et en qualité suffisante. Sans une adaptation des systèmes de production pour préserver l'accès aux moyens de production que sont les seuls la biodiversité et les ressources naturelles pour ne citer que l'une d'entre elles mais la plus éminente l'eau. Et donc souveraineté ne s'oppose pas à transition pour que la souveraineté soit assumé. Il faut que nous assumions aussi des transitions qui sont nécessaires et on a besoin de le dire aussi aux me semble-t-il, en vérité aux agriculteurs. Dire cela ne veut pas dire que l'on doit pudiquement fermé les yeux sur des problématiques comme celle de la compétitivité. Vous avez eu raison de le rappeler, les uns et les autres ou de la compétitivité, près de la pris de l'agriculture, au contraire. Ces questions elles existent, elles sont au coeur de cette proposition de loi, elles sont aussi au coeur des défis que nous devons relever pour l'avenir de notre agriculture et elles sont également présentes dans toutes les concertations sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricole à laquelle j'ai pu assister dont et qui me remonte la compétitivité, ça n'est pas un gros mot et dire que depuis trop longtemps. Nous croyons en France qu'une norme qu'une interdiction produit une solution ce n'est pas remettre en cause notre ambition environnementale et sociale. Dire que nous ne pouvons pas le faire seul. Comme si nous étions sur une île avant tous les autres partenaires et concurrents européens. C'est au contraire considérer qu'il y a un lien indissociable entre la souveraineté alimentaire. Le changement climatique et et la sécurité alimentaire, ça n'est pas en rabattre c'est regarder les choses dans la réalité des faits, dire que nous avons besoin de transition. Ce n'est pas en rabattre sur les objectifs, c'est se donner une perspective et des moyens pour les atteindre parce que si nous sommes sans cesse en train de produire de nouvelles normes et de nouvelles contraint contraintes comme une espèce de course folle devant nous. Pour notre agriculture c'est l'existence même des outils de production agricole et agroalimentaire dans nos territoires qui se posera et des actes, et l'existence même des agriculteurs et des agricultrices dans nos territoires qui se posera et c'est bien ce que nous avons sous nos yeux et c'est bien ce qu'a rappelé le rapport. C'est donc notre capacité à assurer l'accès à une alimentation en quantité et en qualité suffisante, notamment aux plus modestes qui seraient posées, c'est l'importation dans nos assiettes de produits qui ne respectent pas nos standards environnementaux qui deviendrait la norme c'est notre vocation exportatrice, qui peut être aussi un élément de stabilité géopolitique qui serait remise en cause, alors même que la guerre en Ukraine nous rappelle cruellement l'importance de l'enjeu de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Tout cela se tient. Et donc la question c'est celle de l'équilibre du chemin à emprunter mais ce ne peut être en aucun cas d'opposer impératif productif et impératif climatique.

D'abord parce que j'ai voulu que cette concertation puissent débuter sur la base de constats factuels et non pas autour d'objets politiques prédéfinies. Je crois que c'est aussi cela qui fait que les acteurs qui y participent. Salut à ce stade, un exercice plutôt réussi. J'ai voulu que l'on a sur le respect de la diversité des avis des pratiques des solutions des modèles que les acteurs puissent se projeter à l'horizon 2040 et que nous assumions ensemble des objectifs européens et français en matière climatique environnementale, sociale et de souveraineté tout en assurant, donc notre souveraineté alimentaire, c'est sans doute cela la réussite à ce stade de la concertation, faire en sorte que les agriculteurs puissent reparler de ce qu'ils font. Car c'est un élément important de reconnaissance et du pacte que nous leur devons mais aussi mettre autour de la table des personnes issues d'horizons différents pour essayer de penser ensemble un chemin comme vous le savez, la concertation se déploie des haches sont différents et je salue l'implication et des régions et des gens de l'agriculture dans ce travail, c'est une, cette concertation parce que pour moi cette concertation à la fois une dimension nationale avec des groupes de travail ainsi qu'une dimension régionale dans les territoires tant les solutions pour une certain nombre d'entre elles seront différentes selon les territoires et les contraintes territoriales. Se tient également auprès des jeunes dans les établissements de l'enseignement agricole. Avec une consultation dédiée, de même qu'auprès du grand public, ce sont des éléments de méthode précieux sur lesquels je voudrais donc insisté et je sais qu'elle que l'initiative du Sénat ne s'inscrit aucunement dans le dans une forme de remise en cause de la concertation en cours sur le P. ah mais plutôt dans la volonté d'ouvrir avec exigence, comme vous le faites souvent un certain nombre de débats sur l'avenir de notre agriculture et de notre souveraineté alimentaire le Palois aussi sans doute vocation élargir encore le spectre des sujets dont nous aurons à débattre aujourd'hui je pense un certain nombre d'enjeux que nous devons interroger ou réinterroger pour mieux pour mieux notre agriculture au 1er rang desquels le réchauffement climatique. Je pourrais parler évidemment du défi foncier comment nous pouvons nous par exemple massifier les transitions systémique des exploitations et nous préparer à et opérer des transitions de rupture dans des territoires qui en auront besoin. Comment imaginer un nouveau cadre de financement de l'agriculture pour couvrir les besoins de capitaux. Vous ouvrez d'ailleurs en partie ses portes là sans précédent liée à la reprise d'au moins un tiers des fermes françaises. Comment répondre aux besoins d'investissements dans l'appareil productif est à la recherche et le développement pour faire face aux transitions comment améliorer l'attractivité des formations et des métiers y y compris pour les issus du milieu agricole et permettre une meilleure compréhension par la société. Meilleure compréhension et meilleure connaissance par la société des métiers des contraintes et des exigences du secteur comment faciliter, accélérer et systématiser la mobilisation des connaissances produites par la recherche, le développement et l'innovation agricole français pour accélérer la diffusion de la connaissance et rendre opérationnels les solutions et innovation face à l'accélération des situations d'impasse et impact à venir du changement climatique. Enfin bien sûr et c'est l'un des sujets également soulevée par cette proposition de loi. Comment préserver un cadre équitable et soutenable de financement de la transition de l'agriculture et limiter toute concurrence déloyale en matière environnementale climatique et sociale. Dans ce contexte de la même de la question de la compétitivité à laquelle elle ne saurait être réduite cette proposition de loi ouvre des champs de travail utile et nécessaire, soit parce qu'ils mettent à l'agenda des sujets qui méritent de l'être. parce qui sont importants, soit parce qu'ils entrent en résonance avec l'action ou la volonté du gouvernement que le gouvernement mène quotidiennement ou qui le mec qui le mènera dans les mois à venir au service de notre agriculture de nos agriculteurs et nous avec justice soit parce qu'enfin ils font écho avec l'ambition que nous portons avec l'APL. Alors, le sénateur du plomb disait n'ayez pas peur. Bon j'aime bien cette expression. Et la 2ème, chose que je voulais dire je je vous invite à effectivement ne pas avoir peur d'abord ne pas avoir peur. De parler de compétitivité agricole d'abord ensuite de ne pas avoir peur je sais que c'est révolutionnaire dans les temps que nous traversons de trouver des consensus. Vrai révolution me semble-t-il, c'est d'essayer de trouver des consensus que les 10 suce. C'est assez facile et en particulier sur le sujet agricole. Je vous invite à ne pas avoir peur de sortir des caricatures et des postures. Parce que je pense que nous en avons grand besoin que nous en avons besoin pour les agriculteurs de ne pas avoir peur non plus d'affronter les grands défis et de les dire aux agriculteurs en particulier les défis des transitions et les défis climatiques et puis de ne pas avoir peur de ce débat qui est pour moi très utile parce que je pense que nous en avons besoin pour l'agriculture et que nous le devons aux agriculteurs ou agricultrices et en cela, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, je tenais à vous remercier avant que nous entamions l'examen des articles. Nous passons à la dit. Question de la motion. Tendant à opposer la question préalable qui a été déposée. Par le groupe. Écologiste solidarité et territoires. Et. Pour la défense de cette motion. La parole est à Monsieur Daniel Salmon pour 10 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Le groupe écologiste, elle vous le savez viscéralement attachée au débat démocratique. Pourtant nous avons déposé aujourd'hui une question préalable pour rejeter ce texte. En effet, nous devons prendre conscience de la gravité de cette proposition de loi à la fois dans son calendrier de discussions et sur le fond des articles qu'elle propose, composée essentiellement de régression sociale et environnementale majeure. Tout d'abord sur la forme, la discussion de ce texte intervient alors qu'une concertation est en cours sur ces mêmes questions pour construire un projet de loi d'orientation et d'avenir agricole alors que les syndicats, les associations, les élus des territoires s'implique depuis des mois pour faire remonter des propositions alors que ces travaux sont en train de s'achever le Cesena estime avec la discussion de ce texte qu'il n'est ni utile ni pertinente patienter quelques semaines pour s'appuyer sur leur contribution. Dans un contexte où la démocratie est fragilisée, ou les sociétés, les citoyens et la société civile se sentent peu écouté et en décalage avec les instances politiques, il convient pour nous de réfléchir au message envoyé par notre assemblée si elle choisit de rejeter cette motion et du et de discuter ce texte. La concertation organisée sur la LOA est déjà pour nous largement insuffisante. La participation des citoyens a été organisée avec des mois de retard en toute discrétion et via un questionnaire accessible durant seulement 15 jours. Le manque de pluralisme des débats a également été dénoncé. Mais la qualité la crédibilité des dispositifs de participation semble apporter peu pour les auteurs de ce texte pour qui l'essentiel paraît être de verrouiller encore davantage le débat en organisant un 1er round avec le gouvernement pour faire valoir une vision bien particulière de l'agriculture. Certes le Sénat et les parlementaires ont toute légitimité pour faire des propositions dans le cadre des concertations sur l'orientation de notre agriculture. Mais les propositions portées par ce texte figurait déjà dans un rapport sénatorial qui semblait bien suffisant pour contribuer aux travaux en cours. Tout aussi problématique. Ce texte présenté comme étant à vocation agricole propose des modifications substantielles de notre droit du travail en organisant le cumul de revenus d'activité et le RSA. Ou l'orientation active des demandeurs d'emploi vers des secteurs en tension sans réflexion sur leur parcours ou sur les conditions de travail dans ces secteurs. Ces réformes structurantes sont proposés à la veille de discussions sur les lois travail là encore nous sommes dans un contretemps démocratique qui dénote un mépris du dialogue avec la société civile et les partenaires sociaux et ce dans un contexte extrêmement tendu. Par cette question préalable, nous proposons de respecter le temps de la démocratie et de la concertation. Notre modèle agricole et d'autre modèle social sont au coeur des questions majeures pour nos sociétés, nous pensons qu'elle mérite bien mieux que les quelques heures de débat qui nous sont proposés ce soir. Au delà même de ces questions de forme, le fond de cette proposition de loi nous apparaît particulièrement dangereux. Tout d'abord nous estimons que ce n'est pas le rôle du Parlement d'alimenter de fausses informations sur les supposées sur- transposition du droit français. Rappelons que si ne cesse à retirer l'autorisation du S-métolachlore. C'est en application directe d'un règlement européen ni plus ni moins. Rappelons aussi que ces conclusions je dois essayer de le le, ça qui fait état de préoccupation critique sur cet herbicide dont l'autorisation de mise sur le marché au niveau européen expire le 31 juillet 2023. Rappelons enfin qu'un rapport du gouvernement sur le sujet paru l'année dernière, estimait que les surtranspositions était particulièrement peu nombreuses et que quand elles existaient elle correspondait à un choix politique assumé. Doit-on inscrire dans notre droit un renoncement à faire de la France un pionnier en termes de progrès environnemental, social et sanitaire. Cela nous paraît aller contre le sens de l'histoire, alors que les sécheresses, les preuves sur les impacts des pesticides. La pollution de notre ressource en eau devrait nous pousser à accélérer la transition on voudrait par ce texte nous contraindre à la ralentir. Pire, on nous propose même de faire marche arrière de revenir sur les trop rares avancées de ces dernières années. Abandonner la séparation du conseil et la vente et de la vente des pesticides pour garantir aux agriculteurs un conseil indépendant Exit. La loi de 2014 qui favorise en renforçant le rôle de Lanxess l'indépendance de la décision sur les autorisations de pesticides. Pire encore, on nous propose même avec ce texte, de remettre en cause de droit européen de protection de l'environnement et de faire primer les intérêts économiques de court terme. Ainsi sur les pesticides. Vous proposez de contraindre les retraits de produits dangereux au regard d'une balance bénéfice-risque entre la santé et l'environnement. D'un côté et les distorsions de concurrence de l'autre. Cette proposition fait preuve d'un cynisme sans nom, à tel point que l'association phyto Victimes représentant les professionnels malade du fait des pesticides nous interpellait il y a quelques jours dans un communiqué de presse avec cette question, notre santé a-t-elle un prix. Mais en plus d'être cynique, cette mesure est une attaque en règle contre le droit européen. La CJUE vient tout juste de le rappeler le règlement sur l'autorisation des pesticides prévoit que l'objectif de protection de la santé humaine et de l'environnement en particulier devrait primer sur l'objectif de croissance des rendements. Reconnaissons que vous n'êtes pas les seuls à promouvoir ces attaques aussi dangereuse soit-elle. Nous avons tous en tête les déclarations qui regrette l'élimination de molécules comme si ces interdictions ne procédait pas d'étude scientifique prouvant leur dangerosité sur les ni ou ni sur les néonicotinoïdes la phosphine le glyphosate, il ne s'agit pas de créer de la norme pour la norme. Il s'agit de lutter contre une pollution généralisée et d'enrayer l'effondrement de la biodiversité. Nous voulons aussi poser une question, ce mot d'ordre de la compétitivité prix porté par les majorité sénatoriale gouvernemental bénéficient-ils réellement aux agriculteurs car c'est là un enjeu crucial de notre débat. En agitant le chiffon rouge de la surtransposition des cotisations sociales trop élevées, des normes environnementales trop contraignante. On oublie d'opposer dans le débat public. Les vrais sujets qui menacent notre agriculture ces sujets. Vous les connaissez tous, ce sont la promotion du libre-échange de la dérégulation des marchés européens d'une PAC inégalitaire et inefficace d'une répartition de la valeur équitable dans les négociations commerciales le sept a conclu en 2016 n'a toujours pas été soumis au vote du Sénat dans un déni de démocratie que nous n'oublions pas de même de nombreuses inquiétudes persistent sur l'impact de l'accord avec le Mercosur sur les marchés agricoles et nous le partageons c'est en agissant pour une sortie de l'agriculture du libre-échange pour la régulation des marchés au niveau européen pour une PAC juste qui accompagnent transition que nous garantirons un revenu décent à des agriculteurs nombreux. Nous voulons en effet construire une véritable compétitivité pour notre agriculture car la compétitivité prix placé au coeur de ce texte est extrêmement réductrice elle néglige tout un pan des coûts qui sont assumées in fine et par qui. Bah par la collectivité. Bien sûr que devient l'analyse de la compétitivité de notre agriculture. Si on y inclut les coûts cachés des pesticides, des nitrates et des engrais azotés, que devient l'analyse de notre balance commerciale. Si on y inclut les coûts de l'importation massive d'intrants et les subventions publiques visant une fine et à soutenir l'exportation de denrées alimentaires. Pour nous la compétitivité de notre agriculture inclut l'ensemble des dimensions à la fois économique, social, environnemental et sanitaire. Elle prend en compte les emplois générés. La qualité de l'alimentation l'avis des territoires, la réponse aux attentes des consommateurs. Oui il nous faut maintenir et développer une production locale diversifiée à même de nourrir notre population et d'exporter pour équilibrer notre balance commerciale. Oui, l'augmentation des importations est une véritable problématique. Mais la solution pour y parvenir n'est pas de se lancer dans une course au moins disant social et environnemental et elle réside dans l'accompagnement de la relocalisation de l'alimentation et dans la transition vers des pratiques agronomiques permettant de se passer d'intrants dont les coûts explosent de limiter la consommation d'eau et d'énergie. À l'heure où l'efficacité et la sobriété sont des nécessités. Ces solutions sont pourtant les grandes absentes de ce texte qui mise sur le renforcement de nos dépendances à la mécanisation à la radio à la robotique à l'irrigation massive aux pesticides. Le tout à grand renfort de dépenses publiques et d'exonérations de cotisations sociales. L'agro-écologie et notamment l'agriculture biologique fonctionnent déjà sur le terrain et permettent de cultiver l'autonomie la résilience et de produire des excédents. Certes, il nous faudra garantir l'accès à toutes et à tous à cette alimentation locale et de qualité. Nous ne pouvons oublier qu'un nombre croissant de nos concitoyens souffrent actuellement de précarité alimentaire mais pour nous, la réponse se situe dans une politique ambitieuse de justice sociale, pour l'accès à une alimentation de qualité. À l'heure où les inégalités explosent, cette ambition, plus que jamais nécessaire et systématiquement négligée par les politiques publiques. Nous devons agir collectivement pour construire une véritable sécurité sociale de l'alimentation, comme le soulignait notre collègue Mélanie Vogel dans son rapport sur la sécurité sociale, écologie. Chers collègues, nous vous proposons donc par le vote de cette motion de respecter le temps du débat démocratique, nous vous demandons de refuser un texte qui, en s'appuyant sur un diagnostic erroné en attaquant le droit européen et en propageant de fausses informations nous propose une série de régression sociale et environnementale qui ne seront bénéfiques ni pour nos concitoyens, ni pour nos agriculteurs. Merci, Je vais prendre la parole évidemment pour répondre à, à cette. Intervention alors permettez-moi de. De vous répondre. Chers collègues sur plusieurs points, d'abord la loi, la loi d'orientation, ainsi qu'un pacte sont bien à à l'étude environnement en ce moment, mais cela n'empêche en rien le Sénat de poursuivre ses travaux. Nous verrons le moment venu, ce que le gouvernement nous proposera comme avenir pour notre agriculture, Monsieur le Ministre, je crois sincèrement qu'il est de l'intérêt du Sénat d'affirmer dès maintenant sa position sur un nombre de sujets fondamentaux pour nos agriculteurs l'excès de norme. Nous en avons parlé, l'excès de taxes. Ou encore le défi du changement climatique. Je crois que nous n'avons pas été élu seulement pour attendent que le gouvernement nous transmettre des des projets de loi, mais bien pour faire entendre la voix du Sénat c'est. Que nous faisons ici cet après-midi dès lors nous sommes légitimes pour débattre d'une proposition de loi qui vous l'avez rappelé d'ailleurs chers collègues est le fruit d'un travail de longue haleine et par conséquent ce n'est pas un effet d'opportunités. Vous, vous citez dans vos dans votre, dans votre. Dans votre amendement. L'article 7 de la charte de l'environnement, qui dispose que toute personne a le droit de de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence. Sur l'environnement, c'est ce qui est fait dans le cadre des des discussions. Actuel mais cet article n'entend pas je crois déposséder le Parlement de ses prérogatives. Il me semble pas qu'il y ait d'antinomie ici. Ensuite vous expliquer de cette PPL remet en cause la protection de l'environnement et la santé. Est-ce que remettre en cause la protection de l'environnement que de protéger de de proposer dans cette PPL un diagnostic carbone des exploitations. Est-ce que remettre en cause l'environnement et la santé et de proposer une expérimentation l'utilisation des drone précisément pour diminuer les quantités de pesticides utilisés et protéger les applicateurs de leurs effets indésirables. Est-ce que remettre en cause la protection de l'environnement et de la santé, est-ce que c'est cela que de revenir sur des dispositions qui ne fonctionne tout simplement pas aujourd'hui, hé bien je ne le crois pas et si vous me permettez, je vais à mon tour citer la charte de l'environnement. Son article 6 énonce que les politiques publiques doivent concilier la protection de l'environnement et le développement économique. Il me semble que c'est exactement ce que nous faisons. Son article 9, dispose, quant à lui que la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation de l'environnement et c'est exactement ce que fait cette PPL enfin vous évoquez un peu la sincérité du débat. Je pense que le débat il est sincère. Nous jouons de part et d'autre, cartes sur table. Nous allons discuter des amendements. Le ministre s'exprimera. La Commission s'exprima les groupes politiques s'exprimera s'exprimeront et Assemblée votera. Il me semble donc il s'agit d'un débat sincère entre nous. Si madame la rapporteure. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la rapporteure mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur seulement. Alors d'abord je je je je je m'inquiète un peu parce que vous faites au travers de cette motion, le gardien vigilant de l'agenda gouvernemental. Défenseurs, que vous vous érigez du travail gouvernemental. Alors je le prends comme un, un moment de grâce au fond. Au Sénat, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça dure. Et d'ailleurs la suite de votre propos m'a prouvé que ça ne pouvait pas durer ainsi. Mais vous avez raison de saluer la concertation telle qu'elle a été menée pour faire en sorte que nous ayons à la fois avec les professionnels, avec les collectivités avec les responsables agricoles. Un dialogue qui me paraît fructueux. Deuxièmement, vous vous remettez en cause la là aussi c'est un peu paradoxal mais. On peut être à contre-emploi. Le fait que nous ayons ouvert un questionnaire je vous je vous indique juste qu'il y a eu 40.000 réponses. vous en trouverez beaucoup qui trouvent 40.000 réponses et donc finalement, je n'ai pas perdu. D'ailleurs c'était un dispositif de participation citoyenne. Le 10 j'ai été ministre des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Je n'ai jamais prétendu que c'était un exercice mais que j'avais besoin simplement dans un dialogue Direct au travers d'un questionnaire de sentir un certain nombre de choses sans prétendent que ça répondait aux académique. Ça n'empêche pas d'ailleurs que nous travaillons aussi avec les jeunes, sur cette question là et donc j'entends ça. Vous dites, vous avez 1000 fois raison lorsque vous dites que la définition de la politique agricole constitue une décision structurante pour notre société. C'est d'ailleurs là-dessus que nous travaillons pour autant est-ce que ça doit empêcher le Sénat de se saisir d'un certain nombre de sujets, je ne le crois pas, par définition, une loi d'orientation a vocation à embrasser un Champ plus large que celui de la compétitivité qui est plutôt le fil rouge de cette proposition de loi là où cette proposition évoque une urgence à cinq ça n'est pas incompatible avec la volonté que nous avons nous nous projeter à 30 ou 40 ans il me semble que c'est un élément important. Il y a une 2ème, chose que je voudrais dire parce que je peux pas résister à le dire, il y a pas d'un côté les défenseurs de l'environnement et la santé et de l'autre les défenseurs de je ne sais quel intérêt. Nous sommes tous défenseurs. Il y a ici sur tous ces bancs. Pardon Monsieur, et y compris le ministre de l'Agriculture, des gens qui pensent aussi l'intérêt général. Ils ont eux aussi. Des familles, des amis. Dominique. Des prérogatives et des inquiétudes sur l'environnement et ne ne ne nous drapeau pas dans la toge des uns contre les autres. Je trouve que c'est au moins à la fois caricatural et assez désagréable dans ce genre de débat. Nous si nous défendons et l'agriculture. Et la nécessité des transitions en tout cas c'est ce que j'essaie de faire et ce que je crois que je vous essayer tous de faire, il me semble que c'est un élément important et donc je voulais simplement dire, je rejoins ce qu'a dit la présidente. Et je je serai pas trop long. Alors après, on est toujours pris en contradiction de soi-même. Alors je vais vous donner un exemple. Vous avez été de ceux qui ont demandé de remettre en cause la ville sur la grippe aviaire. En disant ça n'est pas normal vous demander des mesures de confinement qui sont beaucoup trop lourdes alors que c'est la demande de Lanxess. Je vous demande. dans une logique économique, d'ailleurs c'est comme ça que vous me là nous vous nous l'avez dit, avec un certain nombre de gens que vous défendez de syndicats que vous défendez. Il faut sortir du confinement pour les élevages dit autarcique. Alors ça, ça vous pose pas de problème. Ça, ça n'est pas une question et c'est normal que vous posiez cette question là sur l'élevage. Grippe aviaire et les difficultés que ça peut produire, d'un point de vue économique mais quand s'est posée de ce côté-là ou par vous, il y a pas de difficulté. Mais moi je pense que c'est la même sujet pose. Personne ne remet en cause les prérogatives de lancer il spicy pas plus qu'ailleurs, mais tout le monde peut se dire, sur certains sujets que l'équilibre comme l'a très bien dit, la présidente est un équilibre entre l'économique et les contingences et les nécessités environnementales et de santé publique et c'est ce que vous nous avez demandé par exemple sur la grippe aviaire 2ème élément je voudrais vous dire, la phosphine. Pardon, la phosphine, c'est un sujet que je connais bien pour avoir débattu publiquement du sujet, on est quand même dans une situation, pardon, il y a des gens de l'autre côté de la Méditerranée qui attendent nos céréales pour se nourrir. C'est pas des petits sujets c'est seulement. Donc il suffit pas de claquer des doigts et de dire on interdit et peu importe ce qui arrive à ces populations qui sont soumises à une contrainte de sécurité alimentaire et qui demandent ces produits-là et que demandent ces produits-là, avec ces traitements nous, nous ne pratiquons pas, mais qui le demande. Donc je trouve que donner la leçon, c'est un peu un peu risqué, donc on s'sent croise les doigts et on regarde les gens banquier d'alimentation. C'est ce que vous proposez en tout cas c'est pas moi ce que je proposerais jamais parce que je pense que la sécurité alimentaire est un problème largement devant nous 3ème élément. Ah peut-être je je vais mettre à dos l'ensemble du Sénat les accords de libre-échange pardon la la question de la compétition ferme France. D'abord il y a 25 ans on se féliciter que sur tous les registres, nous exportons donc faut pas avoir peur de l'exportation. La question c'est d'être compétitif 2ème élément pardon la compétition, elle se nouent pas avec les pays à l'extérieur du vous parlez des de de d'accord qui n'existe même pas encore parler de Mirko sur la perte de compétitivité française elle a 25 ou 30 ans. Donc c'est une perte de compétitivité avec nos voisins européens. Sur les fruits et légumes c'est avec nos voisins européens, sur la viande bovine, c'est avec nos voisins européens. Et donc, n'allons pas chercher des boucs émissaires. À l'extérieur et des accords de libre-échange qui serait la cause de tous nos maux. Parce que ça sont décrit pas la réalité, on ne décrit pas la réalité y compris vis-à-vis des agriculteurs. Il me semble que c'est un élément important, enfin 2 éléments complémentaires. Je je je je pense pas vous apprendre grand-chose mais je crois que le bio aussi aura besoin d'eau. Et donc caricaturer les agricultures en pensant que y compris cette année en 2022, il y a pas des gens en maraîchage qui ont manqué d'eau en bio, c'est faire une erreur, donc on aura besoin d'eau. Ne caricaturons pas l'accès à l'eau et le besoin nous comme un nu les caricatures d'une agriculture que que nous avons envie de voir évoluer le maraîcher a besoin d'eau et donc on a besoin de se poser tranquillement la question d'eau et 2ème élément l'interdiction produit pas la solution. Pardon, je vous le dis parce que je l'ai vécu aussi. De façon un peu compliqué quand vous êtes ministre il n'aimait pas avoir affronté ces situations-là les néonicotinoïdes. J'ai entendu des gens y compris de vos amis politiques ont dit à longueur de plateaux, on a la solution et les alternatives sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Résultat des courses. J'espère que l'épisode de jaunisse ne viendra pas mettre à mal totalement la filière betterave donc à vrai dire c'est pas parce que vous dites et qu'on ânonne qui a des solutions que il y a des solutions et c'est pas parce qu'on dit qu'on fait une interdiction qui a des solutions donc on a besoin de se mettent dans la transition on a besoin de se mettre dans la transition parce que le jour où on a plus de betteraves. Le jour où on a plus de sucre en France, on ira chercher où vous savez on ira le chercher dans l'accord du Mercosur que vous défendez que vous sur lequel vous tapez temps et donc ça c'est pas très cohérent et donc je pense qu'on a besoin, collectivement, de cohérence, merci. Merci monsieur le ministre alors en explications de vote. Je rappelle qu'il y a possibilité d'une explication de vote par groupe. Pour une durée n'excédant pas 2 minutes Monsieur Tissot. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La soirée va être long. Monsieur le ministre, je vous trouve bien. Moi non non je je suis pas pressée de moi non plus mais je vous trouve bien vif après seulement 10 minutes de débat. et les rôles sont établis et le et le débat va être intéressant donc encore en cohérence avec le propos. En cohérence avec le propos que j'ai tenu en commission en cohérence avec le propos que je vais tenir tout à l'heure. Dans le cas de la discussion générale, nous voterons cette question préalable. C'est ça le débat. Nous la voterons quand nous partageons pleinement les remarques développée par notre collègue Daniel Salmon, cette proposition de loi qui réécrit allègrement notre politique agricole ne respectent pas à notre sens la concertation effectué par la loi d'orientation agricole, de nombreuses mesures de ce texte entraîneront des conséquences importantes, que ce soit sur les pratiques agricoles. Le droit du travail ou l'environnement. a minima mérité une concertation plus large et une association des autres commissions sénatoriales. Je pense notamment à la commission des affaires sociales à la commission des finances. Et puis,

à notre avis autant dans sa forme que sur le fond et c'est pour cela. Cette question préalable nous paraît pleinement justifiée nous la soutiendrons donc je vous remercie. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste solidarité et territoires sur cette motion. Je vous rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en commission. Donc il va être poursuivi au scrutin public dans les conditions fixées par Dick 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Nombre de votants, 343. Suffrages exprimés, 338 pour 86 contre 252, le Sénat n'a pas adopté cette motion.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, rapporteur. Mes chers collègues je ne dis rien ici a lieu et place dans mon collègue Henri Cabanel.

Notre modèle agricole arrive à bout de souffle c'est constat aussi c'est que préoccupante nous pousser à rechercher et explorer les solutions les plus à même d'inverser la courbe sommes crimes quelles que soient nos commissions. Nous devons penser à l'agriculture de demain. Autrement qu'à travers le prisme de la critique stérile. Réfléchi aux enjeux d'orientation de transmission d'installation de moins organisations et de dynamisation de la ferme France. Marquée par un contexte inflationniste de transition écologique et climatique, bousculant les pratiques agricoles actuelles mais aussi celle des consommateurs. Rappelons que la France aujourd'hui 5ème exportateur mondial été sur la 2ème marche du podium jusqu'en 2006. Son acquérir un commercial un retrait n'est plus tiré que par l'effet prix de ses exportations vins et spiritueux tête énorme par les volumes du grenier de l'Europe, nous sommes aujourd'hui tout au plus réduits à à naître la cave. Si nos politiques publiques. Si sommes démarqué par la défense de modèle conciliant performance économique et écologique. Elles se sont traduites par la production de produits haut de gamme peu rémunératrice pour les agriculteurs à destination d'une clientèle de niche à fort pouvoir d'achat. Quant aux consommateurs le plus modestes. Ils ont été contraints de se tourner vers 10 réimporter. Produites dans des conditions environnementales et sociales non satisfaisante ou peu transparente. Je rappelle que lorsqu'un franc c'était pas 100 euros ah dans l'alimentation seulement six euros 90. La Poste du producteur. Le partage de la valeur devrait essentiel et dicter nos actions dans les relations commerciales entre le monde agricole. L'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Or, si le 10 dernières années nous avons emprunté le chemin inverse et détruit cette valeur sous couvert de prix le plus bas à ce jeu là. Je rappelle que ce ne sont ni les producteurs ni les consommateurs qui en ressortent gagnants mais les intermédiaires. Alors que vous en nous face au défi du renouvellement des générations. Notre modèle agricole matière n'attire plus les jeunes et nous exploitants. Si nous continuons à ne pas rémunérer les professionnels du secteur à leur juste valeur. D'étouffer les notions et nous enfermer dans le carcan de l'soumis notamment à de multiples surtransposition. Néanmoins, il est fondamental que nous avancions selon un triptyque est indissociable. Ou, économie, santé et environnement ne doivent pas être qui fié au profit l'un de l'autre. Si la compétitivité de la ferme France. Est aujourd'hui handicapé par les normes élevées en matière environnementale sanitaire notamment. Il ne faut pas au nom d'une productivité productivité renouvelé avant d'abandonner le gars qui, qui font du modèle agricole français le plusieurs du monde pour autant toutes les questions d'équilibre à ce égard. Soyons attentifs aux accords de libre-échange. Fragilisant notre agriculture. Je rappelle que le groupe RDSE à présenter au Sénat une proposition de résolution dénonçant l'accord de libre échange avait Marco sur qui compter les germes d'une déstabilisation du marché européen de viande bovine et par ricochet une fragilisation des territoires ruraux attendant aujourd'hui encore le droit de trouver des rustines car la grande loi d'orientation agricole n'est pas au rendez-vous encore Monsieur le Ministre. Le texte aujourd'hui. A le mérite d'enrichir le débat sur le Champ de compétitivité en faveur de la ferme France. Le groupe RDSE souhaiterait améliorer certaines dispositions qu'qui prévoit, nous aimerions notamment que la proposition de loi contiennent des mesures traitant transition globale systématique les exploitations agricoles ou l'atténuation et adaptation aux sérieux mathématiques seront le fil conducteur des nouvelles des marchés agricoles

Deuxièmement. La réalisation d'un diagnostic de réduction de l'impôt carbone et des performances agronomiques des sols incluant des réductions d'émissions de gaz de serre. Tels que définis dans le cadre du Label bas-carbone. Troisièmement, nous désirons que les paiements pour services environnementaux se démocratise aux scènes exploitations agricoles afin de faire de la restauration et du maintien des écosystèmes une source vu en termes de revenus et non pas une contrainte qui peut.

Dans cette perspective, le groupe sera attentif à l'examen de chacun des articles du texte avec un préavis globalement favorable à cette proposition de loi. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion. La parole est à Monsieur Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

Monsieur le Ministre. Madame la rapporteur chers collègues cher président. Je voudrais bien sûr salué en premier. Laurent Duplomb Pierre et cher vieux. Parce que tous les trois vous nous permettez effectivement. D'apporter notre Pierre. À cette discussion. Tellement ambitieuse monsieur Ministre une loi d'orientation. Quand on sait qu'aujourd'hui l'agriculture française globalement fonctionne encore sur les fondements de ces lois de rédaction de 60 62. Et mon propos n'est pas de dire qu'. Se. Cette loi n'est n'est plus d'actualité. Mon propos est de dire il y a effectivement un monde a changé, il y a des attentes nouvelles. Il est essentiel. D'y apporter une contribution. Et cette proposition de loi et participe. Et je voudrais remercier notre rapporteur effectivement de son travail qui vient compléter le travail des 3 dépositaire et des autres cosignataires. Et je voudrais prendre quelques exemples très concrets. Je commencerais déjà par l'article de. L'article 2 qui tout simplement dit. On va donner des perspectives. Tous les 5 ans. C'est ce dont souffrent la France depuis tant d'années à avoir une feuille de route. Avoir des perspectives. Et effectivement, filière par filière, c'est d'inscrire et je partage. Monsieur le Ministre votre propos une loi d'orientation, c'est plus lointain mais elle nécessite des rendez-vous. Cette notion de rendez vous tous les cinq ans sur la compétitivité sur le positionnement de la ferme France est essentielle. L'autre exemple que je voudrais prendre, c'est l'article 4. Je le dis d'autant plus que j'avais été rapporteur sur la loi. 2015 de Jean-Claude Lenoir. Nous avions déjà en 2015 ici dans le Sénat évoqué effectivement ce livret d'épargne. Populaire. L'agriculture c'est pas que l'affaire des paysans et dans ce projet de cet article 4. On va tenter on propose tout simplement de réussir ce qu'on est en train de réussir au niveau de la forêt, puisqu'aujourd'hui il y a des reboisements qui se font ou ce sont des particuliers qui mettent des moyens conjointement je dirais oui aux collectivités à l'État. Eh bien là c'est la même chose c'est faire participer les Françaises et les Français au choix stratégiques de leur alimentation et je trouve que là aussi c'est quelque chose de très. Important Rendre les Françaises et les Français acteurs de la politique agroalimentaire de notre pays. L'article 6, là aussi en titre d'exemple. Parce que là on a un rendez-vous Monsieur le Ministre. On a réformé il y a peu de temps le principe des calamités agricoles. On est parti sur l'assurantiel. Et l'assurantiel. C'est une part importante, plus importante que par le passé sur la contribution des agriculteurs à la gestion du risque. Et là, il est absolument essentiel si on veut réussir le dossier des calamités agricoles. Si on veut réussir ces aléas qui font qu'effectivement les agriculteurs en agriculture, les années ne se suivent pas. Et il est là, absolument. Stratégique là encore de modifier le plafond sur la dotation pour l'épargne de précaution. C'est une nécessité si on veut réussir. Ce que vous avez lancé ce qu'on a là aussi le Sénat il y a contribué. Sur la réforme de la gestion des risques. Et l'article 10. Ah et ça il me fait vraiment plaisir parce qu'on l'avait déjà évoqué en 2015. Et je voudrais là encore. L'information du consommateur. Monsieur le Ministre vous interdisez je sais pas vous mais la France interdit aux paysans français de faire des cultures OGM. L'Europe interdit de faire des cultures OGM et tous les jours des consommateurs français et européens mangent des OGM. C'est là qu'il y ait nécessité effectivement d'avoir l'honnêteté, la transparence sur l'étiquetage et d'information du consommateur. L'article dit cela aussi repositionne notre responsabilité par rapport à la production et à la consommation. L'autre point et j'avais évoqué en. Commission. L'article 19 et 20. Je suis choqué par les propos de notre collègue tout à l'heure. Parce que au contraire l'agriculture peut être une forme de solutions pour celles et ceux qui sont au bord du marché de l'emploi. Nous, nous en avons besoin. Ils peuvent retrouver des perspectives, il peut retrouver quelque part l'étincelle dans le coeur qui leur donne envie de se relancer dans la vie professionnelle. Nous savons aujourd'hui que les fils et les filles d'agriculteurs ne sont pas en capacité aujourd'hui de reprendre l'ensemble des fermes qui se libère. Nous avons plus que jamais besoin d'ouvrir le monde agricole, plus que jamais si nous voulons réussir notre indépendance élémentaire. Nous avons besoin de permettre à des femmes et des hommes de se lancer dans l'agriculture soit dans le salariat et pourquoi pas mais demain, Monsieur le Ministre, je l'avais porté lorsque j'étais aux jeunes agriculteurs sur la transmission et l'installation des jeunes. Voilà, c'est toutes ces raisons qui font que le groupe Les Républicains soutient effectivement ce texte et votera pour ce texte, nous avons besoin de cap. Nous avons besoin de donner envie, nous serons bien sûr avec un avis favorable.

Merci monsieur le président. Monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Comme l'a dit l'ancienne présidente de la FNSEA, Christiane Lambert lors du dernier Salon de l'agriculture. Notre agriculture Davis. En En effet, notre balance commerciale ne cesse de se dégrader depuis 10 ans. Nous sommes aujourd'hui un des seuls grands pays agricoles à voir ses parts de marché reculé depuis 2000. Nos capacités productives s'effrite. Certaines filières s'affaiblissent dangereusement. Notre solde commercial a chuté, passant de 12 milliards en 2011 à 8 milliards en 2021. En matière d'exportation. Nous sommes passés en 20 ans du 2ème rang à la 5ème place. Nos importations explosent, et nous importons de 2 fois plus qu'en 2000. Près de 50% de ne, de ce que nous consommons aujourd'hui est issu des importations et principalement intra- européenne. La compétitivité de notre agriculture décline dangereusement. Il est urgent de réagir et c'est toute l'ambition de ce texte que nous soutenons pleinement. Il propose de réduire les contraintes qui pèsent sur notre agriculture et sur nos agriculteurs d'encourager l'innovation et d'accompagner les transitions. En effet depuis 20 ans nous avons privilégié les injonctions en matière sociétale et environnementale sans intégrer également la dit la dimension de la compétitivité et de la performance. C'est une erreur de vouloir opposer investissements Innovation Santé publique et performance, il faut au contraire et ses objectifs. Cette proposition de loi et dense et techniques et je je veux d'ailleurs et tout d'abord saluer donc le travail des trois auteurs. Et de notre rapporteur chers Sophie Primas, qui a su enrichir et compléter ce texte. Je voudrais maintenant m'attarder sur plusieurs mécanismes de ce texte sous l'article 13, complète l'émission de Lanxess. Elle sera chargée d'établir dans ses avis une balance des bénéfices et des risques. Or dans les faits, il s'avère qu'elle n'a à ce stade ni les moyens ni les compétences d'exercer cette mission et c'est pour cela que derrière Madame la rapporteure. Nous avons j'ai également déposé le même amendement en commission un amendement qui a été adoptée, qui tend à octroyer au ministre de l'Agriculture. Un droit de véto. Cette mesure permet de suspendre la décision de lancer, si la souveraineté alimentaire est en péril et si aucune solution alternative n'est possible. Nous devons la tirer les leçons de nos erreurs et éviter les précédents qui ont lourdement fragile fragilisés des filières toute entière. L'article 9 est un axe majeur de ce texte le stockage du carbone est un enjeu essentiel. L'agriculture que nous devons bâtir doit être porteuse de solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et le stockage du carbone en état. L'article 12 prévoit quant à lui de lutter contres les sur-transpositions des normes. Européennes en fixant un principe de non surtransposition et charge le Conseil d'État dans ses avis de les identifier ces sur-transposition sont souvent source de distorsion de concurrence et fragilise nos filières tout cela contribue également à réduire l'attrait du métier, à exaspérer nos agriculteurs qui coule croule sous les injonctions contradictoires sous des directives mal comprises et souvent déconnectés des réalités quotidiennes de leur métier, il faut absolument redonner du sens. Enfin, l'investissement est cruciale et à ce titre de dispositions sont proposés. D'une part le crédit d'impôt et d'autre part le livret A gris. En matière d'investissements. Toujours il est impératif de soutenir aussi les investissements dans l'otite dans les outils de transformation et dans l'agroalimentaire pour restaurer notre force exportatrice et maintenir notre puissance agricole. Nous devons impérativement allier performance innovation durabilité des produits aucun de ces objectifs n'est à sacrifier. Il faut au contraire les combinés. Ça doit être ça. L'agriculture d'aujourd'hui et de demain. La productivité n'est pas incompatible avec les objectifs environnementaux faute de temps, je ne pourrais pas m'attarder sur la séparation du Conseil des. La vente sur le. Sur laquelle le texte revient. C'est une mesure que j'ai toujours jugé. Contreproductif source de complexité de désorganisation. Il est préférable à mon sens, de renforcer l'exigence et la qualité du conseil pour nos agriculteurs pour conclure Monsieur le Ministre. Je formule le voeu que ce travail transpartisan qui vient à point nommé se un élément constitutif de votre future loi d'orientation et d'avenir de de l'agriculture dont nous soutenons l'initiative. n'ayons pas peur comme l'a dit Laurent Duplomb. Merci. Une délégation de l'Assemblée de la République portugaise. Conduite par son président Monsieur Augusto Santos Silva. Est composé de membres du groupe d'amitié Portugal France présidée par Madame Emilia Cerqueira. La délégation qui vient de s'entretenir avec le président du Sénat est accompagné par notre collègue Louis-Jean de Nicolaï. Président du groupe d'amitié France-Portugal. Du Sénat. La mission de nos homologues portugais porte en particulier sur nos relations économiques, culturels et scientifiques. Elle fait suite à l'accueil à Lisbonne la semaine dernière d'une délégation du groupe d'amitié France-Portugal. La France et le Portugal qui entretiennent des relations historiques étroites et danse se sont encore rapprochés au sein de l'Union européenne. Quelques mois après la clôture de la saison culturelle portugaise en France et un an avant la commémoration du cinquantenaire de la révolution des oeillets, qui a rétabli la démocratie au Portugal. Nous espérons que votre visite ait pu contribuer à consolider encore nos liens parlementaire. en votre nom à tous chers collègues permettez-moi d'adresser un salut solennel et amical à la délégation conduite par le président de l'assemblée de la République du Portugal.

Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Joël Labbé. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, rapporteur, chers collègues. Nous voici donc quelques mois avant les débats de la loi d'orientation agricole à discuter d'une pré- loi d'orientation selon la. Selon une version de la majorité sénatoriale. Car c'est bien de cela qu'il s'agisse ce texte propose des orientations claires pour notre agriculture, mais nous ne pensons pas que ces. Stations de près freineront la chute du nombre de paysans. L'endettement des agriculteurs. L'effondrement de la biodiversité, la pollution de l'eau et l'épuisement des sols. C'est pour nous une fuite, une fuite en avant, je voudrais insister ici sur quelques reculs majeurs contenues dans ce texte. L'article premier propose de subordonner l'ensemble des politiques publiques agricole à la compétitivité Sacrifiant de fait les enjeux sociaux, environnementaux et sanitaires. À l'article 8, on autorise largement l'épandage de pesticides par drone sans prendre en compte les risques de dérives. Pointées par. Nous dénonçons les reculs sur les trop rares avancées de la loi Egalim. Nous, nous voterons contre l'article 11 qui revient en arrière sur la qualité alimentaire en restauration collective.

de durable et de local, c'est la loi. On est loin du compte et on se doit en se devrait dans ce type de texte mais on se devra dans le dans le dans le cadre de la loi. J'allais dire d'avenir agricole, elle doit être d'avenir agricole également. Introduire cela avec force ce qui suppose de donner des moyens aux territoires. Nous sommes aussi particulièrement atterré par l'article 12 qui vise à subordonner la possibilité d'avancer sur la protection de l'environnement et de la santé à l'absence de distorsion de concurrence européenne. Nous dénonçons l'article 13 qui soumet les retraits de pesticides jugés dangereux à une balance bénéfice-risque axée sur l'économie et remettre en cause le rôle et l'indépendance de l'Inde Obtenus depuis 2014. Encore une fois, il s'agit d'acter non 106.000 cynisme la supériorité des intérêts économiques de court terme et de compliqué voire entraver tout progrès dans la protection de nos concitoyens et de l'environnement. les mesures sur l'eau sont tout aussi problématique, notamment l'article 15 qui promeut le stockage et l'irrigation, sans aucune réflexion sur son encadrement. À l'heure du réchauffement climatique. Nous avons aussi à redire sur le volet social que l'on considère nous antisociale les cotisations ne sont rappelons-le pas des charges mais des outils de protection sociale.

Oui comme vous alors allons-y. Le rapport de l'INSERM de de 2014 il m'avait frappé sur sur l'impact des pesticides sur la santé humaine. Qu'est-ce qui en est sorti, on a reconnu la maladie de Parkinson et le cancer de la prostate comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. La Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes sur l'agriculture biologique qui considère que la la l'agriculture biologique et très insuffisamment et des et enfin le dernier rapport de l'INRA agriculture européenne sans pesticide qui montre que des politiques cohérente et articulée permettrait de sortir de ces molécules chimiques. L'actualité de ce matin. Qui s'y invite un article dans le monde et qui n'est pas inventé la chute des populations d'oiseaux, 60% en 40 ans sur le sur le continent européen, c'est dire s'il y a vraiment des soucis. Alors c'est très probablement je je suis prudent ma dernière intervention en discussion générale hein je, je dois vous exprimer mon dépit mes regrets par rapport à tous ces sujets. Monsieur le Ministre, vous avez dit tout à l'heure oui mais l'agriculture biologique utilise aussi de l'eau mais encore heureux, Monsieur le Ministre. Après c'est une question de quantité. L'agriculture biologique n'est pas industriel. Et je tiens à le à le mettre en avant et je tiens à la défendre comme une véritable agriculture d'avenir et dans ce texte il y a pas un mot. Pas une pensée sur l'agriculture biologique. Pas une et on va dire ouais arrêter d'opposer les les les agriculteurs procureur ça heureusement qu'il y a encore des gens qui qui la défendent. Pour la défendre. Absolument. Si cher collègue. Merci. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à madame Patricia Schillinger pour le groupe RDPI pour six minutes. monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est largement issu les recommandations du rapport de la mission d'information sur la compétitivité de la ferme France. Les discussions que nous avons pu avoir autour des conclusions de ce rapport nous ont permis de cheminées et de convenir, en commission, qu'il ne s'agissait ni d'opposer des modèles les uns aux autres ni de condamner en bloc la stratégie de montée en gamme si la compétitivité de notre modèle agricole ne peut s'opposer uniquement sur le haut de gamme ne miser que sur les volumes sans tenir compte des externalités négatives que cela implique serait passé notre agriculture, à côté des grands enjeux qui s'imposent non seulement à elle mais aussi à toutes celles de la planète. En plus d'assurer la souveraineté alimentaire et doit répondre à une exigence croissante de qualité et s'orienter vers les pratiques plus durable, respectueuse de l'environnement et du climat. Face à la concurrence internationale croissante de nombreux producteurs français ont ainsi fait le choix de bio ou d'inactivité ce signe de qualité synonyme de valeur ajoutée de prix de plus plus rémunérateur et de conquête de nouveaux marchés, la France fait ainsi en Europe figure de leader en matière bio lorsque nous réussissons soyons-en fiers persévérant et maximise notre Avantage comparatif les évolutions des pratiques et exigences sociétales sont partagées par des jeunes agriculteurs installés ou en devenir qui souhaitent être acteurs de la transition. Leur réussite sera notre réussite car d'ici 10 ans un tiers des agriculteurs sera en âge de partir à la retraite, le renouvellement des générations et donc une priorité. C'est même le principal défi de notre agriculture. Car sans agriculteurs il n'y aura pas de ferme France le dérèglement climatique et les évolutions démographiques nous impose d'évoluer en profondeur de nous adapter et d'anticiper, c'est pourquoi depuis 6 ans. Nous sommes aux côtés du gouvernement pour que les transitions nécessaires s'engage rapidement de manière pragmatique et efficace, les concertations nationales et locales pour le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricole préfigure un débat riche pour notre agriculture, et une loi structurante pour son avenir. Aujourd'hui, c'est de la compétitivité de notre agriculture dont nous à nous débattons lutter contre la concurrence déloyale rééquilibrer la fiscalité agricole favoriser l'innovation et les investissements nous y souscrivons cependant en examinant le texte nous notons que si nous partageons ces objectifs, nous avons des réserves sur certaines mesures qui parfois semble en contradiction avec. L'esprit affiché ainsi alors que la bureaucratie et la surabondance de normes sont les freins de la compétitivité. L'agriculture, la mise en place d'un haut commissaire à la compétitivité et d'un plan quinquennal de compétitivité peuvent étonner. Il faut toutefois reconnaître et saluer la qualité du travail fourni par Madame la rapporteure dont certaines modifications apportées au texte en commission constituent des. Des évolutions positives. Je tiens à insister sur celles apportées à l'article 8 l'expérimentation de la pulvérisation par aéronefs téléguidés tout en tenant compte des observations de Lanxess. Elle lève les freins à l'innovation à l'innovation qui a entravé le développement de toutes filières. Le recours à des drone permettra en effet de réduire significativement l'utilisation de produits de produits phytosanitaires. Le groupe RDPI a cependant déposé pour la séance deux amendements de suppression portant les mesures qui seront sans aucun doute rediscuté au cours de la de l'examen de la loi d'orientation s'il s'agit d'abord. De l'Arctique et il s'agit d'abord de l'article 15 et de la déclaration d'intérêt général majeur des ouvrages visant à prélever et stocker l'eau à des fins agricoles. L'article 18 ensuite qui abroge 2 avancée significative de la loi Egalim. La séparation de la vente et du conseil l'interdiction des remises rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques l'article 15 touche en effet à un sujet sensible qui fait débat dans l'ensemble de la société. La solution préconisée en en plus de susciter des crispations affaiblirait la concertation locale de l'article 16. Proposent pourtant de renforcer au sein des PDG. Le revirement opéré par l'article 18, quant à lui nécessiterait que l'on prenne le temps d'en évaluer l'impact en en terme de recours aux produits phytopharmaceutiques. Enfin, les mesures de maîtrise de charges sociales et de charges de production, si elle ne paraissent pertinentes semble davantage relever de l'examen du projet de loi travail et de finances que nous examinerons cet été Mes chers collègues, le chemin parcouru depuis la parution du rapport semble préfigurer de potentiels consensus sur le projet de loi d'orientation agricole. C'est important de le souligner sans masquer les désaccords qui subsistent pour ces raisons et sous réserve des débats que nous aurons sur ce texte. Le groupe Air dépérit RDPI aura la liberté de vote. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour 9 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous y voilà. Alors que les concertations sur la loi d'orientation agricole viennent à peine de se conclure. La majorité sénatoriale nous propose avec ce texte un 1er round pour définir une autre politique agricole. Nous commençons maintenant à nous habituer à ce jeu politique entre la droite sénatoriale et le gouvernement ou les propositions de loi sénatoriale. Certes à influencer les futurs projets de loi avec un terrain d'entente. Toujours plus à droite toujours plus libérale. Nous aurions pu espérer que l'agriculture qui est au coeur de l'histoire de notre pays puisse échapper à ces nouveaux calculs politiques et à cette volonté incontrôlée de tout vouloir déréglementer de tout vouloir déconstruire dans des logiques purement économiques. La proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui s'inscrit pourtant dans cette trajectoire, vous l'aurez compris par cette courte hein. Introduction, mes chers collègues. Mon groupe s'opposera avec vigueur à la très grande majorité des dispositions de ce texte, avant de revenir de manière plus détaillée sur les principaux aspects qui justifient notre opposition, je souhaite aborder le débat idéologique. qui justifient notre opposition peut être même philosophique sous-entendu par le rapport qui a initié ce texte, il s'agit de la fameuse opposition entre les modèles agricoles chers collègue Laurent Duplomb. Nous ne pouvons pas nier qu'il existe entre cette promotion doit le prouve une nouvelle fois. De vision de l'agriculture avec leur spécificité et leur valeur si 2 visions différentes toutefois, mes chers collègues. Et je pense pouvoir dire par mon expérience par mon métier d'agriculteur. L'opposition entre ces 2 visions ne peut pas se résumer à un simple adage un bon modèle celui de la raison qui servirait à nourrir les hommes face à un modèle de l'utopie des écologistes qui n'aurait l'objet que de bobos en tous genres de, des croissants et nos chers collègues les 2 modèles ont cette même vocation nourrir les hommes, les 2 modèles peuvent être s'ils sont adaptés à leur territoire compétitif et pérenne. Mais la principale différence entre ces 2 visions et que le modèle de l'agroécologie que et de l'agriculture biologique a élargi son approche en essayant de trouver un système qui soit autant respectueux du producteur que de l'environnement et je pense très sincèrement, Monsieur le Ministre, que c'est le rôle des pouvoirs publics et des législateurs d'apporter un soutien de long terme à un modèle qui tente d'allier santé humaine et préservation de l'environnement. Pour revenir sur la question de la compétitivité France Stratégie une institution autonome auprès de la Première ministre a présenté en 2020 une étude sur la rentabilité des exploitations agricoles en fonction de leur modèle. Après de nombreuses études de terrain, les 2 auteurs de ce rapport en sont venus à la conclusion suivante, je cite, les exploitations agricoles, agro-écologique présente en général des résultats économiques à moyen terme supérieurs à ceux d'exploitation conventionnelle. Mes chers collègues. Il nous sommes donc totalement aberrant de considérer que l'agriculture française souffrirait actuellement des shows engagés lors de l'ouverture à ce nouveau modèle en 2014 pour revenir sur les divergences de fond. Je souhaiterais commencer pour aborder l'ensemble des articles fiscaux de cette proposition de loi en effet pour les auteurs du texte. La question de la compétitivité semble se résumer à 2 termes crédit d'impôt et exonérations au sein de mon groupe nous les défendons à chaque PLS. Nous croyons à un impôt juste et redistributeur qui vient affecter uniquement les personnes qui peuvent en payer. Toutefois, nous n'avons pas de difficulté à aborder la potentielle question du trop d'impôts lorsque cela peut mettre en difficulté des concitoyens ou des entreprises mais il me semble quand même qu'il y a un problème dans vos dispositions fiscales, elle ne semble construite. Que pour les plus favorisés qui réalise déjà des bénéfices conséquents et elles n'aideront aucunement les agriculteurs en difficulté sans trop se tromper. Je pense qu'on peut dire que proposer une augmentation du plafond pluriannuel de la déduction pour l'épargne de précaution pour le fixer à 200.000 euros avec une déduction maximale par exercice amené à près de 60.000 euros. C'est surtout proposer une disposition pour les exploitants agricoles qui ont la chance de faire des bénéfices et de pouvoir des sommes importantes de côté. on peut ajouter le crédit d'impôt pour la mécanisation de l'article 5 que la rapporteur, madame la rapporteur vous avez plafonné à 20.000 euros. Un amendement qui descend en Corse plafond la création d'une déduction que vous avez donné un avis défavorable, c'est dommage quoi. Réaction d'une déduction fiscale pour favoriser la contractualisation à l'article 7 ou encore l'augmentation des seuils d'exonération de l'impôt sur le revenu. Prévue à l'article alors que nous devrions réfléchir à des aides pour aider les agriculteurs les plus en difficulté. Cette volonté de contourner l'impôt pour les plus favorisés est inquiétante pour notre pacte républicain. Dans un second temps. Je souhaite faire part de mon profond. Étonnement sur la teneur de l'ensemble des articles qui réécrivent allègrement le droit du travail, alors que ce texte est centré sur la question agricole. Ses auteurs ont fait le choix d'instaurer la notion de secteurs prioritaires. En tension dans l'émission de Pôle emploi ou encore de créer une exonération inédite au sein du dispositif dit de bonus malus sur les contrats courts et Monsieur le Ministre. Il serait peut être pertinent. C'était, c'était un truc que je vous propose. Que votre collègue Olivier Dussopt, ministre du Travail Vienne vous accompagner sur le banc pour présenter la position du gouvernement sur l'ensemble de ces points d'autant plus que ces mesures proposées sont moins des trains Nîmes. Anodine pardon et mériterait a minima une étude d'impact et sur ce large sujet du travail agricole il me semble quand même important de rappeler que le secteur agricole bénéficie déjà d'une particularité et je le soutiens à chaque PLF avec le dispositif TODE. Qui permet. Oui oui c'est ça qui permet une exonération de cotisations des employeurs du secteur agricole, et en cohérence avec nos. Positions précédentes nous ce qui nous soutiendrons cette pérennisation. C'est la raison pour laquelle au sein de mon groupe. Nous sommes profondément surpris par la fille de philosophie des articles 19 et 20 août cette idée l'tente d'envoyer des personnes éloignées de l'emploi dans les champs qui relève d'une vision bien particulière du travail d'autant plus que ces articles ignore déjà les conditions de travail difficiles, rencontrées par de nombreux saisonniers mais aussi les difficultés pour les exploitants agricoles d'avoir des locaux adaptés pour recevoir convenablement. Une telle main d'oeuvre pour ces raisons nous nous opposerons à l'ensemble des articles qui reviennent sur le droit des travailleurs enfin et il s'agit certainement du point le plus inquiétant de cette proposition de loi. De nombreux articles prévoient des retours en arrière inconcevable sur les aspects environnementaux. Alors que le président du Sénat vient de mettre en demeure l'un des principal lobby des pesticides Pittis pour avoir fourni des informations erronées. Ou parlementaires, vous faites le choix. Mes chers collègues de rouvrir la porte à un certain nombre de pratiques et de revenir sur des acquis pourtant difficilement obtenu la réautorisation d'épandage aérien pour des produits phytopharmaceutiques revient de manière incompréhensible incompréhensible sur les conclusions d'un rapport sénatorial je cite le titre pesticides le risque 0 initiée par notre collègue Nicole Bonnefoy et adopté à l'unanimité ici même la réautorisation des promotions sur les pesticides et la suppression de la séparation du conseiller de la vente pour ces mêmes produits représente également un retour en arrière sur une disposition difficilement acquise ici-même lors de l'examen de la loi Egalim. Je rappelle simplement que nos collègues rapporteur sur ce texte, Michel Raison, qui n'est plus avec nous et Anne-Catherine Loisier qui est présente dans l'hémicycle, avait défendu le maintien de la séparation du conseiller de la vente, prévue dans le texte gouvernemental en 2018 seulement 5 ans plus tard, vous faites le choix de les déjuger et de revenir sur ce maigre acquis. L'Artec le 13. De cette proposition de loi est certainement le plus problématique. Alors que l'Inde c'est c'est une agence d'expertise scientifique indépendante vous choisissez de lui donner un rôle politique en incluant dans ses missions, la réalisation d'une balance détaillé des bénéfices et risques sanitaires, environnementaux et économiques de la décision envisagée et en plus de tout cela, madame la rapporteur vous avez ajouté la possibilité au Ministre de l'Agriculture de suspendre certaines décisions de l'inceste et même la faculté pour le ministre, de prendre une décision relative à une autorisation de mise sur le marché. Très sincèrement, mes chers collègues, très sincèrement, comment pouvez-vous avoir cette vision d'une agence indépendante indispensable pour éventuelle pour évaluer scientifiquement un produit ça phytosanitaires. Comment pouvez-vous en tant que parlementaire souhaiter une concentration d'autant de pouvoirs dans les mains du ministre. J'aurais pu parler des délais de grâce sur les pesticides interdits mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans les débats. Enfin, concernant l'eau. La majorité sénatoriale fait le choix de jeter de l'huile sur le feu en créant un motif d'intérêt général majeure dont personne, alors là pour le coup, personne n'est capable d'en donner la définition précise. Et en réduisant les contentieux dans une triste vision du rôle joué par la justice. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, au sein du groupe socialiste du Sénat. Nous nous opposerons fermement à cette proposition de loi et nous proposerons logiquement la suppression d'une grande partie des articles ce 1er est donc particulièrement engageant mais nous serons mes chers collègues, défendre un autre modèle agricole compétitif. Pérenne. Respectueux de l'agriculteur du consommateur et de l'environnement. Je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. S'il y a bien une chose que notre groupe partage avec ce texte. C'est l'idée que notre modèle agricole doit être transformée en profondeur. Pour le reste. Nous ne partageons ni la vision de l'agriculture développé dans cette proposition de loi ni les solutions. Qu'elle entend mettre en avant, c'est donc 2 visions qui s'opposent. Poser le sujet de l'agriculture, c'est aborder un système complexe. Plongée au coeur de l'économie mondialisée et qui mêle entre elles plusieurs questions essentielles. La question d'abord des ressources naturelles de l'eau. De l'air de la terre qui nous nourrit et dont nous devons prendre soin. Car nous n'en avons aucune. La question également central du travail. Et de la rémunération des femmes et des hommes qui nous permettent de nous nourrir et qui vivent où chaque jour les conséquences d'un changement climatique qui s'accélère et enfin la question du droit à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous. L'enjeu est de taille. Nous ne pouvons désormais que le constater c'est une alimentation à 2 vitesses qui s'est mis en place dans notre pays. Propulsé par une inflation alimentaire sans précédent et par les échecs de décennies entières à favoriser les traités de libre-échange plutôt qu'à encourager et accompagner une agriculture locale bio et paysanne les phénomènes d'agrandissement de spécialisation qui entraîne des accaparement foncier et qui conduisent à une disparition des paysans sont ignorées et passé sous silence la compétitivité par le prix pardonnez-moi de réflexion mandat après mandat, gouvernement après gouvernement sans reconnaître les spécificités de l'agriculture ni l'absolue nécessité d'une exception agricole, les traités de libre-échange reste la logique de la politique agricole française sans cesse guidé par le moins-disant social et environnemental, sans parler de la PAC. Donc il faut revoir les priorités et les critères. Ces raisonnements nous conduisent sur une pente dangereuse celle du renoncement, mais aussi du dénigrement parfois de l'administration et des agents publics en particulier Lanxess. Dont vous Monsieur le Ministre nous avait dit qu'elle n'a pas vocation à décider de tout tout le temps en dehors du Champ européen et sans jamais penser aux conséquences pour nos filières. Alors vous avez raison, Monsieur le Ministre, parfois on peut concilier intérêt économique et sociale mais souvent. Souvent. Privilégié les intérêts économiques de court terme va à l'encontre de la défense de l'intérêt général de la Santé et de l'environnement et non nous n'avons pas le temps de faire une pause environnementale de 5 ans, n'en déplaise au président de la République, ni sur la qualité de l'air, ni sur la qualité de l'eau, ni sur la qualité des sols, sur ce dernier point, d'ailleurs nous allons d'aberration d'aberration et nous le voyons bien sur la question des retenues d'eau déclaré systématiquement sans distinction qu'elle relève de l'intérêt public majeur reviendrait à autoriser toutes les mégabassines. L'eau doit être considérée comme un bien commun et sa gestion doit reposer sur le triptyque préservation. Partage et juste répartition car l'eau est une ressource indispensable à la vie et la réalisation de tels ouvrages se faire à partir de critères de faisabilité de pertinence scientifique et d'objectifs d'utilité publique. Quant au projet de territoire pour la gestion de l'eau, ils n'ont pas vocation à donner blanc-seing à toutes les mégabassines mais bien m'a interrogé l'ensemble des possibilités sur un territoire pour optimiser répartir et préserver la ressource en eau enfin. Dernier point et non des moindres, la question de l'emploi et du travail agricole. Le milieu perd des actifs, il peine à renouveler les départs à la retraite et c'est toute une politique de l'emploi qu'il faut revoir pour lutter contre les conditions de travail dégradées et notamment contre les dispositifs fiscaux qui encore encourage le recours aux contrats courts et saisonniers. Plutôt que le précariser le travail agricole il faut renforcer son attractivité et garantir des conditions de travail dignes aux hommes et aux femmes qui nous permettent de nous nourrir en France mais aussi partout dans le monde car c'est tout un système mondial qu'il faut repenser un système ou des multinationales toujours plus avides de profits épuisent les Terres des pays en voie de développement. Exploite les populations locales. Condamne la biodiversité et avec elle toute notre humanité. Un système où le capitalisme règne en maître sur des marchés mondiaux et où les agricultures vivrières et les petites structures n'ont pas leur place au traité de libre-échange à la compétition mondiale, il faut opposer les coopérations entre pays inverser les logiques à l'oeuvre dans ce capitalisme dévastateur pour lui même pour la planète. Pour finir, la rémunération du travail paysan. La réduction du réchauffement climatique, l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous la préservation de la biodiversité sans les seules conditions d'une sécurité alimentaire française et mondiale et elle sont incompatibles avec les lois du profit. Je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion. La parole est à Madame. Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Merci monsieur Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues. Alors où le commerce international de produits agroalimentaires n'a jamais été aussi dynamiques. La France est l'un des seuls grands pays agricoles, dont les parts de marché recule était elle est ainsi passée du 2ème au 5ème rang d'exportateur mondial en 20 ans 2 tiers de ses pertes de marché s'explique par son manque de compétitivité, la France décroche en raison de plusieurs facteurs, la hausse des charges liées au coût de la main-d'oeuvre ou sur-transpositions à une fiscalité trop trop lourde, une productivité en berne du fait de moindres investissements dans l'agroalimentaire et de l'effet de taille d'exploitation de la ferme France ayant historiquement, un modèle familial à la différence de bon nombre de nos concurrents et enfin sept ans gris bashing qui vitupère un modèle agricole comptant pourtant parmi les plus vertueux du monde en matière environnementale. Face à ces constats. Notre responsabilité politique et dès lors d'adapter notre modèle agricole et nos politiques publiques nationales afin de concilier compétitivité Innovation, transition environnementale et attractivité. Mot d'ordre réaliste qui doivent désormais guider nos politiques publiques à court, moyen et long terme. La proposition de loi issus de l'initiative transpartisane de nos collègues, Laurent Duplomb, Pierre Louÿs et Serge mais Riou que je salue propose des premiers éléments de réponse déterminant pour l'avenir de la ferme France et offre aussi des perspectives pour les générations d'agriculteurs qui vont s'engager. Parmi les mesures stratégiques pour le groupe Union centriste, la facilitation du financement des investissements agricoles face aux grâce au au Livret A gris, le soutien aux filières ayant recours aux saisonniers TODE en raison de leurs spécificités. L'augmentation des seuils d'exonération de l'impôt sur les revenus agricoles afin de redonner des marges de manoeuvre aux agriculteurs et enfin la fin des discriminations comme les surtranspositions ou la non application des clauses miroirs, le travail en commission et l'investissement de notre rapporteur Sophie Primas a permis d'enrichir le texte afin de mieux protéger notre agriculture des distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne a permis aussi elles nous ont permis aussi de modérer les charges pour que le revenu des agriculteurs ne soient plus la variable d'ajustement de la compétitivité et que nos atouts relevant de la compétitivité hors prix soit mieux prise en compte, enfin elle nous a permis de faciliter, en tout cas elle nous engage à faciliter l'innovation agricole clé de la transition énergétique et écologique. En commission, nous avons ainsi clarifier le rôle du haut commissaire à la compétitivité pour pour simplifier, et pour structurer les politiques agricoles. Nous avons validé l'usage des drone afin de permettre une pulvérisation aérienne de précision des produits phytosanitaires. Nous avons approfondi le sujet décisif et tant attendue des clauses miroirs, enfin il nous a paru effectivement déterminant de redonner la main aux politiques en ouvrant la possibilité au Ministre de l'Agriculture de suspendre temporairement une décision de l'an cessent de retrait de mise sur le marché des produits sanitaires dans des conditions déterminées. Avec plusieurs de mes collègues centristes nous présenterons des amendements complémentaires qui viseront à mettre un terme à cette concurrence déloyale qui sévit dans le commerce des Miel à soutenir l'emploi de saisonnier dans les entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers a accéléré la prise du décret de la loi Egalim 2 visant à rendre obligatoire l'indication du pays d'origine ou le lieu de provenance des viandes utilisées en ingrédients à mieux valoriser le stockage de carbone dans les sols agricoles ou encore à renforcer les fonds propres des coopératives. Alors que la loi d'orientation. Et d'avenir agricole sera présenté à l'Automne au Parlement, le Sénat prend ainsi date avec ces propositions qui engage notre modèle pour les 15 années à venir, modèle pour lequel nous souhaitons concilier et non opposés pour assumer les défis sociétaux de décarbonisation de gestion de l'eau qui sont devant nous, la survie et la prospérité de nos entreprises agricoles dépendra de notre capacité à concevoir ses modèles multifonctionnel qui servent les trois piliers d'un développement durable économique environnemental et sociétal avec ma collègue, Nadia Sollogoub, qui complétera mes propos. Nous saluons les avancées portées par ce texte et confirmant qu'une grande majorité du groupe centriste votera en sa faveur. Je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion. La parole est à monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui, je le souhaite vivement, fera date pour la compétitivité de notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. Je tiens d'ailleurs à saluer ici le travail de nos collègues, Laurent Duplomb, Pierre Louÿs et Serge Méry, auteur du texte. Issu d'un excellent rapport d'information sur la compétitivité de la ferme France adoptée en septembre 2022 par la commission des affaires économiques. Cette proposition de loi transpartisane a pour but d'inverser le déclin de notre puissance agricole le Sénat alerte d'ailleurs le gouvernement à ce sujet depuis plusieurs années maintenant. Car la situation est vraiment alarmante. La France importe plus qu'elle n'exporte de produits alimentaires et la concurrence européenne et internationale lui a fait perdre des parts de marché très importantes. Comme le point très justement nos collègues, nous nous sommes repliés sur une production de denrées haut de gamme qui certes fait la fierté de la France mais qui pour autant n'est pas suffisamment rémunératrice pour nos agriculteurs. Et beaucoup de nos concitoyens, notamment parmi les plus modestes se trouve ainsi contraint de consommer des produits importés sans parler de la restauration hors domicile, cela n'est plus concevable. Les causes de cette perte dramatique de compétitivité, nous les connaissons. Surréglementation, charge des producteurs excessive productivité faible coût de la main-d'oeuvre fiscalité trop lourde, manque d'investissement. Ce à quoi s'ajoute aujourd'hui la crise des prix de l'énergie et l'inflation. Or, la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Ne nous ont que trop bien rappeler l'importance géostratégique de la souveraineté alimentaire. Il est grand temps de réagir et de rendre du souffle à l'agriculture française dans son ensemble, notamment par des investissements d'avenir et les et les innovations en matière de transition des pratiques agricoles. C'est l'esprit de cette proposition de loi. En effet, le texte que nous allons examiner, composé de 26 articles à plusieurs objectifs. Assouplir le cadre normatif lutter contre les sur-transpositions améliorer le cadre fiscal pour susciter l'investissement encourager l'innovation pour la productivité et accompagner l'agriculture dans sa transition. Madame la présidente, rapporteur Sophie Primas dont je salue également le travail il y a adjoint des dispositions pour alléger les charges pesant sur les agriculteurs et des mesures pour préserver davantage l'agriculture française des distorsions de concurrence européenne et internationale. La ligne d'horizon de ce texte reste le triptyque bien mangé prix abordable pour le consommateur français est juste rémunération des agriculteurs. Ce que nous défendons ardemment au Sénat. Parmi les mesures phares, la création d'un Haut commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires françaises auprès du ministre de l'agriculture et la mise en oeuvre d'un plan quinquennal vont permettre de définir de véritables objectifs agricoles avec de vrais responsables. Le rapporteur a également introduit la possibilité pour le ministre de l'Agriculture, de suspendre à nouveau une décision technique du directeur général de l'ASS. Par ailleurs, le fonds de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficultés et l'augmentation des plafonds de la déduction pour épargne de précaution viendront soulager les producteurs notamment les éleveurs les éleveurs en difficulté. Enfin l'accompagnement de nos agriculteurs face au dérèglement climatique étant crucial pense aux défis du partage de l'eau, notamment au risque aussi d'd'aggraver encore les pertes de compétitivité ce texte rend possible la réalisation d'un diagnostic carbone et de performances agronomiques des sols pour les structures agricoles cofinancé par l'État. Le rôle de l'agriculture dans notre transition écologique et faut-il le rappeler à ce titre-décisif. Il est donc nécessaire de donner à nos agriculteurs les moyens d'agir encore plus pour la préservation de la biodiversité, notamment notre bocage. En somme, à travers cette proposition de loi, il s'agit d'être cohérent. Si nous voulons défendre notre puissance agricole et retrouver notre souveraineté alimentaire il nous faisons. Il nous faut nous en donner les moyens. Car, ne soyons pas naïfs sans compétitivité nouvelle nous ne parviendrons pas à rendre aux métiers agricoles leur pleine attractivité avec des rémunérations justes et à enrayer aussi l'érosion du potentiel de production que nous constatons constatons dans nos territoires, par exemple, dans mon département de la Mayenne. Entre 2010 et 2020, nous avons perdu plus de 1000 fermes dans le même temps le nombre de chefs d'exploitation a diminué de 17%. Donc ne perdons pas de temps et saisissons l'opportunité de cette proposition de loi ambitieuse pour construire une agriculture française forte dynamique et durable. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Si le président, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui de la compétitivité de la ferme France à peine quelques heures après une manifestation organisée à Versailles par le président Macron et intitulé tout sens la la terre de France nos agriculteurs l'ont choisi, il la travaille tous les jours et à l'instar des autres entrepreneurs à qui s'adresse notre chef d'État. Ils font chaque jour de la production et du négoce. Ils sont comme les autres chefs d'entreprises dans des obligations de rentabilité des problématiques de cours nationaux et internationaux, des soucis de recrutement des galères administratives, ce sont des businessmen Farmer. Mais leurs clients nationaux et internationaux, les consommateurs de leurs produits eux choisissent de moins en moins la France. Très conscient de cette forme de décroissance et faisant suite à leur rapport d'information nos collègues Laurent Duplomb Pierre-Loup et Serge mais Riou nous propose un texte aux mesures concrètes, opérationnelles, inspiré des difficultés identifiées dans les exploitations. Il y a urgence à ce que les politiques publiques décide de donner un cap à une reconquête stratégique national, ne pas attendre de de voir un jour re agree Colisée la France comme nous devons aujourd'hui essayer de la ré-industrialiser ne pas devoir pleurer notre agriculture perdu comme nous pleurons aujourd'hui notre industrie perdu. Créer un Haut Commissariat à la compétitivité agricole lui donner des outils du pouvoir et des moyens. Ce sera un signe fort, à condition que ce ne soit pas un machin de plus et surtout pas une coquille vide. Oui la compétitivité agricole doit être surveillée avec la plus grande attention, et pas seulement constaté a posteriori ou plutôt son absence à l'aune des disparitions d'exploitations ou des des capitalisations du cheptel. Oui nous devons éradiquer la sur-transposition des normes qui entravent là comme ailleurs le fonctionnement des entreprises. Ce qui est particulièrement grave en agriculture c'est qu'on lui demande dans le même temps de s'adapter aux changements de l'environnement, tout en restant dans un carcan rigide et de plus en plus contraignant. L'agriculture depuis la naissance de la vie sur Terre n'a cessé d'évoluer selon les besoins des hommes et le contexte naturel. L'agriculture a suivi l'évolution du monde poursuivant constamment sa mission nourricière. Si elle ne l'avait pas fait l'homme aurait disparu. Et pourtant en France aujourd'hui pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. On enchaîne, on la ligote dans des injonctions contradictoires, prenant le risque insensé de l'affaiblir gravement. Nous devons lui rendre la liberté d'évoluer. Donner plus de moyens à son soutien qu'à son contrôle et encourager massivement l'innovation en agriculture, comme le propose cette PPL ce n'est pas le chant qui fait la moisson c'est le Labour dit justement un proverbe espagnol sanctuariser des parcelles agricoles n'est pas une fin en soi. S'il n'y a pas de bras pour les exploiter et et n'est pas inutile de rappeler ce prérequis face au risque d'excès du zéro artificialisation nette. La folie administrative les sur-transpositions malvenu quoi que pétrie de bonnes intentions, mais aussi les distorsions de concurrence par rapport aux autres pays producteurs sont autant de verre qui ronge la ferme France il faut avec bon sens et de toute urgence éradiquer les inepties décrété un vrai plan de relance d'une production agricole compétitive et concurrentielle, la fiscalité est un vieil outil qui sait être souvent efficaces, utilisons-le à bon escient. Un enjeu essentiel est aussi la transmission des exploitations et surtout le renouvellement des générations. D'une façon générale, une entreprise déficitaire ne trouve pas de repreneur. Aussi l'enjeu de prospérité compétitivité est-il d'autant plus vital. Nous déplorons aussi qu'actuellement, il soit beaucoup plus facile de s'agrandir, que de reprendre une exploitation et c'est une dérive que nous risquons de dont nous risquons très vite de faire les frais. Enfin, je souhaite vous faire partager ma réflexion sur la non-valorisation des apports de l'agriculture à notre société elle doit s'adapter aux évolutions climatiques, elle est en charge de notre souveraineté alimentaire et s'inscrit désormais comme un producteur d'énergie, elle est l'acteur essentiel de la décarbonation elle est dépositaire des enjeux de biodiversité. Il est temps de comprendre qu'on ne peut pas avoir tout pour rien. Je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame, Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. C'est le président, Monsieur le Ministre, madame. La présidente de de la commission des affaires économiques, Madame Prima, mes chers collègues. Quelques mots au lieu et place de Jean-Pierre Vogel, le président du groupe cheval qui devait intervenir dans cette discussion mais qui a été retenue et éloigné de nos bancs ne je prend ainsi sa place si je puis dire, en qualité de vice-présidente du groupe cheval. Quelques mots sur. L'économie générale de cette proposition de loi mais je crois qu'elle a été très largement présenté depuis le début de cette discussion générale je m'y attarderai assez peu. Nous connaissons tous la situation de nos agriculteurs en France d'une agriculture qui est percluse de de normes de charges les normes étant une charge particulière et qui se trouve dans un environnement juridique si contraints qu'elle a perdu de sa compétitivité. Lorsque l'on connaît la la démographie agricole, hé bien il était urgent je remercie les 3 auteurs de cette proposition là d'avoir fait de pouvoir redonner ce choc de compétitivité à notre agriculture dont nous avons tant besoin, et qui je crois brille par son excellence unanimement reconnu. Pour autant, c'est l'article 25 de cette proposition de loi qui m'amène à prendre la parole. Il s'agit de l'application à la filière équine d'un taux de TVA intermédiaire de 10%. Cela est assez technique, cela a néanmoins été fort bien compris par Madame Prima et monsieur du plomb qui ont soutenu cette disposition qui émane du du groupe cheval et plus particulièrement de de son président et qui remercie tous les co-cosignataires de cet amendement. Je rappelle pour mémoire que. Pendant. Quelques années de de 2004 à 2012, la filière équine bénéficie d'un taux de TVA de 5,5% qui était particulièrement bénéfique à son développement que malheureusement en 2012, la Cour de justice, des communes de la communauté européenne s'appuyant sur une directive européenne. A imposé que ce taux de TVA passe de 5,5% à 20%, vous imaginez que 14,5 points de plus de TVA a été extrêmement préjudiciables à la filière. Tous les gouvernements successifs depuis, se sont engagés à revenir sur ce taux élevé et qui empêche la compétition la compétitivité de notre filière équine. Dans la mesure où le cadre européen évoluerait cela est désormais chose faite, sous la présidence française ce cadre européen et évoluer. Il est donc important. Je crois que les engagements des gouvernements successifs soient tenus et que nous puissions maintenir ce taux de TVA à 10% comme cela a été fixé dans le texte qui se présentent à vous, c'est bien sûr à vous monsieur le ministre aussi que que je m'adresse pour que. Cette attente importante de la filière équine. Soient. Effectivement respectées et qu'il y soit répondu en maintenant ce ce taux à 10% pour la filière équine. Merci à vous. Merci cher collègue. Monsieur le Ministre, vous souhaitez. Pour. Sur cette discussion générale. Son engagement continu sur les sujets agricoles hé bien noté les points qu'il a évoqué. Indiqué aux sénateurs Gremillet aussi sur la question de l'épargne de Pro caution. Alors on en reparlera dans les amendements mais il me semble que nous avons fait une première un premier travail et je sais que c'est un sujet important de stabilisation, y compris de compétitivité. On a fait une une première étape me semble le-t-il en 2023 sur le budget 2023 en stabilisant le dispositif sur 3 ans. Il faudra qu'on en reparle au moment des amendements ou de de l'examen de cet article. On a besoin aussi de redéfinir ce que les les épargne de précaution. Quels objectifs elle vient viser parce que ne serait-ce ne n'être que dans la prolongation d'un dispositif qui a montré son intérêt. Il me semble que ça suffirait pas monsieur mais villes vous avez évoqué la question de. de dire qu'on a, on a perdu en compétitivité depuis un certain nombre d'années, je cherche du regard. À vrai dire, ça fait 23 ans au moins. Je pense qu'il faut aussi qu'on assume collectivement. Ce qui a été fait sous plusieurs septennat quinquennat le principe de précaution, c'est sous le septennat. De Jacques Chirac. Le Grenelle de l'environnement, c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et et l'oeuvre est continue depuis 25 ans. Alors soit on dit qu'on se met en rupture. Total avec ce que nous avons fait depuis 25 ans soit on sait qu'on est dans un cadre. Qui est un cadre intéressant qui encadre que nous assumons collectivement que le gouvernement peut prendre sa part. Mais tout le monde devrait là la prendre à la vérité, nous sommes dans un pays qui a le seul du monde à avoir décidé du principe de précaution et s'est inscrit dans la constitution là on pourrait revenir sur ces débats-là mais. Il me semble qu'on aurait plutôt intérêt à essayer de dire dans le cas de qui est le nôtre avec notre tempérament français qui est différent des autres pays, comme on essaie d'évoluer sans remettre en cause ce qui a été une oeuvre commune même si elle peut avoir, mais semble-t-il des défauts. Je je je je je pense que c'est important de le dire, c'est le sénateur. La baie de de choses. On en reparlera tout à l'heure mais la question. La question des drone. Il faut qu'on essaie de pas caricaturer ces questions. Vraiment. Je ne crois nullement que l'intention du législateur là et que d'ailleurs il y a des expérimentations qui soit en cours, soit de. De. Dépendre plus c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et donc quand on est dans une voie qui vise plutôt à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires que nous encourageons et que nous partageons collectivement je crois. N'essayons pas de dire que, par nature, le drone. Parce que nous aurions un sujet par rapport à. À l'outil lui-même. Alors il a d'autres usage parfois le droit enfin le drone il peut avoir des usages agricoles qui sont intéressants, y compris d'ailleurs en terme de sécurité, je le dis pour les agriculteurs notamment dans les territoires qui sont un peu escarpé. Alors c'est moins le vôtre et moi le mien. Les territoires escarpé. Mais il y a des territoires où la l'utilisation du drone elle vient sécuriser aussi le travail des agriculteurs. Donc faut aussi le regarder comme ça et pas forcément comme une contrainte et puis de vous dites. Vous avez dit hou la tomate a besoin d'eau alors je on va on va même se mettent d'accord la tomate bio et la tomate conventionnels ont besoin d'exactement la même quantité d'eau. Et c'est valable même pour le maïs. Et même pour l'agriculteur éleveur qui décide de passer en bio qui a besoin de maïs pour compléter son alimentation en bio, il a besoin d'autant d'eau en maïs. Que quand il est en conventionnel. Alors après qu'on ait un sujet sur est-ce qu'on réfléchit sur la manière de mieux utiliser l'eau et comme on fait pour mieux stocker l'eau dans les sols et ça c'est un sujet qu'on peut partager mais essayons de nous dire de grâce que l'agriculture a besoin d'eau. Sans caricaturer non plus un besoin qui serait excessif et sans dire. Aussi et ne, et oublié de dire que nous sommes parmi les les les pays qui utilise le moins d'eau qui a le moins de surfaces irriguées. fond a moins de surface irriguée, que les Pays-Bas. Et il m'avait échappé, que nous étions un pays qui étaient moins soumis à contraintes. Climatiques que les Pays-Bas sont jugés de la météorologie des Pays-Bas qui par nature ne me regarde pas. Madame la sénatrice j'nagé vous avez évoqué les questions qui peuvent éventuellement faire l'objet de réserve et je comprends et on en reparlera dans un moment, mais merci en tout cas de ce que vous avez dit sur le sujet Non, il n'y a pas de jeu politique. Il peut arriver entre le Sénat. On a des débats avec le Sénat, on est penché pas la courte échelle les. Ça serait faire grief quand même hein. Monsieur du plomb à madame la présidente Prima et à moi-même que nous serions capables de nous influencer vedette des influencer somme des esprits suffisamment libre et indépendant. Pour vivre nos vies séparément si vous me permettez de le dire ainsi, pour avoir des points de vue. Parfois des équivalents, mais parfois même des points de vue différents et qu'on l'assume dans la liberté du débat démocratique, on ne cherchait pas des choses compliquées. Il me semble que il y a des sujets d'ailleurs qui sont dans ce texte et je le dirai tout à l'heure qui remonte, y compris des concertations. Et il faut les entendre aussi, quand bien même, vous ne soyez pas d'accord et il me semble que c'est un élément qu'il faut entendre a dans les concertations. Les sujets de l'eau sont remontés. C'est la vérité et et ne pas et faire comme si ça n'existait pas, je pense qu'on a besoin. j'ai pas dit vous disiez ça, je dis on a besoin, collectivement, de se dire on a un sujet autour de l'eau, il faut qu'on essaie de le dépassionner d'avancer concrètement et donc. C'est ça qui est important. Monsieur Monsieur Guey, je vous remercie d'avoir cité les grands auteurs puisque vous m'avez cité, ça me touche beaucoup. Sur un certain nombre de sujets mais simplement dire que sur la question. De de. J'ai dit effectivement sur ne cesse pas tout pas tout le temps. J'ai j'ai rien à retirer de ce que j'ai dit pas tout, pas tout le temps comme je l'ai dit aux sénateurs. Seulement il y a des cas où monsieur seulement me demande de revenir sur les avis de Lanxess. Pas tout pas tout le temps. Et j'ai pas l'impression d'avoir commis un acte révolutionnaire. Enfin j'ai l'impression que si parce qu'en fait. J'en ai un peu. Fait les frais, si je peux dire mais j'assume ce que j'ai pas tout pas tout le temps mais jamais j'en rabattre sur des questions de santé. Et personne ici n'a envie d'en rabattre sur les questions de santé et puis 2ème élément il n'a il n'est nullement question. Pardon. Regardez les trajectoires dans lequel on est sur les questions de carbone. Il n'est nullement question de faire une pause environnementale enfin on est quand même sur un objectif de neutralité carbone en 2050. Si vous appelez ça une pause. Enfin faut quand même regarder la trajectoire ce qu'il faut pas changer les règles tout le temps parce qu'après on peut pas organiser des filières quand les règles sont changées, tout le temps il me semble, c'est un élément important sénatrice loisirs et voter vous Khalek voit comme ça a été fait. Par d'autres. La question du financement agricole et la nécessité des des innovations. Moi je crois beaucoup à la, au sujet des innovations leur c'est moins dans ce texte, mais on a besoin de porteur. Le drone en est un élément mais il me semble qu'on a besoin de, de penser que les innovations peuvent être. Importantes. Monsieur je vous dis vous avez OK alors que la situation alarmante. Tout le monde est d'accord là-dessus j'ai j'ai évoqué l'idée que c'était une oeuvre collective au mauvais sens du terme. Vous avez parlé d'un triptyque, il me semble qu'il manque dans votre triptyque un, trois et un 4ème pieds si vous me permettez cette expression. C'est quand même la question de la transition. vous avez des qualités vous avez mais la la la neige je finirais là dessus dans deux minutes. La nécessité de la transition. Elle est importante, on ne peut pas ne pas dire aux agriculteurs qu'il va y avoir des sujets de transition pas pour faire de la norme parce que c'est le moyen de garantir la compétitivité parce que à la vérité l'érosion du potentiel de production, il n'est pas les qu'à la norme. Le potentiel des sols est moins élevé aujourd'hui qu'il n'était il y a 20 ans, 25 ans, y compris dans un territoire comme le mien et y compris les agriculteurs, vous le. Donc on a besoin d'y réfléchir quand même de façon me semble-t-il, apaiser enfin malin ce look Madame Jourda. Vous vous êtes sur un sujet très particulier donc on on en débattra la volonté du gouvernement d'essayer d'avancer même si là on est sur un débat budgétaire et disons que c'est plutôt un peu plus tard mais je vois bien ce que vous avez voulu évoquer au nom de votre collègue en particulier un seul groupe sur la question. À la fois de la fiscalité, je partage des éléments à la question sur les. Vous dites, on a les entreprises qui sont déficitaires ne sont pas reprises.

C'est où tu l'as de la rentabilité que les choses se font et qu'on a besoin de porter mieux me semble-t-il avec. Les agriculteurs. La question du partage du du. De la mise à disposition des enfin, je voudrais juste conclure en disant puisqu'on va entamer mais les armements dire que hein vous me trouverez sur ce texte plutôt à regarder les sujets qui sont ouverts parce qu'on a besoin de se dire les sujets d'essayer d'éviter les caricatures. Deuxièmement, je le dis en particulier à monsieur l'abbé dont je doute quand même que ce soit sa dernière intervention au Sénat sur ces sujets-là. Même en discussion générale nous ne sommes qu'au mois de mai au fond. Moi j'essaie toujours dans le débat public de d'écouter ce qui sont y compris mes contradicteurs pour dire peut-être qu'il y a des choses à entendre des choses dont il faut tenir compte et je ne vous fais pas grief.

Que parfois je puisse défendent des positions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais qui ne sont pas des positions qui sont forcément à ne pas écouter quand on essaie d'écouter la position qui est la note sur la question de la productivité. Je ne crois pas qu'on fasse défaut. Vous ne trouverez toujours sur le chemin d'essayer de trouver la souveraineté de l'agriculture française

il faut donner des injonctions aux agriculteurs et puis, puis il y a ceux qui vous disent il faut les laisser faire. Tout va bien. Et continuons comme avant. Et vous ne me trouverez ni sur chemin là ni sur l'autre. Parce que je pense que ça serait une erreur de dire aux agriculteurs que les contraintes climatiques vont pas des contraintes puissant, ce serait une erreur de ne pas dire aux agriculteurs que nous avons intérêt à décarboner notre agriculture 4 degrés de plus. C'est le drame absolu pour nos agriculteurs et donc on a besoin de penser des systèmes qui soient plus résignant et donc j'essaie de trouver un équilibre que je vais essayer de trouver dans les dans les éléments du texte et les réponses que je serai sur les différents éléments pour faire en sorte qu'on ne tombe ni dans un ni d'un côté ni de l'autre et c'est pas du en même temps hein. En tant que telle, ce que je sens que vous allez me dire que c'est ça mais on a besoin de trouver un équilibre. Je ne me satisferait pas qu'on soit dans une situation, on ne puisse pas continuer à exercer nos prérogatives de souveraineté. Je ne me satisfait pas que plus de 50% des fruits et légumes produits en France consommées en France ne viennent pas de France et donc on a besoin de regagner en compétitivité en souveraineté de poser la question de l'accès à l'eau mais le dire aux agriculteurs que rien n'a va changer, ça c'est une autre démagogique que je me refuse à faire. Parce que celle-là. C'est confortable à la tribune. Mais celle-là elle amène aussi à la disparition de la souveraineté agricole française si on ne répond pas à cette question de la résilience du système on perdra aussi en souveraineté j'étais l'autre jour, dans les Pyrénées-Orientales, si je ne sais pas répondre à la contrainte sans dire à l'agriculteur, il y a qu'à changer de modèle. Parce que c'est facile de dire il y a qu'à changer de modèle. Vous êtes des gens qui font de la ville de l'arboriculture de l'élevage et un peu de maraîchage bon loin des caricatures de l'agriculture que vous nous mais parfois industriel et il va bien falloir qu'on les accompagne parce que ai la résilience. C'est pas la disparition de l'agriculture la résilience et comment continuer à exercer nos prérogatives de souveraineté sous les contraintes climatiques mais il faut décrire les contraintes. Il faut essayer de trouver des solutions et c'est ça qu'on doit aux agriculteurs il me qu'on a besoin et on doit ça aux agriculteurs et j'en termine par là, d'avoir un débat apaisé on n'a aucun intérêt à ce que la société se dresse, qu'on ne les agriculteurs que les agriculteurs soient dressés contre la société ou une part de la société et donc mais c'est pas pour tout le monde. Et je pense qu'on a besoin aussi de montrer qu'on construire ça parce que je sais, les témoignages de nombreux agriculteurs qui tous les jours, on a le sentiment de pas être compris. De pas être compris dans leur contrainte de pas y compris dans leurs pratiques agricoles. Donc on a aussi besoin de décrire les pratiques agricoles sans les caricaturer pitié n'essayons de ne pas caricaturer. Je vous assure on rendrait non seulement un service à l'agriculture et aux agriculteurs, mais aussi un service aux transition que nous allons être amenés à prendre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Ministre. Alors, nous passons. Ah la discussion du texte de la commission avec sur la 2 un article additionnel avant l'article 1er, deux amendements identiques, le 70, qui le défend. Sûr. Ce drame il aime. Non. Monsieur. C'est l'amendement de Madame, Noël c'est ça. Cet article vise à intégrer le la souveraineté alimentaire à la liste des intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que son indépendance de l'intégralité de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité de la forme républicaine de ces institutions. Des moyens de sa défense et de sa diplomatie de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel, scientifique, économique et de son Patrimoine culturel. À la lumière de la crise liée au Covid-19, qui a mis au jour la vulnérabilité de nos approvisionnements. De nombreux domaines, il est apparu avec une évidence renouvelé dans l'opinion publique et dans l'action des pouvoirs publics que la souveraineté alimentaire bien au nombre de ses intérêts fondamentaux de la nation pour autant à ce jour, cette notion de souveraineté alimentaire n'est consacré dans aucun code ni dans aucune loi cet amendement propose de corriger cette anomalie en donnant enfin toute sa portée symbolique à ce principe qui recouvre la capacité de production agricole et le taux d'auto-approvisionnement alimentaire mais diffère de loin l'auto-suffisance alimentaire qui elle ne serait ni possible ni souhaitable. Cet amendement présenté par Madame Noëlle permet ainsi de resituer la recherche de compétitivité. Érigée en priorité par la présente, proposition de loi comme un moyen parmi d'autres d'atteindre la souveraineté alimentaire objectif consensuel sur tous les bancs du Sénat. Sénat. Chers collègue le le amendements identiques, 79 monsieur Menonville. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. L'amendement a été admirablement défendu seulement pour dire que cette souveraineté alimentaire aujourd'hui et ne donne notamment depuis la crise sanitaire prend tout son sens et qu'il que cet amendement est donc extrêmement important.

sur ce que devrait être le monde de l'après-Covid. Comme le disent très bien les auteurs de ces amendements, il faut rappeler que l'impératif qui nous réunit tous aujourd'hui et celui de la souveraineté alimentaire. Je donne un vide l'avis favorable. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, messieurs les sénateurs. Justement, madame la présidente, je, je me permets madame la rapporteure. En l'occurrence. Je trouve que justement parce que c'est symbolique et que je sais qu'au Sénat, vous êtes vigilants pour faire la loi et pas faire dans le symbolique. Il me semble que d'abord je ne vois pas très bien la portée d'abord la la 2ème question ces souveraineté ou sécurité. Semble-t-il, parce que c'est pas tout à fait de même nature et que d'ailleurs une partie des actions qu'on a pu mener. Dans le cas du du de l'épisode malheureux de de la Covid ont ils ont été pris sous le registre de la sécurité parce qu'il y a un certain nombre de dérogations qui ont été produites sous le registre de la sécurité alimentaire j'entends bien le symbole et je et le nous partageons vous l'avez compris, la question de la souveraineté. Je ne vois pas ce que ça va bouleverser et deuxièmement, je ne suis pas sûr que c'est une portée dont on mesure tout à fait les choses, ça ne veut pas dire d'ailleurs que, y compris dans les travaux sur la le le le projet de loi d'orientation, nous n'ayons pas cette question de, comment on introduit le concept de souveraineté qu'viennent aussi balancer les politiques publiques et je ne suis pas sûr que sous cette formulation là ça sur la bonne donc c'est c'est une demande de retrait mais sinon c'est un avis défavorable. Merci donc je mets aux voix ces deux amendements. 70 et 79 identique, avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils sont adoptés. Article 1er une prise de parole de Stéphane Nomis. Madame la rapporteure, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est une réponse nécessaire aux problèmes rencontrés par le monde agricole ou plus exactement, c'était une des réponses nécessaires. Est-il utile de rappeler le truisme selon lequel de notre modèle agricole dépend notre souveraineté alimentaire. Le défi est grand, d'une part assurer une production agricole répondant aux critères quantitatifs, qualitatifs et environnementaux. Et d'autre part contrecarrer l'épuisement et le découragement de nos agriculteurs, notamment des plus jeunes qui s'interrogent, finalement sur la pérennité de leur métier que Daniel Gremillet l'a très bien dit tout à l'heure une inquiétude alimentée par des statistiques mortifère. Le nombre d'agriculteurs a été divisé par IV en 40 ans. Quant à cette réalité structurelle implacable. Se greffe en plus de violence, d'éléments conjoncturels. Nous sommes en droit de comprendre cette désaffection permettait aux sénateurs Picard que je suis de prendre l'exemple emblématique de la filière betteravière une filière victimes comme vous le savez du séisme de la jaunisse. Entraînant 30% de perte au niveau national et parfois jusqu'à 70% localement. Nous avions accordé des dérogations temporaires d'utilisation de protection des semences à la filière dérogations finalement proscrite par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en janvier dernier, la filière se retrouvant ainsi à être la seule en Europe dans une situation d'impasse technique complète, ce qui est aussi dramatique qu'ubuesque. Ce pan de l'économie agricole pèse de façon directe et indirecte 90.000 employes répartis autour des 21 sucrerie de notre pays. La présente, proposition de loi tente d'apporter une solution via son article 12 luttant contre les surtranspositions de mesures législatives si nous voulons que la maison agricole France a été dit reste debout dans les tempêtes climatiques, sanitaires, environnementales, économiques et administratives. Nous devons la soutenir avec force. Je sais que vous en êtes conscient et que tu allais votre objectif et je vous remercie Monsieur le Ministre de votre écoute et de votre détermination à relever ce challenge compliqué, vous l'avez compris, je voterai naturellement en faveur de ce texte. monsieur le président. C'est le ministre, mes chers collègues. L'institution d'un haut commissaire à la compétitivité des filières agricoles, alimentaires et agroalimentaire française, nous sommes pas utile voire même contre-productif cet article propose de faire de la compétitivité prix l'axe premier des politiques agricoles, alors que cette taxe correspond à la course au moins disant social et environnemental, comme l'affirme le rapport du CESE quel levier pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français, il convient de redéfinir la compétitivité qui ne doit pas être réduite à une question de prix et de coûts de production mais au contraire prendre en compte la qualité gustative et sanitaire des produits leur adéquation avec les attentes des consommateurs. Les emplois générés les impacts environnementaux. Car ces derniers éléments sont susceptibles vous le savez de générer d'importantes dépenses qui sont assumées de manière collective. Plutôt que de centraliser la gouvernance de l'agriculture sur une personne unique, il est de la responsabilité du ministère de l'agriculture en lien avec les ministères de l'environnement et de la santé de mener une politique à la fois agricoles et alimentaires qui prennent en compte l'ensemble des dimensions économiques mais également sociale écologique territoriale et sanitaires. C'est un ensemble, ça ne peut être simplement une compétitivité prix cela donc au lieu de focaliser uniquement sur cet axe de compétitivité prix c'est pour cette raison que, avec le groupe écologiste. Nous demandons la suppression de cet article, puisqu'haut-commissaire ne sera pas un élément déterminant pour aller vers une agriculture durable. Bien au contraire. Monsieur le président. Ils sont également que la création d'un coup d'un haut commissaire à la compétitivité des filières agricoles et alimentaires n'apportera pas de réponse à la crise profonde que connaît le monde agricole. outre que la compétitivité ne se décrète pas, elle ne saurait se résumer à une question de volume et de prix dans une recherche d'optimisation économique. Comme le souligne et ça a été dit très justement le 16. Dans son avis de 2018. La compétitivité ne peut se limiter à comparer les coûts de production et de vente où les volumes et les prix des produits souvent. La compétitivité inclut une large palette d'enjeux sanitaires, environnementaux, sociaux alimentaire foncier, ce qui n'apparaît pas dans la proposition de loi. Et ce n'est pas le manque de compétitivité entendue dans un sens restreint, voire dépasser qui tue notre agriculture mais bien la guerre des prix à laquelle se livrent les enseignes de la grande distribution et les grands groupes de l'agroalimentaire ainsi que la concurrence entre les États membres. C'est bien la financiarisation et la banalisation du secteur agricole qui met en danger le modèle d'agriculture familiale, c'est bien le libre jeu du marché, la course effrénée au meilleur rendement qui entraîne une forte forte volatilité des prix préjudiciable aux agriculteurs comme aux consommateurs d'ailleurs le libre jeu du marché est en ce sens. Contreproductif dans le domaine de l'alimentation. Enfin, il nous semble qu'en lieu et place d'une énième instance il importe de s'appuyer sur l'existant à l'exemple du conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux, qui est présidé d'ailleurs par le ministre en charge de l'agriculture et qui assurent des missions de conseil d'expertise d'évaluation, d'audit et d'inspection par exemple sur les questions stratégiques, comme l'agro-écologie et la lutte contre le changement climatique, la gestion des crises du marché ou de crise sanitaire, la pluie aussi à l'international. Il peut aussi participé à la conception des lois il nous sommes dès lors que la création d'un Haut commissaire serait redondante. Merci cher collègue madame la rapporteure. auprès des pouvoirs publics. Le haut commissaire, Monsieur le Ministre, n'a pas vocation à concurrencer votre poste de ministre chargé de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire mais plutôt d'alerter de recenser les sur-transpositions de regarder les bénéfice-risque mais aussi d'être un véritable relais pour les filières et également par les. Les compétences que nous lui avons donné, nous souhaitons également qui convoque la conférence annuelle de filière. Une conférence qui a été institué dans le cadre de la loi sapin de qui n'a jamais fonctionné et nous lui avons donné des compétences supplémentaires et donc nous demandons à ce qu'au au commissaire de la convoqué et de l'animer. Le rôle de ce haut-commissaire est aussi un rôle d'agrégateur des différents plans que subit l'agriculture le plan au le plan des filières le plan phyto. Et cetera et cetera et pour trouver une forme de cohérence sur l'ensemble et de guides sur l'ensemble de ces plans qui tombe sur l'agriculture. Voilà donc la commission est défavorable à ces deux amendements. Si Monsieur le ministre. Oui, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les députés. Les sénateurs pardon madame la rapporteure pardon pardon pardon pas. C'est la première fois que ça m'arrive en 6 ans. Mais je vois que vous êtes vigilant toujours. Sur cette question là en fait il y a il y a de de de registres dans cette question, il y a à la fois les amendements qui visent à la suppression, puis la création de dans le texte du saut commissaire ça a permis d'en dire juste un mot et je vais être court. Je le promets. que toujours quelque chose de paradoxal, a demandé à ce que le ministre. Et plus de poids politique dans les décisions et en même temps. De créer un commissaire qui pourraient d'une certaine façon. Créer une forme de concurrence. Politique, pour le coup, puisque c'est un haut commissaire. À ses prérogatives de ministres. Bon alors, en revanche je reconnais que votre proposition. Dans le texte initial a ceci d'intéressant qu'elle vient poser la question et ça vous avez raison de le dire, de la cohérence des politiques publiques c'est est ce qu'il y a un endroit. Est-ce que c'est le commissaire ou est-ce que c'est ailleurs. Et ce qui est a un endroit où on se soucie de regarder ce que tout ça est bien cohérent de message vis-à-vis des agriculteurs et de est-ce que ça va ça vient conforter l'idée de souveraineté agricole alors le c'est dans le texte initial et donc par ailleurs les amendements qui sont des amendements qui ne reviennent pas en cause qui ne remettent pas en cause au fond l'idée d'un commissaire, mais qui vient de dire je supprime parce que au fond je suis pas d'accord avec la terminologie sur la compétitivité au qui viennent amendé en disant il faut rajouter alors n'ayons pas peur du terme, je le répète, n'ayons pas peur du terme compétitivité la compétitivité c'est pas seulement le rendement la compétitivité, c'est la capacité dans un marché qui est ouvert à moins qu'on est ici encore l'idée qu'on puisse rester sur un marché fermé que français, d'avoir une ferme France qui ne soit pas et et non européens. Alors il une ferme France et des agricultures françaises qui soit compétitive dans l'espace européen d'abord déjà et d'abord et donc voilà, il me semble que le sujet que vous posez est un vrai sujet de coordination des politiques publiques qui est valable, sans doute en agriculture comme dans d'autres domaines. Je suis pas sûr que la réponse au commissaire sur la bonne mais étant juge et partie vous jugerai que mon avis là-dessus ne serait pas le bon mais en revanche l'idée de pas poser cette question me paraît pas bonne et donc il me semble, c'est un avis de sagesse de retrait mais sans que ça serait plus logique de le, de faire un retrait mais sinon c'est un avis de sagesse du Sénat. Merci, monsieur le Ministre donc je mais aux voix ces deux amendements. 11 et 57 avec un avis défavorable de la commission. Sagesse du gouvernement. Qui est pour. Qui est pour. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adopté le 27 monsieur Tissot. monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 1er de cette proposition de loi propose donc d'instituer, nous venons d'en parler. Au commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires, chargée notamment de piloter un plan quinquennal. De compétitivité des filières. Les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain ne s'opposeront pas à cette création, même si nous nous interrogeons fortement sur d'une part la nécessité de créer un nouveau commissaire quand nous pouvons nous interroger sur l'utilité de certains déjà en activité et. Je pense que celui auquel nous pensons tous ne fait pas beaucoup. Concurrence à un ministre. Eu égard à oh oh production et à l'activité que que nous avons tous noté mes chers collègues D'autre part sur les moyens dont il disposera pour mener à bien sa mission, nous pouvons lire dans l'article premier, qu'il pourra mobiliser à son gré des fonctionnaires ou des salariés de différentes structures du ministère de l'Agriculture. Au Auchan avec. Des chambres d'agriculture en passant par FranceAgriMer ou l'INRA en tout état de cause notre présent amendement vise à préciser. Les missions de ce futur haut commissaire à la compétitivité en inscrivant explicitement dans la loi que cette recherche de compétitivité devra se faire dans un cadre durable et le mot à à tout son sens et ne saurait être seulement guidée par des impératifs économiques ou des conquêtes de parts de marché donc cet amendement pourrait apparaître pour certains qu'on me rédactionnelle mais eu égard à cette création à là cette demande, portée par ce cette proposition de loi, nous estimons au contraire que cette précision est la bienvenue et nécessaire pour que nous l'on ne perde pas le un des objectifs qui a été notamment rappelé par notre groupe. Merci madame la rapporteure. Oui, comme il est ni dans les intentions de l'auteur ni dans ceux de la commission d'opposer durabilité compétitivité son à Novi favorable. Si Monsieur le Ministre sagesse. Je mais on voit le 27 avec un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient il être adopté le 121 de la commission. de nos filières agricoles et agroalimentaires n'est pas à la hauteur des enjeux. La conférence publique de filière semble être l'enceinte adaptée pour discuter de ces produits. Si d'accompagnement à l'exportation particulier sur l'agriculture et sur ces leviers c'est donc évidemment un amendement de la commission sur lequel on est. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la rapporteure mesdames et messieurs les sénateurs, c'est aussi un avis de sagesse, je dis juste en nous écoutant qu'on aurait besoin singulièrement dans le travail qu'on a affaire ici et, plus tard. De de mieux organiser les différentes instances qu'on a en agriculture, parce qu'on a beaucoup d'instances. Et c'est peut-être ça qui crée aussi le l'absence de coordination et qui nécessite qu'on ait besoin d'un haut commissaire. Et donc je pense qu'on aurait besoin aussi d'avoir une réflexion mais ceci dit c'est un avis de sagesse. Merci donc je vais au voile l'abonnement, 121 de la commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui. Pour.

Merci monsieur le président. Oui cet article. Additionnel article 1er vise à reconnaître le caractère d'intérêt général de l'agriculture dans le code rural et de la pêche maritime, l'agriculture est toujours dit me semble-t-il la grande oubliée des activités qualifiées d'intérêt général. Contrairement, des domaines comme la défense de l'environnement ou la mise en valeur des forêts. L'accès à ce statut d'intérêt général permettra les ruptures d'être davantage protégés par l'État. En favorisant les actions en faveur du maintien des exploitations existantes et de l'installation des jeunes agriculteurs. Cela permettra aussi et surtout de protéger davantage les activités agricoles contre les différentes attaques ou autres entraves dont certains se traduisent par des actions violentes contre les biens, ou les personnes. Qui touchent les agriculteurs et se multiplient. Afin d'assurer la liberté publique fondamentale, en particulier la liberté d'entreprendre. Droits de propriété. Droits de propriété qui a été singulièrement oublié dans l'histoire de Sainte-, Soline à particulier. je rappelle qu'on a mobilisé des escadrons de gendarmerie de forces de l'ordre pendant plusieurs week-ends uniquement pour, pour. Assurer la défense du droit essentiel de propriété. Merci cher collègue madame la rapporteure. Oui, chers collègues. Ça va être une demande de retrait puisque avec l'adoption de l'amendement de Madame Noël et celui de Monsieur mais nos villes qui étaient identiques. En fait il est satisfait. Merci, monsieur le Ministre. C'est la même avis que celui que j'ai porté tout à l'heure en disant qu'on est un peu dans le déclaratif et au-delà de ce qu'a dit la la présidente Prima ce sénateur. Ne pouvait pas dire qu'on n'a pas défendu à Sainte-, Soline et qu'faut quand même rendre hommage sans. Je crois qu'on le partagera. Rendre hommage aux forces de l'ordre, on a défendu le droit de propriété. Vraiment. Donc nous ne croyons pas qu'avec un amendement comme ça de toute façon je voudrais quelque chose de droit de propriété, il y a pas besoin de de cet amendement il existe. Il est d'ailleurs constitutionnelle, il est même déclaration des droits de l'homme et donc je pense que. Essayons de ne pas caricaturer les choses là non plus le doigt propriété ceci est bien ce qui a été défendu et le droit aussi d'autres et de de vivre dans des conditions pacifiques et donc c'est bien ça ce qu'on a essayé de faire, à Sainte-, Soline il faut rendre hommage aux forces de l'Ordre qui l'ont fait. Merci. Il est retiré monsieur Benamou est maintenu. Non il est retiré mais ça me donne l'occasion de préciser que c'était pas le gouvernement en particulier qui, mis en cause. Non non moi c'est tous les organismes, les les associations sous bénéfice de protection de l'environnement qui mettent en cause de manière permanente sous forme de mise en accusation de suspicion.

qui nous orientent des des des études à cinq caution scientifique enfin là par un scientifique. Qui va. Aboutir dans le Champ médiatique et qui donnent lieu à des reportages très suspicieux et très mettant en cause notre modèle agricole. qui a beaucoup d'effets qui a des effets indirects par les agressions, les violences, les intrusions dans les exploitations. Tout ça c'est l'effet indirect de cet environnement là c'est ça que je mets en cause et excusez-moi, j'aimerais que ne le discours public non seulement l'État effectivement poursuite de plus en plus fortement les personnes qui se rendent Coupat de violence à l'égard des agriculteurs mais qu'on remercie tous les matins, les agriculteurs de produire pour la France. C'est dans ce sens que je j'entendais que l'agriculture soit reconnue d'intérêt général au même titre que le boulanger et au même titre quelque part qu'un agent du service public. Imagine-t-on notre pays sans puissance agricole et sans capacité productive. Non c'est, c'est justement pour changer totalement le logiciel que on nous serine. De manière à au goutte à goutte depuis quelques années sur l'agriculture je. C'est dans ce sens là que mon amendement. Était proposé.

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de l'amendement que nous venons de défendre à l'article 1er, il s'agit de préciser que le plan quinquennal qui sera mis en oeuvre et pilotée par le haut commissaire devra intégré intégré une dimension durable. Le choc de compétitivité que certains de nos collègues appellent de leurs voeux ne saurait être guidé uniquement par des considérations économiques. L'urgence climatique nous appelle à des solutions durables prenant en compte la préservation de notre environnement de notre biodiversité et de notre santé. Je vous remercie. Oui, monsieur le Président en cohérence avec ce que nous avons fait à l'article 1, c'est un avis favorable. Merci, monsieur le Ministre. Avis de sagesse. Sagesse donc je mets aux voix l'amendement 28, avec un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté le 12 monsieur l'abbé.

et le ministre, chers collègues. L'objectif de ce, de cet amendement d'élargir le périmètre du plan quinquennal. L'idée d'en faire un outil de planification au service d'une compétitivité prise dans sa définition élargie qui comprend des dimensions sociale, environnementale et sanitaire la prise en compte de ces aspects permettra à ce plan de construire une véritable politique agricole et alimentaire de la transition agroécologique nécessaire au regard des enjeux environnementaux de santé d'emploi de bien-être animal nous en élargissant aussi la gouvernance qui est à ce stade exclusivement agricole à la fois au ministère de la santé et au ministère de l'environnement mais aussi à une représentation de l'ensemble des représentants agricoles à la société civile aux élus locaux et aux citoyens. sur l'investissement, l'investissement qui pour nous n'est pas l'unique solution et a des effets pervers la sur capitalisation le surendettement qui fige le système et empêche les transmissions nous proposons donc de le réorienter. Il s'agit de déterminer les priorités d'accompagnement de projets de territoire d'innovations sociales d'accompagnement de pratiques agronomiques vertueuse de rémunération des services écosystémique via des paiements pour services environnementaux et d'agriculture de groupe. Ce plan prévoit ainsi de définir collectivement objectifs chiffrés ambitieux, notamment pour organiser la nécessaire sortie des pesticides et des engrais azotés pour le développement de l'agriculture biologique pour des installations agricoles nombreuses dans les années à venir et il s'agit tout simplement pour nous de donner un cadre juridique pour définir un véritable plan de transition agricole et alimentaire que notre groupe appelle de ses voeux. durable et d'adaptation. Très au-delà de ce que les auteurs de la proposition de loi souhaitait et probablement très au-delà du possible et pour le coup il y aurait probablement un doublon avec le ministre de l'Agriculture avec beaucoup d'objectif dans ce plan qui dilue son objectif central qui reste la compétitivité durable il exclut également le le co-au commissaire, ce qui est pas dans l'esprit du dispositif et par ailleurs, je tiens à souligner que cet amendement est d'ores et déjà partiellement satisfait puisqu'à l'issue des travaux en commission ce plan quinquennal a été élargie, pour prendre justement en compte la problématique de l'adaptation des filières agricoles, donc c'est un avis défavorable. monsieur le président, monsieur le sénateur. C'est un avis défavorable également je dis juste que d'abord. C'est à la fois un texte qui vise à avoir des prérogatives très très large sur un périmètre très interministériel donc on, on va encore plus loin que ce que j'ai déjà trouvé un peu original tout à l'heure et puis 2ème élément vous c'est à la fois. un ministre a quasiment un un commissaire. À trois en tête ministériels plus voulu définissait la politique agricole française dans le même article, donc disons que. Là pour le coup, on est encore trop excessif dans le sujet, ça n'empêche pas qu'il y a des sujets sur lesquels on ait besoin de travailler et d'essayer de penser interministérialité, il me semble que c'est un avis défavorable pour ce motif là il me semble que nous n'avons pas besoin d'avoir des prérogatives qui viendrait dépossédé non seulement le ministre de l'agriculture mais aussi le ministre de la transition écologique et ministre de la santé de leurs prérogatives. Merci monsieur l'abbé. Oui, personne ne m'a demandé de le, de le retirer. Donc je vais surtout pas le retirer, mais simplement pour vous dire Monsieur le Ministre, que c'est un amendement d'appel d'appel au secours. Par rapport à un véritable plan une véritable trajectoire dont on a besoin, ce qui est attendu, parce que vous disiez tout à l'heure on ne peut pas passer du jour au lendemain. C'est vrai qu'on ne peut pas passer du drame mais il y a un moment où on se doit de se donner des objectifs et une trajectoire pour y arriver, alors par cet amendement on vous enlevez de votre grande solitude pour vous proposer de travailler avec vos de collègues de la santé et de l'environnement et à égalité. Monsieur le Ministre. Merci chers collègues dont je mets aux voix l'amendement 12 avec 2 avis défavorable qui. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 122 la commission madame le rapporteur. Cet amendement vise à indiquer que le plan quinquennal de compétitivité et d'adaptation doit tenir compte des. Spécificité des territoires ultramarins. Je rappelle que les secteurs agricole et agroalimentaire représentent dans les Outre-mer, 60% des effectifs salariés et je souhaite donc que ce plan se focalise non seulement unis sur l'Hexagone mais englobe l'ensemble de l'agriculture française. Oui, monsieur le président, madame la rapporteure. Par souci de cohérence puisqu'on est au dernièrement sur ce texte. C'était un avis favorable sur cet amendement qui vient quand même montrer aussi la préoccupation que nous devons avoir sur les territoires ultramarins, la question de la souveraineté de la sécurité alimentaire n'est pas posé du tout de la même façon et c'est bien de montrer d'identifier la nécessité que nous avons de relever des défis qui sont des défis absolument immense en particulier des territoires qui sont les plus éloignés. De la, de la métropole. Donc on a vraiment besoin d'avoir un regard particulier sur donc sans doute des actions spécifiques sur ces questions de compétitivité de souveraineté mais qui se pose dans des termes beaucoup plus en tout cas très différents, pardon du de la France. Hexagonale et donc c'est un avis favorable en cohérence malgré ce que j'ai dit au démarrage sur le le dispositif lui-même.

notamment lors du rejet en décembre 2018 de la proposition de résolution en faveur de la création des paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs. Il me semble important de rappeler qu'agriculture constitue un maillot l'essentiel de la stratégie d'atteinte. L'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. 2050. Fantassins agricoles font face à des contraintes climatiques économiques conjoncturels tout en son sexe pour voir autres des attentes sociétales de plus en plus forte en terme de préservation de notre environnement et la qualité des produits et des aliments

d'attractivité du notamment à un niveau de rémunération est suffisante de ses exploitants. Nous faisons face à une un défi inédit de renouvellement des générations. Il est désormais d'urgent que nécessaire de diversifier les ressources financières de agriculteur si nous souhaitons une agriculture attractive innovantes comme Benguigui durable sur. Cela passera par faire de la restauration. Et du maintien des écosystèmes une source. Inter de revenus et non pas une contrainte supplémentaire par l'exploitant. Ainsi, sur le modèle du principe. Pollueur-payeur, selon lequel frais résulte des mesures de prévention de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doit être supportés par le pollueur. Cet amendement a pour objet de Generali. Cela dit, je kiffe sur le problème. J'ai eu 2 dépollueur bénéficiaire. Ce bazar sur l'ai critères mesurables de service et sismique. Si madame la rapporteure. ou à maintenir les écosystèmes dont la société tire des avantages. Les paiements peuvent être réalisés par des entreprises ou par des collectivités publiques. Le principe est en réalité similaire à celui du Label bas-carbone que nous verrons tout à l'heure à l'article 9, le fonds spécial dont il est question dans cet article est un fonds de soutien à la compétitivité agricole il est destiné à soutenir les filières en difficulté notamment en finançant de la recherche. Ce fonds n'a pas vocation à financer des collectivités ou encore des entreprises qui veulent s'engager dans cette démarche. Cependant évidemment j'entends bien l'argument que je connais bien d'Henri Cabanel et de votre groupe sur la nécessité de massifier les PSE. Ils nous aurons l'occasion de re-aborder ce sujet. Notamment au travers d'une demande de rapport un petit peu plus tard dans la discussion donc un avis défavorable. Oui, monsieur le président. Monsieur le Président Roquier. Porter c'est un moment vous présenter l'amendement de monsieur Cabanel c'est la la même position que la commission qui est une demande de retrait ou avis défavorable, si il y avait pas de retrait. D'après ce qu'on a besoin. À mon avis, d'avoir de creuser la pensée sur la question de ce que sont les paiements pour services environnementaux. On est en train de démarrer les choses, il me semble que vous avez raison madame la présidente. On va en parler aussi dans la question du carbone. Parce que c'est un service environnemental et donc on a besoin de penser le système et c'est pas très simple hein de savoir ce que c'est qu'un service environnemental. J'ajoute un. Un, un 3ème argument ici dans la chambre des collectivités en tout cas qui représente beaucoup les collectivités c'est attention à ce qu'on ne crée pas. J'entends parfois des jeunes agriculteurs qui disent qu'ils ne voudrait être adoptée par telle ou telle région parce qu'ils ont pas les mêmes dispositifs d'aide, je le dis en regardant le sénateur du plomb il verra de quoi je parle. Selon telle conseil régional ou telle autre attention à ce qu'on est pas des distorsions de clémence pour services environnementaux entre collectivités que chacun on a besoin d'avoir une définition des services environnementaux qui soit quand même un peu homogène au niveau national parce que j'imagine que sur la question DS sur la question. On pourrait dire les choses et donc on a besoin de dialoguer avec les collectivités, si voulait s'y adjoindre et on a besoin de penser globalement, ce que sont les services environnementaux sur la biodiversité parfois sur les paysages parfois sur l'eau. Parfois sur le stockage carbone parfois sur tout ça à la fois d'ailleurs, donc il me semble que c'est on a besoin d'y réfléchir et donc tels que s'est posée, à mon sens, ça ne va pas dans le bon sens et donc c'est une demande de retrait sinon un avis défavorable.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, nous souhaitons réorienter le fond prévu à l'article 3 nous semble axée presque exclusivement ça déjà été dit sur la recherche d'une compétitivité prix via l'investissement ce qui n'est pas souhaitable l'orienter vers une politique agricole qui prend en compte un véritable une véritable définition de la compétitivité dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales et sanitaires nous paraît bien entendu essentiel. Nous proposons donc de redéfinir l'objectif du Fonds associées à sa gouvernance. Le ministère de la Santé et de l'environnement et le réorienter vers la transition agroécologique des filières en difficulté et le soutien à l'agriculture biologique qui aujourd'hui ne rentre pas dans les dispositifs existants de soutien aux filières. Dans le même ordre d'idées, nous insistons pour que ces financements soient accessibles même pour les petites fermes. Celles-ci sont trop souvent exclus des dispositifs de soutien, nous proposons aussi que les montants d'aide proposées soit plafonné afin de ne pas encourager l'agrandissement des exploitations. J'entendais tout heure répéter ce qu'on entend depuis 50 ans nos fermes sont trop petites pardon nos exploitations puisqu'aujourd'hui, on exploite et on est toujours dans ce rêve ce rêve américain du toujours plus grand, avec plus de mécanisation et je pense qu'il convient d'orienter ces fonds vers une agriculture intensive en emploi et respectueuse de l'environnement et pas forcément toujours des exploitations plus importante et plus grande avec une mécanisation toujours plus fort. Si même le rapporteur. Merci, monsieur le Président, comme vient de le dire notre collègue cet amendement réoriente radicalement l'objectif du fond. Qui. Qui dans la proposition de loi est là pour soutenir prioritairement les filières qui sont en en déficit aucun type d'agriculture n'est visé par ce fonds, ce qui signifie que l'agriculture biologique pourrait tout à fait bénéficier des financements disponibles. De même, aucun type d'exploitation n'est visé en particulier ceux qui s'il finit fit là aussi que les petites exploitations ne sont pas exclues et aurait tout à fait accès à ce dispositif. À contrario, à la lecture de l'amendement, il apparaît que c'est vers un certain type d'agriculture que le fonds devraient être réorientés, nous pensons que ce n'est pas souhaitable et nous pensons que chaque agriculteur doit pouvoir être soutenu et que chaque filière doit pouvoir être soutenu qu'elles soient conventionnels ou en en biologique de plus je laisserai probablement le ministre-énumérer l'ensemble des fonds et des soutiens qu'il y a à la filière bio. je propose donc de maintenir le périmètre de l'article 3 tel qu'il est dans cette. Proposé en de loi de sortie de notre commission. C'est donc un avis défavorable demande de retrait ou avis défavorable. monsieur le président, madame la présidente, monsieur le sénateur. Même avis que la présidente rapporteur. Alors plus je vais le faire très vite d'abord sur la question. Du bio, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, qui sont des dispositifs fiscaux qui sont des dispositifs de la PAC et d'autres dispositifs. Je le dis d'ailleurs au passage, on a besoin et ça n'est pas un gros mot pour moi d'améliorer la compétitivité, y compris du bio. À la vérité. Donc le fond il viendrait. Dans cet article aussi améliorer la compétitivité. Il me semble que le sujet c'est quand même à la fois de d'essayer d'améliorer la compétitivité de toutes les filières sans exclusive. Et d'essayer de couvrir le besoin dans la variété des besoins ou des demandes de ce que sont seuls les demandes des consommateurs. J'annoncerai demain un certain nombre de mesures sur le bio qui sont en dehors du registre mais. On a besoin de conforter la filière bio mais y compris dans sa part de compétitivité. Parce qu'elle a besoin d'être le plus compétitif possible parce que sur les étals. C'est quand même sens ce que regardent les gens, la question du prix. Vous l'avez évoqué, vous-même et puis 2ème élément pardon. Faut qu'on essaye de se dire des choses sans caricature parce que. Le modèle américain, c'est pas le modèle français. La taille moyenne des exploitations en France et 66 hectares. Franchement. Allez voir mais il y a pas besoin d'aller passer l'Atlantique. Il y a pas besoin de passer le Pacifique. Allez, juste de l'autre côté des frontières françaises les plus proches et vous verrez la taille des exploitations, donc on a un modèle d'agriculture qu'on soit tous défendent, qui est un modèle qui n'est pas un modèle industriel qui n'est pas le modèle qu'on caricature et donc si on pouvait aussi ça participerait de l'attractivité du métier pardon hein. Y compris vis-à-vis des jeunes qui veulent s'installer que dire qu'on a une agriculture qui est plutôt exemplaire dans ce domaine-là qu'une agriculture qui faudrait qui a été qui a été caricaturée et par ailleurs il y a des agricultures qui souffrent des petites. Des parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Puis il y a des agricultures parce qu'on est sur d'autres types de produits et d'autres types de production qui nécessitent des exploitations de plus grande taille. Y compris d'ailleurs en élevage extensif, acceptons-le et arrêtons de rentrer les gens dans des cases en disant la bonne taille d'agriculture ça serait 66 hectares de moyenne pour les les exploitations françaises. Si vous trouvez que c'est un modèle industriel et intensif. Alors je sais pas ce que vous je, je ne vois pas comment on peut tomber d'accord. Monsieur du plomb. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, je voudrais juste revenir sur la jeunesse de cet article. Je pense qu'on s'en éloigne vraiment la réalité de cet article. C'est de revenir sur un fonds spécial pour soutenir les petites filières. De quoi parle-t-on. On parle de toutes ces petites filières qu'on a connu sur notre pays, qui ont fait parfois le bonheur économique et l'équilibre des exploitations, souvent des petites parce que souvent diversifiée et qui au final par le dogme que vous développez commence de disparaître. J'en prends une, oui, oui votre dogme j'en prends une, celui de la moutarde. On sait. Tous s'offusquer de ne plus trouver de moutarde dans les étalages.

Pourquoi y trouver plus de moutarde de Dijon parce que votre dogme a fait qu'année après année, on a interdit toutes les mesures possibles pour cultiver de la moutarde en Côte d'Or. Ce qui a fait qu'au bout du bout, les agriculteurs se sont détournés de cette culture en fait que ils ont arrêté de produire de la moutarde en France ce qui a fait qu'on s'est jeté dans les bras des Canadiens dans un 1er temps et après des Ukrainiens pour trouver la même graine de moutarde. Alors que la réalité et l'objectivité et le bon sens aurait été de ne moins interdire de laisser la possibilité aux agriculteurs de faire leur travail et on aurait tout ai toujours trouver de la moutarde de Dijon et française. Concernant l'agrandissement. Concernant l'agrandissement il suffit de regarder les trajectoires effectivement. Depuis des décennies les tailles s'agrandissent, même si on est peut-être à 66 en moyenne. vous savez ce que c'est qu'une moyenne, la moyenne ça cache beaucoup de diversité et il faut vraiment regarder les choses avec un peu plus de détails. Non non mais je vous ai écouté. La compétitivité dont vous me parlez, et vous savez que la compétitivité le prix il y a une relativité effectivement parlait du bio qui devrait être compétitif. Eh bien il est le bio compétitif il est si on fait payer à l'autre agriculture ses externalités négatives effectivement il paraît plus cher comme ça à partir du moment où c'est le contribuable. C'est la collectivité qui paye in fine et tout les externalités négatives et tous les problèmes d'eau, les problèmes sanitaires liés à un type d'agriculture, effectivement on est moins compétitif. Mais il y a une relativité de la compétitivité. J'aimerais bien qu'on. Ici on l'entende. À un moment parce que ça me semble fondamental de ne pas externaliser toujours les coûts vers le contribuable.

vient en complément de ce qu'a dit mon collègue concernant les les externalités négatives. Il se trouve qu'en 2014 on a on avait demandé au ministre Le Foll. Que soit menée une étude justement pour évaluer les externalités négatives. Cette étude a été a été menée partiellement par l'INRA table je crois savoir, Monsieur le Ministre. Mais vous le savez mieux que moi. Cette étude est reprise. Alors ma question sera une fois qu'on aura véritablement les chiffres je crois savoir que pour l'eau c'est de l'ordre de 1 milliard à un milliard 5 chaque année, la réhabilitation de la qualité de l'eau sur les questions de pesticides et de nitrates. Une fois que l'on aura ces chiffres là que pour le la quantification par rapport aux pollinisateurs également parce qu'il y a un rôle économique. On sait que les pollinisateurs vont mal par au regard d'une certaine d'une certaine agriculture. Une fois qu'on aura tous ces chiffres là, comme le disait Daniel Salmon, non seulement les produits bio seront à égalité mais ils seront moins chers que les produits

de monsieur l'abbé. Oui, monsieur le président. Chers collègues cet amendement vise à alerter le gouvernement, Monsieur le Ministre sur une problématique aujourd'hui complètement orpheline des politiques publiques en effet chaque année des centaines de milliers de tonnes de production agricole sont détruites ou déclassés du fait de contamination phyto- sanitaires due à l'épandage d'un pesticide sur une exploitation voisine et ce, sans qu'aucune indemnisation du producteur concerné ne soit possible. Rappelons que certains produits phytosanitaires, notamment l'herbicide prosulfocarbe ont une volatilité sur des kilomètres. Ainsi, dans le cas de ces contaminations bien souvent le responsable ne peut être identifié. Or le régime de la responsabilité civile qui implique que la personne responsable de la contamination soit identifié est le seul dispositif permettant à ce jour une indemnisation. Cela laisse sans solution. Les agriculteurs et notamment les producteurs bio qui sont particulièrement concernés, cela pénalise des filières toute entière et notamment la filière sarrasin bio en cours de structuration. On a des producteurs bio qui s'engage pour mettre en oeuvre des pratiques sans pesticides mais subissent à leur frais de déclassement et destruction de de production du fait de l'usage autour de de produits phytosanitaires. Et les producteurs bio ne sont pas les seuls concernés l'ensemble de la filière cidricole est également touchée par cette problématique. Cette situation génère des difficultés humaines économiques et elle doit cesser c'est pourquoi cet amendement propose de mettre en place un système d'indemnisation pour les producteurs, victimes d'une contamination par un produit phytosanitaire. Dont le responsable ne peut être identifié. Merci madame la rapporteure. Oui, chers collègues, la question de que cet amendement soulève est plutôt de la politique d'indemnisation des assureurs, ainsi que du bon dialogue entre les agriculteurs eux-, même en cas de contamination d'une parcelle bio. elle est un peu décalé par rapport à la vocation de ce fonds qui est mis ici en place pour soutenir les filières, notamment sur la recherche. C'est donc une demande de retrait ou un avis des. Demande de retrait ou avis défavorable pour exactement les mêmes motifs. Qui a évoqué la présidente Prima. J'ajoute que sur les questions de compétitivité j'voulais le dire tout à l'heure il qu'on a un certain nombre de dispositifs qui vient qui viennent a accompagné les filières. Ce qu'on a fait sur les fruits et légumes ça vient aussi encourager d'ailleurs la filière bio sur un certain nombre de secteurs et ça n'empêche pas la question que vous posez qui est une réelle question mais qui ne me paraît pas correspondre à ce qui le d'esprit de l'article 3 de ça relève plutôt du système assurantiel des pratiques entre agriculteurs, me semble-t-il étroit du PLF, donc c'est un avis défavorable. Et d'abord une une demande de retrait Oui mais ils ont tenté de se retourner vers leurs assureurs. Mais les assureurs ne prennent pas du tout en compte, mais parce que de toute façon ces volatiles, ça peut être à 3 kilomètres en fait sur le fond cet herbicide prosulfocarbe il faudrait qu'il soit interdit. Selon le ministre, vos relations avec. Vous pouvez leur demander de revoir leur. Leur autorisation de mise sur le marché. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 29. Madame Filleul. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre. Cet amendement vise à ce que la gestion du fonds spécial de soutien à la compétitivité filières agricoles en difficultés intègre un objectif de parité, on est fait de nombreuses femmes agricultrices rencontrent des difficultés pour obtenir un crédit bancaire soit pour lancer leur exploitation agricole soit pour réaliser de nombreux investissements peut représenter moins payé parfois même pas compter les femmes sont les grandes oubliées de nos politiques agricoles. Le ministre, le ministre de l'agriculture estime que les femmes représentent 30% des actifs agricoles en France en France plus nombreuses dans les petites structures, les femmes sont aussi plus diplômés et plus âgés que les hommes. Pourtant, leurs revenus sont quasiment un tiers plus faible et leurs retraites atteint péniblement 750 euros par mois dans l'agriculture. Les femmes font face à des inégalités multiple de revenus d'accès au foncier à l'investissement aux aides et aux formations de charges domestiques, les politiques sectorielles n'enraye pas voir renforcer ces inégalités de gens la très faible disponibilité des données genre et et d'ailleurs un frein au traitement des inégalités entre autres bâtons dans les roues, les agricultrices bénéficient de prêts bancaires plus faible de moins d'aide à l'installation et elles sont moins représentées dans les syndicats professionnels, à l'instar des dispositifs existants déjà dans d'autres secteurs où à travers l'action de la banque publique d'investissement. Il convient donc d'instaurer dans le fonds spécial de soutien à la compétitivité filières agricoles une proportion minimale de bénéficiaires par sexe. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président, je comprends l'objectif qui est poursuivi par Madame Préville qui est celui de féminiser l'agriculture et et d'avoir un accès équitable aux dispositifs de soutien et d'aide mais je voudrais dire que le fonds de soutien vient en aide à des exploitations mais il vient aussi et surtout en aide à des filières par l'intermédiaire de financement aux instituts techniques par exemple ou encore des appels à projets donc il semble difficile pour ne pas dire impossible, de faire la liste des potentiels bénéficiaires d'une mesure de soutien pour s'assurer de la juste représentation des femmes un soutien par exemple à la recherche de solutions pour lutter contre la drosophile a Suzy Quick, tout le monde connaît bien ici qui infecte la cerise. Sera un soutien non pas un exploitant mais une filière, il est donc impossible de calculer le nombre de femmes qui bénéficient de ce soutien. Je vous demanderai donc devant l'impossibilité d'appliquer cet amendement de le retirer, sinon ce sera un avis défavorable. Même avis, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président. Même avis que la présidente. Madame la sénatrice. En fait vous poser de question et je pense que l'amendement ne vient pas répondre à la question principale qui est celui de. d'une plus grande féminisation de la profession agricole, là on est sur un. Un, un article qui vient. Assumer l'idée de compétitivité des filières et comme l'a très bien dit par son exemple la présidente. C'est c'est pas une question de genre. C'est une question de filière. Ça n'obère pas ce que vous dites par ailleurs et donc d'une certaine façon fait ce qui est assez original dans un texte qui vise à supprimer les sur-transpositions fait une surtransposition d'ailleurs dont on ne saurait pas comment la mettre en oeuvre. Ce qu'on fait avec ce qu'est la structure de la filière aujourd'hui en revanche, je partage votre sentiment. Ça n'est pas qu'un objet d'ailleurs de genre mais c'est un objet de d'origine de jeunes qui veulent s'installer, il faut qu'on arrive par les questions du portage du foncier c'est évoquer un peu dans le texte qui vous est soumis, et ça c'est le travail que nous faisons dans l'APA lois qui sont du portage du foncier, la perception de portage des capitaux, c'est souvent un franc. Pour des femmes, pas que pour des femmes et aussi pour des femmes et notamment pour des femmes à l'accès. Au statut de d'exploitants agricoles, donc ça on a besoin d'y travailler. Mais cet amendement il ne vient pas répondre à ça en fait et donc par rapport à la question de la compétitivité. Disons que il faut qu'on le regarde différemment et plutôt dans l'accès aux moyens de production au foncier aux capitaux au siège d'exploitation à la filière et c'est comme ça qu'on arrivera à féminiser cette filière reconnaissons aussi que je crois que l'enseignement agricole. Et. En majorité aujourd'hui féminin dans toutes les femmes qui sont les les femmes ou les jeunes femmes qui sont inscrits dans l'enseignement quoi donc à terme. à terme, compte tenu du fait qu'on a plutôt d'ailleurs une majorité de gens qui ne sont pas issus du milieu agricole la féminiser la féminisation fera son oeuvre, on a un travail à faire pour la facilité, mais c'est une demande donc de retrait, sinon c'est un avis défavorable. Merci, elle est maintenue.

Mais vraiment choqué. Parce qu'aujourd'hui, ça serait intéressant. Vous nous donniez un cas. Une agricultrice. Le seul pays d'ailleurs à à travers l'Europe. Qui a obtenu qu'une femme puisse devenir agricultrice, comme son mari. C'est comme ça qu'on a fait les ORL parce qu'à l'époque les GAEC entre. Mari et femme n'était pas possible. Le seul pays qui a, qui l'a fait, c'est la France. Seul pays qui a fait évoluer GEC puisque maintenant on peut faire un GAEC entre époux, c'est la France. Quand un dossier est examiné au niveau financier, comme vous l'évoquez dans votre amendement mais jamais on traite un dossier sur un projet par rapport au sexe de la personne, c'est le projet de d'installation, c'est le projet d'investissement. Oui, je dis ça, excusez-moi de m'emporter un peu parce que quelque part en se comportant de cette manière-là, ben voilà comment on détourne des femmes et des hommes de se lancer dans la profession agricole. Personne n'a jamais été abordé d'une manière par rapport au sexe de l'individu, c'est toujours le projet qui l'a emporté et je pense que beaucoup de professions devraient copier ce qui a était venu vous l'agriculture. Voilà ce que je voulais dire. Merci cher collègue. Oui madame Maria. Je me permets de vous répondre parce qu'effectivement. À la délégation aux droits des femmes. Nous avons été 8 rapporteur des territoires ruraux à rendre un rapport sur la situation des femmes dans la ruralité et je puis vous dire qu'à cette occasion, moi j'ai beaucoup auditionné comme mes autres collègues des agricultrices des cette profession, c'est un fait Leur réflexion a été récurrentes, elles ont oui des difficultés pour obtenir des emprunts. Oui c'est vrai c'est une réalité et je puis vous dire Je n'ai pas été la seule mes collègues rapporteurs qui n'étaient pas forcément d'ailleurs du même obédience que moi l'ont constaté, elles ont des difficultés à obtenir des emprunts, c'est vrai. Merci cher collègue. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 29 avec 2. Monsieur Boyer. Oui, merci Monsieur le Président. C'est c'est un peu surprenant d'entendre un débat comme ceci ou. Quelque part, on stigmatise. Les femmes à travers la profession agricole. Le peu le peu le peu d'expérience que j'ai pu avoir comme enseignant dans l'enseignement agricole où j'ai vu de nombreuses filles donc et femme s'installer dans le domaine agricole mais qui est bien souvent avaient d'une famille et des parents qui agriculteur et donc elle savait un projet et les aides lorsqu'elles sont demandées pour une installation, elles ne sont pas faits en fonction du sexe. Sont faites en fonction du projet. S'il y a un projet qui tient la route, effectivement les femmes elles ont leurs aides exactement de la même manière comme un homme peut l'avoir. a on a aujourd'hui dans l'enseignement. Beaucoup de de jeunes. Qui par rapport à 10 ou 20 ans où on avait une population dans les lycées qui étaient avec des élèves qui venait de de profession agricole avec des parents agricole aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez peut être. À peine 15 20 d'élèves dans l'enseignement agricole qui sont d'origine agricole avec des parents qui sont agriculteurs, qui ont donc un projet de transmission aujourd'hui ce n'est plus le cas et si vous présentez un projet où vous n'avez pas effectivement les moyens financiers de pouvoir subvenir au fonctionnement de votre exploitation. C'est là qu'il y a des des difficultés et qu'il faut essayer de trouver des solutions, mais ce n'est pas en fonction du sexe de la personne. C'est en fonction du projet. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mais on voit l'article 3 qui est pour l'article 3. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Un article additionnel l'amendement 30, Monsieur Montaugé.

Le modèle économique des exploitations agricoles, donc en zone intermédiaire est aujourd'hui à bout de souffle depuis des années, les années 80. Ces exploitations ne cesser de s'agrandir. Alors moi je, c'est un constat hein c'est pas un jugement de valeur et de se spécialiser tout toujours davantage un gramme de culture entre 88 et 2010 le nombre total d'exploitation a été divisée par 2 le nombre d'exploitations avec vaches laitières a divisé par 5 et le nombre de vaches allaitantes divisé par 2,5. Cette hyper spécialisation pose de nombreuses difficultés. Ces exploitations ont ainsi un problème structurel de rentabilité avec des productions à faible valeur ajoutée leur forte dépendance aux marchés mondiaux du fait de leur caractère de monoculture les rames très sensible aux aléas économiques et peu résilientes, parallèlement, elles sont très dépendantes des aides de la PAC qui ne suffisent plus à leur survie. Les terribles Roger n'ait été agronomique et pédo-climatiques de la SAU française justifie la proposition et la mise en oeuvre de dispositions de politiques agricoles nationales permettant de soutenir de façon ciblée les territoires de plus en plus en difficulté au regard de critères de performances agro-environnementales sur certaines de ces territoires des mecs spécifique. Sont une première réponse mais les écarts de performance et du rémunération. Reste très élevé, donc ça ne préjuge préjudice des acteurs de la politique agricole commune. le rapport. Pourrait consister à à proposer une définition. De ce que, de ce que sont les zones intermédiaires et et proposer des politiques. Territoriales pour rétablir l'équité entre entre terroir français dans le sens de ce que vous avez indiqué, Monsieur le Ministre d'un vote. Oh dis merci Si Monsieur le président, Monsieur Montaugé. Chers collègues, je connais votre engagement pour ces zones. Intermédiaires à faible potentiel. Vous savez que nous n'aimons pas beaucoup les rapports on a déjà de rapports dans ce texte, on essaye de de garder ce qui nous semble l'essence. Même la problématique du soutien à l'agriculture en zone intermédiaire à faible potentiel et très documenté, elle est dans un rapport du CGER de janvier 2019 elle est d'ores et déjà largement traitée dans le programme stratégique national français qui fait pour sa part 975 pages donc je je crois que ce ce ce sujet et. Tout à fait connu et documenté et je crains qu'un rapport ne suffisent pas. À à régler les soucis qui qui sont ici, il y a différentes mesures agro-environnementales et climatiques ont été adaptés mais je préférerais. Qu'on passe du rapport à l'action. J'ai passé, du coup la parole au ministre. Et je donne un avis défavorable sur ce rapport en en considérant quand même que c'est un sujet très important. Merci, monsieur le Ministre.

Qui donnerait une balle les législatives un zonage alors. On sait en agriculture ce que c'est que la question des zonages, on rentre dans une machine d'abord dans un. Sur un sujet comme celui-là, dire qu'on peut dans la loi définir ce qu'est une zone intermédiaire. D'abord, courage et de ça sera l'objet de demandes conventionnel partout parce que ce que vous avez dans le Gers n'est pas la même chose que ce que j'ai. Dans le Berry, au sud de ma région où les difficultés sont pas de même nature. Il y a des questions parfois d'accès à l'eau, il y a parfois des questions de potentiel agronomique a question des parfois des questions de modèle agricole. S'enfermer dans une définition législative. C'est un peu parfois le mal français de la rigidification. Et donc on a plutôt besoin de regarder, territoire par territoire. Les mesures qu'on peut avoir, vous avez évoqué les les mecs qui peuvent être une première réponse. Ça c'est des outils de compensation mais on a besoin aussi de penser et c'est tout l'objet du travail qu'on aide doit on être la faire la la transition de ses modèles. La question n'est pas de compenser. La difficulté dans laquelle il se trouve seulement la question c'est de dire quel est le modèle sur lequel c'est ces types d'agriculture dans ces zones intermédiaires pour fonctionner. Donc je rejoindrai assez volontiers ce qu'a dit la présidente Prima. On a besoin de regarder les mecs. Et au-delà des mecs. Quelles sont les mesures de soutien qu'on peut apporter au delà des zonages parce que la contrainte. Climatique, elle n'est pas la même aujourd'hui qu'elle n'était il y a 10 ans il n'est pas la même aujourd'hui qu'elle ne sera dans 10 ans et donc on va pas faire évoluer à ce à ce degré-là les choses on a besoin plutôt d'essayer d'engager des agriculteurs dans cette transition. C'est vrai que dans certains cas, la réponse a pu être l'agrandissement. Et c'est vrai que dans, dans certains cas maintenant la réponse ne peut plus être l'agrandissement ce qu'veut au contraire ça vient aggraver parfois la situation économique, il faut se le dire en lucidité aussi. Mais parfois c'est la réponse parfois ça l'est pas. C'est mon côté vous voyez. Pas caricaturale monsieur seulement c'est peut-être qui parfois fait nos débats entre nous, j'essaie de trouver un point d'équilibre et donc c'est ça qu'il faut qu'on trouve mais c'est plutôt des mesures que des zonages ou des rapports donc c'est un avis, une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci monsieur

des des des intentions. Et d'autant plus quand on peut les les les partager. Mais moi ce que je constate c'est que lors de la de la discussion de la PAC. Lors de l'élaboration du PSN. Ce genre de sujet n'a pas été abordé en tout cas à la mesure qui est la sienne, qui est, qui est effectivement celle de la transition que vous appelez de de de vos voeux et et sur laquelle on est on est on est tous d'accord. Voilà, on va encore perdre des années par rapport à ces zones à moins que vous proposiez effectivement dans le cas du du PSN. Des actions spécifiques particulières, je, je peux vous dire que les mecs qui existe en rapport avec ses, ses terroirs apporte des choses mais c'est absolument pas à la hauteur des enjeux de transition que vous évoquez. Voilà et sur lesquels on on est d'accord qu'il faut mener une action rapide et efficace. Voilà donc je. Pour ces raisons là je je maintiens cet amendement tout en comprenant. Notamment les les arguments de Madame la rapporteure. Je vois l'amendement 30 avec 2 avis défavorable qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté à l'article 4 3 amendements discussion commune de 105, monsieur l'abbé. Utiliser l'épargne pour soutenir l'agriculture, c'est une bonne idée. Maintenant ce livret A gris pour nous ne nous convient pas les subventions à l'investissement en agriculture sont déjà massive entre France relance France 2030. PCAE suramortissement. C'est la Cour des comptes qui l'indique. Ces subventions sont beaucoup trop importantes et freine l'installation de nouveaux agriculteurs ces mécanismes. Peuvent aussi conduire à du surendettement et à l'agrandissement excessive des exploitations. Phénomène hélas bien trop courant en agriculture. De plus, ces incitations à l'investissement sont majoritairement orienté vers une forme d'industrialisation de l'agriculture. À rebours de la nécessaire prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux mais aussi des attentes de nos concitoyens. Et on nous propose avec cet article de mettre l'épargne des Français au service de cette industrialisation de l'agriculture. Quant à nous nous proposons de cibler ce dispositif est rebaptisé ce livret Livret A mais agro-écologie ils viendraient financer uniquement l'installation dans des systèmes en agro-écologie. Ou en bio de façon encadrée par un cahier des charges. Nous ne souhaite en aucun cas venir ajouter une incitation de plus pour les agriculteurs assure investir au détriment de la viabilité économique de leur ferme et de la transition agroécologique.

La création d'un livret A Green est en effet pas une nouveauté, et a déjà été évoquée dans le passé dans plusieurs textes agricole sans pour autant jamais voir le jour en 2015 et 2016, il avait ainsi été adopté au Sénat sous la forme d'un livret Vert dans le cadre d'une proposition de loi là aussi portant sur la compétitivité agricole. Cette proposition a toujours été rejetée pour divers motifs. Je tiens d'ailleurs à rappeler à mes collègues du groupe Les Républicains qu'en 2015 lors de l'examen de ce texte, c'est bien l'un de vos anciens collègues. Antoine Herth alors rapporteur et membre du groupe et un UMP qui, je le cite, s'interroger sur l'utilité d'une telle mesure. Avant d'ajouter que l'épargne des Français n'est pas extensible et le fléchage de l'épargne sur ce livret ne se fera qu'au détriment d'autres produits d'épargne. Donc en tout état de cause, si nous nous interrogeons également sur la pertinence d'un tel outil. Nous proposons toutefois dans un esprit constructif que les ressources collectées par les établissements en distribuant le Livret A gris soit employé au financement des investissements des structures agricoles et agroalimentaires sous signe de qualité ou en agriculture biologique. Nous estimons en effet que se livrer, s'il venait à voir le jour devra accompagner la transition vers l'agro-écologie et le soutien aux productions de qualité bénéficiant de signe ou d'une mention reconnu. Merci cher collègue le. 3 58 Madame Barilla. Merci monsieur le prix. Avec ce livret A gris. Vous souhaitez réorienter l'épargne populaire vers l'agriculture afin d'en améliorer la compétitivité voir la mécanisation. notre point de vue. Ah nous c'est que ce livret à gris doit permettre de financer la transition de notre modèle agricole. Vers une agriculture durable et permettre de faire face au changement climatique, c'est l'urgence et c'est de cette urgence à laquelle nous devons tous faire face comme le souligne le rapport de la commission. L'agriculture ne souffre pas d'une insuffisance majeure de financement puisque l'on constate que les encours d'emprunt progresse d'un air d'année mais elles souffrent pour de nombreuses exploitations d'un surendettement qui fragilise l'installation des agriculteurs et ce surendettement quelques fois il est dû à un sur-équipement si l'aide à l'installation des agriculteurs est une bonne chose. Il ne demeure pas moins que le vrai problème reste le renchérissement du coût du foncier et le risque est grand de voir se livrer à gris accompagner l'augmentation du coût du foncier, alors même que si dans un encadrement et dans une et et de régulation dont nous avons besoin pour lutter contre la pression de plus en plus forte de la part d'investisseurs ni armes d'ailleurs souvent rien à voir parfois pas souvent mais parfois rien à voir avec l'agriculture et même parfois étrangers en fin, comme le rappelle le réseau Solidarité paysans tout pour ses agriculteurs à investir les revues et salons spécialisés valorise à outrance une technologie sation, signe de modernité de performance mais aussi d'appartenance à une profession n'est pas forcément un marqueur social de réussite sur le plan fiscal ils sont encouragés à investir pour payer moins d'impôts, moins de cotisations sociales. Or le surinvestissement peut rendre une exploitation vulnérables et devenir un frein pour la transmission. C'est pourquoi nous pensons que telle qu'il est rédigé cet article le quatre. Il est à rebours de la nécessité de redonner de l'autonomie aux ferme et limiter les dépendance à l'égard merci. Merci monsieur le président je ne résiste pas à l'envie de faire, rendre hommage à la PPL de notre ancien collègue le noir qui est à l'origine. Effectivement de cette idée de création d'un livret agricole qui a pour but non pas de conduire au sur investissement mais de créer un lien entre les Français et l'agriculture car. Il est très important dans la relation entre les Français et l'agriculture de recréer ce lien. Alors cette ces amendements qui sont identiques dans leur finalité mais différents dans leur forme ou pour but de réorienter l'objet du Livret A gris et de réduire les financements soient à l'agriculture biologique ou en agro-écologie, c'est l'amendement de notre Cowell collègue Joël Labbé soit aux exploitations qui qui sont sous signe de qualité ou en bio. C'est complètement contradictoire avec l'objectif général d'aider l'ensemble des agriculteurs de ne pas opposer les agricultures les unes aux autres. Une fois de plus et d'aider de façon indifférenciée, l'ensemble des agriculteurs je voudrais noter que nous avons rajouté dans les investissements éligibles les investissements immatériels qui sont trop souvent oubliées et qui sont pourtant des investissements qui permettent justement d'éviter des mécanisation trop forte et d'aller. De, d'aller vers des agricultures de précision et je voudrais également dire que nous avons permis d'inclure la question de l'accès au foncier agricole aux jeunes agriculteurs,

il fait disparaître le mot de compétitivité qui dans le cadre de cette proposition de loi serait pour le moins incongru. Vous l'avez compris, c'est un avis défavorable sur ces trois amendements. Merci, monsieur le Ministre. Oui, monsieur le Président. Madame et messieurs les sénateurs, madame la rapporteure. D'abord dire l'intérêt pour nous de l'article IV quand même. Au passage.

Et donc d'améliorer et d'essayer d'améliorer la compétitivité, telle est l'objet d'ailleurs de cette proposition de loi. Et puis la 2ème intérêt qui n'est pas des moindres, y compris dans la réflexion que nous menons sur le Pacs, c'est de mieux connecter la société avec l'agriculture. C'est-à-dire que les français portent une part donc il y a une question de dialogue avec la société dans cette affaire-là. Et dans cette volonté que l'épargne des Français viennent servir l'agriculture et donc je le dis, cet article 4, il nous paraît intéressant. Dans le débat qui se poursuivra des attendus, y compris de la loi d'orientation, c'est des éléments qui remontent beaucoup. Des débats que nous avons eu en région au niveau national, d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qui est présenté dans cette PPL non je voudrais d'abord souligner l'intérêt de cet article 4 dans ses 2 composantes compétitivité dialogue entre la société et ses agriculteurs 2ème au Liban, on le voit bien d'ailleurs dans les trois amendements successifs. Ils sont pas de même nature pour les uns, c'est le bio pour les autres c'est le bio. Les circuits courts, les signes de qualité pour les troisièmes. C'est la question de l'investissement. Ça prouve quoi. Ça prouve qu'on a besoin de continuer à travailler sur ces sujets-là c'est pour ça que c'est plutôt une demande de retrait à défaut un avis défavorable sur les amendements eux- mêmes parce que je pense qu'on a besoin de qualifier les choses, on a besoin d'engager tout le monde, c'est vrai qu'on a besoin de penser ces systèmes d'épargne en disant, qu'est ce qui permet d'engager la transition parce qu'on ne peut pas dire on veut la transition est pas en donner les moyens il me semble que les rédactions qui sont proposées. Donc je me dois de le dire, ne correspondent pas tout à fait à l'idée qu'on se fait de la question de la compétitivité. Il y a la question des jeunes, vous avez évoqué, madame la sénatrice, à juste titre. La question du surinvestissement. Alors c'est à la fois je ne sais pas tellement le sujet de l'article 4 à mon avis, c'est une question les questions fiscales qu'il faudra poser globalement, qu'est-ce qu'on a comme dispositifs fiscaux qui améliore la transition qui permette de répondre à ce que disait le sénateur Montaugé sur les zones intermédiaires mais l'article 4 il vient plutôt essayer de renforcer non pas le surinvestissement mais de le portage de capitaux, de faire en sorte que le foncier de faire en sorte que des jeunes sans distinction du modèle dans lequel il s'installe à ce que le sujet principal c'est un sujet de renouvellement de générations et donc pour tous ces motifs, c'est une demande de retrait des fois un avis défavorable mais favorable à l'idée, je le dis très volontiers que nous travaillons sur ce sujet-là dans le prolongement à la fois l'article IV et de la manière dont on l'oriente pour face favoriser ou encourager au transition.

avoir qui qui devrait être celui qu'on n'aurait jamais dû perdre entre les Français et leur agriculture. Parce que le modèle français de distensions entre la population et l'agriculture, il n'est pas vrai partout. Nous avons été en Italie et nous avons vu la différence avec les Italiens. Aujourd'hui les italiens sont 57 millions d'ambassadeurs des produits italiens, nous en France on a 30 millions de procureur de l'agriculture française. Et quand on écoute ce qu'on vient d'entendre à travers les bancs et en particulier. Le groupe communiste. Mais c'est des messages qui sont d'arrière-garde. Aujourd'hui il y a plus d'agriculteurs qui font le plaisir d'investir pour le plaisir d'investir ben. Là le sur le suramortissement, certes peut être un élément fiscal. Mais aujourd'hui regarder la réalité des exploitations. Il y a pas une exploitation qui achète pas au cumin. Il y a une pas une exploitation qui se regroupent avec une autre pour acheter du même matériel parce que tout simplement les différences de prix font qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus se payer le luxe d'acheter des tracteurs pour le plaisir d'acheter des tracteurs. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il peut y avoir entre, il y a 10 ans et aujourd'hui il y a 10 ans pour changer 3 tracteurs sur mon exploitation c'était 80.000 euros de Soultz entre les anciens et les nouveaux aujourd'hui c'est 240.000 euros. Vous pensez que les agriculteurs font plaisir à acheter des tracteurs pour simplement le plaisir de défiscaliser d'acheter des tracteurs. C'est plus du tout ça c'est terminé tout ça. Il faut sortir de ce message-là, donc au contraire le livret hein peut être la possibilité pour les Français de reprendre par message de l'agriculture mais aussi ça pourrait être à l'avenir peut être les solutions pour retrouver des choses qu'on a abandonné trop vite quand on parle tous d'installation de renouveler les générations et ce que demain il ne faudra pas remettre en place des prêts bonifiés, quand les taux d'intérêt passe de 0 il y a encore quelques mois à 4% aujourd'hui et que le Patrimoine d'une exploitation à transmettre. Faire une somme colossale de capital. Il faudra peut-être le faire à travers le. le monsieur le président. Effectivement j'entends bien ces aides doivent être indifférencié doivent être large, hé bien non, nous effectivement on a des préférences. On estime qu'il y a des modèles qui sont plus vertueux que les autres alors c'est ça qui nous différencie. On nous dit qu'on ait caricaturaux. Non, simplement on a des convictions et on pense qu'il y a des modèles qui s'inscrivent dans une vraie transition et qui vont nous amener de la résilience et on veut aider ces modèles-là tout simplement et ça me semble limpide. Une politique publique ça sert à orienter l'agriculture donc nous voilà on veut orienter d'une certaine manière, on n'est pas d'accord, mais effectivement ça se justifie avec nos. Notre vision qu'on a de l'agriculture. Alors je simplement répondent à. Vos collègues Laurent Duplomb sur la moutarde. Il a fallu le temps qu'elle me monte un peu au nez mais voilà. Je reviens sur la moutarde effectivement votre moutarde. Eh bien ces 2 modèles totalement différents. Vous nous parlez d'un modèle ouvert libéral où on est en concurrence avec les Ukrainiens sur la moutarde et vous nous dites, hé bien pour être compétitifs avec les Ukrainiens. Hé bien on s'assoit sur nos normes environnementales et puis on essaye d'avoir le le coût salarial le plus bas. Donc vous êtes dans ce dans cette dynamique-là d'un marché libéral qui a été défendue depuis des décennies et ça se justifie. Eh bien nous effectivement on n'est pas dans ce. On ne veut pas rester dans ce cadre-là, on veut des clauses miroirs on veut de faire en sorte de protéger notre agriculture et de protéger par là-même notre environnement et la santé des Françaises et des Français et de maintenir un monde habitable. Voilà notre différence, c'est une différence macroscopique. Effectivement c'est une défense d'économie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais. À mon tour défendre ses amendements comme vient de le faire. Mon collègue Daniel Salmon en soulignant que puisque l'enjeu, c'est au fond par ce livret A gris de créer un lien entre la société et les agriculteurs. Prenons exemple sur ce qui se passe avec le livret du développement durable, qui n'a de développement durable souvent que le nom et qui du coup n'incite pas un grand nombre de nos concitoyens qui souhaitent soutenir une transition à s'engager sur ces produits financiers. Donc je crois qu'il serait très sage d'avoir un livret A gris qui viennent soutenir la transition écologique et qui permettent à nos concitoyens qui souhaitent soutenir cette transition, de s'engager avec confiance sur ce produit financier et sur ce soutien un nouveau modèle agricole ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'ailleurs d'avoir un livret A grille conventionnelle pour ma part, j'ai pas de sujet. Par contre je pense il y a un sujet de clarté et croire qu'on veut soutenir tous les modèles agricoles ne me paraît pas correspondre à la réalité des points de vue de beaucoup de nos concitoyens qui souhaitent participer face à la gravité de la crise climatique face au danger lié à la pollution et au modèle agro-industriel. Il souhaite participer activement à cette transition agroécologique permettons le. madame la rapporteure. et de son aveu ou en tout cas de son. Témoignage en tout cas ils financent. Directement par cette plateforme en ligne de collecte de fonds beaucoup de projets agricoles dans leur totale diversité, donc je pense que il faut être tout à fait neutre par rapport. Au projet d'installation, notamment des jeunes qui sont souvent financées par ces plateformes permettre au Livret A d'être très large dans son dans son n'éligibilité et c'est une différence idéologique Monsieur Salmon et effectivement mais nous l'assumons pleinement. Pardon. Merci Monsieur le Président. Juste un mot. Un petit pas de côté par rapport à ce que ce que ce qu'il y en ait dit sur. On peut, on peut à la fois essayer de regarder ce qu'on fait, comme transition et puis aussi on a un besoin dans cette PPL de répondre à des besoins de compétitivité. Et de produits qui manquent. Moi il me manque des éleveurs en novembre. Il me manque pas, des éleveurs en au vin bio, il me manque des éleveurs en ovins parce qu'on ne pouvait pas à la fois dénoncé le fait qu'on aille chercher des ovins à l'extérieur. Des frontières. Et dire non moi je prends que les bio Et vous savez comme c'est des marchés qui sont compliqués. J'ai besoin de reconquérir 60% quasiment de la filière fruits et légumes et de répondre à l'ensemble des besoins. Des consommateurs français qui sont parfois du bio parfois autre chose.

D'avoir besoin de l'ensemble des modèles ça veut pas dire que c'est là ma petite différence avec l'expression qui avait la présidente Prima. Je pense qu'on a besoin d'encourager les transitions mais on a besoin aussi de reconquérir notre souveraineté sinon on parle dans le vide parce qu'on peut toujours dire on veut ça et ça, si ce n'est pas ce que les gens consomment. Ça n'empêche pas de faire les transitions mais si ce n'est pas ce que les gens consomment à la fin ça vient de l'extérieur parce que l'exemple de la moutarde et bon parce que à la vérité si je vous écoute monsieur. Vous vous proposez non seulement qu'il y ait pas de moutarde en France mais qui est pas. Tout court. Parce qu'à la fin si je pousse votre raisonnement vous dit je n'accepte pas les produits du Canada mais comme on a du mal à produire aujourd'hui dans les conditions actuelles de la moutarde en France à la vérité, c'est ça, c'est pour ça qu'on en produit plus c'est même pas une question de compétitivité hein c'est même plus une compétition compétitivité sur la c'est qu'on ne sait pas le faire Essayons, essayons de le comprendre et si on ne le documenter sait-on de trouver des solutions parce que je ne me résous pas à ce qu'on n'ait pas de moutarde. En France, je ne me résous pas non plus à ce que les Français n'aient pas moutarde. Je préférerais qu'il faisait de la moutarde en France. Merci monsieur l'abbé. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de transition. Ça va dans le sens des 3 amendements qui vont véritablement dans le sens de la transition. Ah il ne s'agit, il ne s'agit que d'épargne populaire dans le cadre d'un Livret A.

avant la la prochaine loi votre prochaine loi si un, un à un, une consultation. Populaire et citoyenne était menée pour savoir si nos concitoyens souhaitent financer un Livret A ou un Livret agroécologie. Voilà ça et sans opposer. On sait que si c'est un livret agro-écologie il y aura beaucoup plus d'entrain pour y aller et c'est pas voilà je. Merci, cher collègue, Monsieur Montaugé. merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. J'ai, je suis un peu surpris de votre propos concernant la moutarde je je vous invite à goûter celle de Don trace. Le berceau de l'Armagnac une excellente moutarde.

je mais aux voix l'amendement 105 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté même vote pour le 31. Même vote il n'est pas adopté même votes pour 58. Il n'est pas adopté. On passons 123 de la commission, madame la rapporteure. Attends. Rédactionnelle avis favorable, Monsieur le Ministre donc je mais on voit le 123 de la commission avec un avis favorable du gouvernement. C'est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté, je mais aux voix l'article 4 qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient il être adopté à l'article 5, une prise de parole de monsieur Tissot. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 5, nous amène à travers un crédit d'impôt à aborder la question de la mécanisation en agriculture. Sur le fondement de cet article. Nous ne sommes bien sûr pas favorable à la création d'un nouvel. Crédit d'impôt. Toutefois la écriture de la rapporteure avec un plafond nous paraît un peu plus raisonnable et c'est pour cela que nous nous trouvons pas de nous ne proposerons pas de suppression de l'article. Pour revenir sur l'enjeu de la mécanisation, le Conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux Monsieur le Ministre a rendu un rapport intéressant en 2021 sur la charge de mécanisation des exploitations agricoles. Dans leurs conclusions, les auteurs rappellent que ces charges de mécanisation peuvent représenter de 30 à 50% des charges totales et que le pouvoir de négociation des agriculteurs. Hé bien faible face à un marché fermé avec des prix en constante augmentation. Sur le conseil à l'achat, ils indiquent également que la plupart des organisations d'appui au développement peu à peu quitté ce domaine et il n'existe aujourd'hui que très peu d'outils d'aide à la décision pour aider les agriculteurs à raisonner leurs investissements et je pense que tout l'enjeu est là. Car oui, les agriculteurs ont indéniablement besoin de machines agricoles mais. Il y a un mais, ces achats doivent se faire de manière raisonnée et adaptée à leur exploitation. Et pour cela, je pense qu'ils ont davantage besoin d'un conseil indépendant que d'un crédit d'impôt qui le servira que d'argumentaire de vente aux producteurs et aux vendeurs de machines agricoles, la sur-mécanisation avec parfois des crédits très importants pour acheter des machines. Représente un risque bien plus concrets sur lesquels les pouvoirs publics devraient se pencher plus sérieusement. Merci. Merci monsieur le président, chers collègues. Sans nier que de nombreuses exploitations font aujourd'hui face à la transforme transformation des systèmes de production et que les outils de l'agro-équipement sont au coeur de cette transformation, il n'en demeure pas moins que la recherche d'optimisation des charges sociales et fiscales accélère bien souvent la prise de décision des agriculteurs et n'applique pas nécessairement une réflexion stratégique d'équipements. C'est un des constats du rapport. La charge de mécanisation des exploitations agricoles du conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux de 2021. Constat partagé par la Cour des comptes cet encouragement à l'investissement n'est pas sans lien avec des pratiques d'optimisation fiscale et sociale qui nuisent à la constitution de droits à la retraite des agriculteurs dans la mesure où elles réduisent le résultat comptable qui constitue l'assiette d'imposition et de cotisations. Il renchérit le montant des reprises et des installations et semble mal articulé avec les dispositifs destinés à pallier le coût croissant des équipements comme les pratiques de mise en commun des équipements par les exploitants. Exemple, la coopérative d'utilisation de matériel agricole, les achats groupés ou là seulement commun. Ou quand cela est pertinent. Le recours aux entreprises de travaux agricoles en outre aussi des investissements apparaissent indispensables pour réduire l'usage d'intrants et des énergies fossiles. Il faut par exemple recourir à des pulvérisateurs plus précis donc plus coûteux. Les avantages fiscaux ne sont pas toujours orienté vers des outils mécaniques ou d'aide à la décision qui s'inscrirait dans une dynamique d'activité agricole durable. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article, merci. Merci monsieur le président. Je comprends les arguments qui sont avancés par cet amendement de de suppression et je tiens. À rassurer ses auteurs par rapport aux arguments qui viennent des des d'être développé. L'article 5 ne vise pas à permettent d'acheter un tracteur à 150 ou 200 ou à 300.000 euros puisqu'à l'occasion de son passage en commission le crédit d'impôt de cet article. De cinq a été plafonnée à 20.000 euros donc ce crédit d'impôt et par ailleurs instituée pour une durée seulement 3 ans pour inciter les entreprises agricoles, notamment les plus modestes à investir. Je tiens aussi à rappeler que, malgré certaines pressions. Nous avons maintenu le crédit d'impôt car l'Avantage du crédit d'impôt par rapport à la défiscalisation et de permettre à des entreprises ayant un résultat modeste d'investir le cas échéant en se faisant rembourser le surplus évidemment. Si le montant du crédit d'impôt est supérieur aux résultats. Par ailleurs j'ai souhaité que ce crédit d'impôt puisse soutenir des des investissements également immatériel qui peuvent aussi remplir des fonctions sur la compétitivité et sur l'amélioration du changement et des transitions nécessaires, donc avis défavorable le ministre. Oui, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice. C'est un avis favorable sur cet amendement. Parce que nous avons un désaccord avec la proposition telle qu'elle est posée sur sur la question du crédit d'impôt, d'abord on est quand même toujours un peu paradoxaux les uns les autres, c'est-à-dire qu'on ne veut pas sur-transposition et parfois on on produit à chaque texte et on ne veut pas de niches fiscales et au fond on vient créer une niche fiscale supplémentaire. Bon, ça nécessiterait quand même qu'on essaye de se poser une question globale sur les questions fiscales qu'on aura à poser d'ailleurs madame la présidente. On en a déjà. On l'a déjà évoqué. Sur la question de la fiscalité de l'agriculture et est-ce qu'elle vient servir comme objectif. Et donc pour ce motif là je je profite pour livrer un sentiment général sur la question de l'investissement dont on a besoin l'agriculture. J'entendais parfois des propos sur la question de la mécanisation de la robotique. il y a pas de chemin autre à moins qu'on pensait être sur une île déserte que celui qu'on prend tous les pays agricoles du monde qui est celui de la mécanisation et la robotique qui dans beaucoup de cas, d'ailleurs à libérer les agriculteurs d'un certain nombre de contraintes physiques, enfin je veux dire, personne n'a envie ni ici ni ailleurs, j'imagine, de revenir à ce qui était l'agriculture nos mécanisé donc on a besoin de mécanisation, on a besoin d'investissements mais on n'a pas besoin de surinvestissement et 2ème élément, on a besoin, me semble-t-il de de se fixer comme objectif global d'éviter le sur-investissement et de d'orienter vers des investissements de transition. 2ème élément c'est qu'il faut qu'on pense, l'évolution des structures et peut-être d'accroître les structures collectives. Le sénateur du plomb évoqué. Alors je ne suis pas sûr que ça soit aussi. Aussi blanc et noir que ce que vous dites sur la question de l'investissement, il y a encore des gens qui investissent et d'ailleurs ils ont tout à fait le droit de manière individuelle. Il y a des structures d'investissement qui sont les Pumas. Il y a d'autres structures aujourd'hui qui ne sont pas forcément reconnus ou d'autres dispositifs qu'on aura besoin de travailler, y compris dans le texte. Que je serai appelé à à vous soumettre, c'est qu'est-ce qu'on fait de collectif qui ne soit pas forcément dans des structures collectives actuelles. On a besoin d'encourager le collectif mais il y a d'autres formes de collectif qui s'organise et donc essayons de ne pas imposer là aussi un modèle sur ces questions là et donc on a besoin de travailler sur quelque chose qui vient plutôt encourager la transition. Et deuxièmement, quelque chose qui Vienne plutôt encourager le collectif renforcer encore la question collective sous des formes qui sont un peu différentes, en particulier avec des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et par ailleurs il me semble que cet article 5, c'est pour ça qu'on est favorable à votre amendement. Et à celle à celui de votre collègue. qui est celui de votre collègue aussi Fabien Gay mais. Ça pourrait faire doublon d'abord avec des soutiens financiers qui sont prévues dans le cas de France relance puisque pour ce qu'on termine conversion aux agro-équipement, on est dans la transition de 121 millions d'euros, puis le guichet FranceAgriMer qui vient aussi. Aider. Et subventionner les la transition et les agro-équipements pour les agriculteurs qui veulent s'engager dans toutes les filières. Et puis cet outil fiscal viendra également peut être en double, en tout cas ça mériterait expertise avec le dispositif de déduction pourrait pas de précaution qui est un autre élément du du texte que vous présentez donc pour toutes ces raisons, je suis favorable à cet amendement et par voie de conséquence, même si je reprendrai la parole mais ça gagnera du temps. Et, et le président sera heureux, j'imagine. Je serai défavorable à tous les autres, parce que le le principe sur cet amendement-là c'est de dire qu'on est défavorable à l'article 5. Merci. Monsieur le Ministre donc je mais aux voit cet amendement de suppression 59 avec un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est pour. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Donc nous avons cet amendement en discussion commune 106 monsieur Oui, monsieur le président, Monsieur 1000. Chers collègues, j'ai déjà évoqué tout à l'heure à l'article quatre toutes les roses, les réserves que nous avions sur le soutien massif à l'investissement, qu'ils sont dans bien des cas nécessaire et utile pour les exploitations je pense notamment aux investissements qui permettent de mettre en oeuvre des alternatives aux engrais chimiques et aux pesticides, mais aussi à ceux qui permettent d'améliorer l'ergonomie et le confort de travail, notamment en élevage et en maraîchage, mais la politique actuelle de soutien massif à l'investissement encourage l'agrandissement des des exploitations. On l'a dit déjà, avec ses conséquences sur l'emploi, elle organise à leurs dépens la perte d'autonomie des agriculteurs. Comme la Cour des comptes. Nous pensons qu'il faut donc réorienter le soutien à l'investissement vers la mutualisation de matériel et c'est pourquoi nous proposons de réserver ce crédit d'impôt Okuma. Nous pensons aussi qu'il nous faut une politique ciblée sur la transition écologique. C'est pourquoi nous proposons de réserver ce crédit d'impôt aux alternatives aux pesticides, aux engrais de synthèse. Par ailleurs, nous sommes aussi convaincus que l'avenir de l'agriculture ne se joue pas seulement sur des investissements matériels ou numérique. Les échanges entre agriculteurs au sein des Civam des groupements en arrive en agriculture bio. Le système de mutualisation et d'organisation collective comme les services de remplacement comme Solidarité paysans Terre de Liens l'atelier paysan toutes ces initiatives reconnue par le code rural sous sous le terme dont var organisme national à vocation agricole et rural mais peu soutenues sont pourtant bénéfique pour notre agriculture, elle perd, elle permet aux agriculteurs de développer des solutions innovantes et collective pour gérer différemment l'ferme mettre en oeuvre des pratiques agroécologiques. Améliorer leur qualité de travail. Si cher collègue 2 amendements identiques, le 19 et le 54 le 19 il est descendu. 54 va être présenté. Madame Jouanno. Il est défendu le 19 de 54 Madame Losier. Merci merci président. Donc cet amendement revient donc sur l'article 5. Qui je le rappelle, met en place un crédit d'impôt. Et pour. Pour rebondir sur votre intervention, monsieur le Ministre. Je pense que justement les crédits d'impôts sont sont des outils pour bouster une politique publique. Alors après comment on le gère dans le temps il y a un vrai sujet. Mais aujourd'hui, face aux nombreux enjeux que nous avons largement évoqué notamment la réduction des coûts de production, l'amélioration de la compétitivité prix l'adaptation au changement climatique ou la lutte contre les aléas climatiques. Eh bien la mécanisation est un outil majeur au service des agriculteurs et en fait, cet amendement a pour objectif d'ouvrir ce crédit d'impôt explicitement aux entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers qui font face face à ces mêmes problématiques et à ces mêmes enjeux puisque nous avons là des entreprises polyvalente qui oeuvrent globalement dans l'entretien des espaces naturels, mais aussi en matière de défense des forêts compte l'incendie en matière de mise en oeuvre des eaux Elder et nous savons aujourd'hui, il y a un manque notoire d'entreprise pour agir et et et réaliser ces travaux absolument nécessaire pour la préservation de nos, de nos espaces, et pour la sécurité de nos concitoyens. Donc c'est-tu c'est une demande d'élargissement du dispositif. Crédit d'impôt. Merci de 90. Montaugé. Oui, merci Monsieur le Président, dans le, dans le même esprit, donc un crédit d'impôt de 20.000 euros. Au au maximum dans le but. Voilà, de réduire les les coûts de production. Dans la même perspective compétitive et pris compétitivité prix adaptation au changement climatique et on pense également comme ça vient d'être dit qu'il faut absolument que les les entreprises de travaux ruraux agricoles et forestiers

Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, c'est juste d'élargir tous les secteurs, parce que si on est sur un crédit d'impôt qui favorise par exemple les investissements concernant les aléas climatiques. L'aménagement en termes d'arboriculture et autres je pense qu'on peut aussi avoir la possibilité de l'ouvrir sur tous les secteurs agricoles.

notamment pour les organisations sociétaire. Nous tenons à rappeler que la course c'est la mécanisation et sur équipement des exploitations agricoles conduit bien trop souvent si je te dis tout à l'heure à des situations de surendettement parfois fatale à nos agriculteurs. En commission, conscient que cet article allait beaucoup trop loin et ne respectait pas le régime des minimise la rapporteure à plafonner le montant maximal du crédit d'impôt pour, je cite, limiter les éventuels effets d'aubaine, d'une part, ainsi que le coût pour les finances publiques. D'autre part, madame la rapporteure pour une fois nous partageons totalement et sans réserve aux préoccupations. C'est pourquoi pour les mêmes raisons. Nous proposons d'aller un peu plus loin dans votre démarche en diminuant ce plafond afin de s'assurer que ce crédit d'impôt ne soit pas un appel d'air du surinvestissement. Il y a de la spéculation qui ne bénéficiera pas aux agriculteurs. nous proposons donc de plafonner ce crédit d'impôt à 10.000 euros contre 20.000 dans le texte issu de la commission. Ça, c'est un président voilà expéditif. Alors je vais prendre un petit peu de temps. Pardon, Monsieur le Président pour donner l'avis de la commission donc sur l'amendement 106 de notre collègue Joël Labbé. Il a la il métamorphose en fait complètement le principe de ce crédit d'impôt qu'il a bel et bien déjà que pour objet d'accompagner les petites et les moyennes structures. Le la critique de la sur-mécanisation je l'ai dit et d'ailleurs notre collègue Jean-Claude Tissot la l'a redit à l'instant a déjà été traité en commission avec un plafonnement à 20.000 euros du crédit Je vous donne un exemple. À titre d'exemple, investissement dans des filets para-grêle en arboriculture rendu souvent nécessaire par l'augmentation des aléas climatiques. Coûte à peu près 15.000 euros l'hectare. Voilà un type d'investissement qui pourraient bénéficier de ce crédit d'impôt et qui me semble être de bon aloi vous mentionnez les cumin et d'ailleurs vous réduisez le crédit d'impôt Dumas les Pumas sont effectivement indispensables, elles sont très intéressantes. Et d'ailleurs elles sont intégrés dans ce dispositif qui est mis en place par l'article 5. Donc compte tenu du fait que vous métaphore métamorphosé complètement le crédit d'impôt, c'est un avis évidemment défavorable sur les amendements, 19 et 54 qui sont identiques, mais également 90 qui n'est pas tout à fait identique vous proposer d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt crédit d'impôt aux entreprises de travaux agricoles ou de travaux agricoles ruraux et forestiers. Nous savons que sur ce domaine là le défi actuel, notamment pour les forestiers et principalement la disponibilité de la main-d'oeuvre au car les métiers sont quand même assez pénible. C'est pourquoi je proposerai un à notre assemblée tout à l'heure de voter plutôt plusieurs amendements identiques visant à étendre le TO des à ces entreprises ce qui constitue, à mon avis une réponse qui est plus approprié. C'est donc une demande pour ces trois amendements de retrait ou un avis défavorable pour l'amendement de monsieur du plomb qui étend ce crédit d'impôt à à tous les secteurs d'activité, alors que le dispositif que nous proposons est destiné aux secteurs les plus intensifs en main d'oeuvre, c'est aussi un avis défavorable. Nous souhaitons que ce dispositif s'adresse à ceux qui ont le plus de désavantages en matière de main-d'oeuvre et c'est donc particulièrement plutôt les maraîchers plutôt les arboriculteurs plutôt tous ceux qui qui ont beaucoup de main-d'Oeuvres c'est. Voilà c'est un, un soutien particulier à ces entreprises agricoles et c'est aussi. Et je sens que Monsieur le Ministre attaque hein la bonne gestion des données publiques qui veut que l'on maintienne ce ciblage de crédit d'impôt donc c'est un avis défavorable, c'était quasiment un avis des. Favorable à l'amendement de notre collègue Jean-Claude Tissot qui vise à diviser par 2 le plafond du crédit d'impôt le je ne vais pas prendre le filet. Contre la grêle de l'arboriculture, mais il me semble que 20.000 euros est un est un chiffre raisonnable avis défavorable et bien sûr sur l'amendement rapporteur. Merci madame la rapporteure. Monsieur le Ministre, évidemment, vous avez envie de reprend la parole. Oui non non mais je ne veux pas ne pas tenir mon engagement. Juste dire je partage que. Parce que la la présidente m'inviter à être taquin. on a un certain nombre de dispositifs ou d'élargissement que vous proposez qui peuvent être aussi. Couvert par d'autres dispositifs, je pense à ce que nous faisons ce que nous avons fait dans France relance. Nous ce que nous faisons dans France 2030 et vous. Moi je pense qu'on a besoin dans le débat que qui se noue aujourd'hui qui démarre aujourd'hui de réfléchir aux dispositifs fiscaux au dispositif financier d'aide pour avoir quelque chose, soit un peu cohérent parce qu'on ne peut pas faire émarger sur 3 ou 4 guichets d'abord les agriculteurs nous diront c'est trop compliqué. J'ai trois ou quatre guichets. Même s'ils sont complémentaires. Et donc on a besoin, y compris pour la lisibilité d'avoir ces éléments-là Il m'a pas échappé que les sujets forestier étaient des sujets qui sont des sujets qui nécessitent aussi de se poser cette question là. Disons qu'en plus on est sur un texte au-delà de maintenir mon avis défavorable globale la question forestière est une question qui doit être prête à part. Disons que ce n'est pas de même nature, y compris en termes d'orientation. C'est une question de mécanisation tout court et et de matériel dont ont besoin, ce qui n'est pas la même chose que ce que je pensais la nécessité de transition par les matériels du modèle agricole. totalement polyvalente et qui émarge au guichet à agricole et vraiment j'insiste même si madame la présidente, vous avez raison, il y a une pénurie de main-d'oeuvre mais on est aussi sur des secteurs d'activités au a une forte pénibilité et où la mécanisation est absolument essentiel pour justement attirer de la main-d'oeuvre.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 32 avec 2 avis défavorable est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté de 124 de la commission. Avec un avis défavorable du gouvernement mais c'est un rédactionnelle. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il être adopté je mais voir l'article 5. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je vais suspend la séance elle sera reprise à 21h 30 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.